est reprise et l'ordre du jour appelle l'examen des crédits de la mission Anciens combattants, mémoire et Liens avec la nation et article 41 41 bis du projet de loi de finances, sa parole est à monsieur Marc Laménie, rapporteur spécial de la commission des finances. Ben Merci madame la présidente, madame la ministre, je salue ma collègue de la commission des affaires sociales, Josiane Guinness, mesdames et messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, les crédits de la mission Anciens combattants, mémoire et Liens avec la nation continue une baisse inexorable malheureusement liés à la démographie l'année 2023 donc que représente cette baisse particulièrement marquée de à hauteur de 161 millions d'euros les crédits, tombant à 1 virgule 9 milliards d'euros, due à la diminution, malheureusement, du nombre de bénéficiaires de pensions militaires d'invalidité et de la retraite du combattant, combinée à une revalorisation limitée de ses pensions se démarque par une revalorisation de droit commun qui doit s'élever à 4 pour 100 cette revalorisation reste inférieure à l'inflation de 2022 qu'elle a pour objet de compenser cependant cette approche globale cache un certain nombre d'éléments qu'il faut également souligner l'année 2022 a vu un renforcement particulièrement important de l'effort de la nation envers les harkis et autres rapatriés les crédits qui leur sont dédiés, c'est aussi un acte de respect de reconnaissance ont été multipliés par 4 compte entre l'exécution 2021 et la prévision pour 2023 les actions qui ne sont pas liées aux rentes versées aux anciens combattants sont globalement en hausse, et notamment les crédits dédiés à la politique de la pierre, soit l'entretien des tombes de morts pour la France, les nécropoles nationales et ainsi que les au lieu de la mémoire nationale du fait de la forte dimension de ces actions de plus, l'année 2023 ne prévoit plus de prélèvements sur la trésorerie dont le niveau est désormais faible de l'ONAC VG Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou l'opérateur principal de la mission sur lequel j'ai réalisé, je remercie notre administrateur ainsi que l'école les les les le, le personnel de la commission des finances pour ce travail d'engagement et les et Madame la Ministre, ainsi que l'ensemble de vos services pour la bonne coopération et collaboration donc une mission de contrôle budgétaire sur l'eau que je associe un autre opérateur de l'État, l'institution nationale de des invalides, enfin, le gain pour les finances publiques liées aux baisses de crédits de la mission est largement l'article 3 Quiès, c'était la première partie de la loi de finances, qui étend le bénéfice de la demi-part fiscale des veuves d'anciens combattants, représenter un coût de 130 millions d'euros lorsqu'il a baissé la condition d'âge de décès de l'époux soit à l'âge de 60 ans, or nous avons fait le choix en votant des amendements identiques au gouvernement, Madame la Ministre de la commission des affaires sociales et plusieurs de nos collègues de supprimer totalement cette condition d'âge de décès de l'époux ancien je serais intéressé Madame la Ministre, de connaître le chiffrage du dispositif qui résulte de ces amendements, la baisse de 160 millions d'euros de crédits sera donc compensé par le renforcement des dépenses fiscales sur la mission mais c'est des dépenses fiscales, c'est aussi la notion de respect et de de reconnaissance avec une des valeurs hautement symbolique pour l'ensemble du monde combattant, ainsi, s'il est possible de regretter la revalorisation toujours inférieure à l'inflation des rentes viagères la baisse globale des crédits ne doit pas non plus caché les efforts budgétaires consentis pour les harkis et autres rapatriés ainsi que ceux qu'ont consentis pour les veuves d'anciens combattants toute l'école tous les collègues sont aussi dévoués impliqué dans nos départements et territoires respectifs sur le notion de devoir de mémoire de coopération avec l'éducation nationale en particulier, Jocelyne Guinness, préside le groupe d'étude au Sénat du du monde combattant et je crois que c'est aussi des valeurs de reconnaissance, de respect que nous avons aussi pour l'ensemble de nos associations patriotiques et de mémoire nos porte-drapeau, c'est les sous qui se dévouent réellement pour la mémoire, donc, et est impliquée aussi les jeunes donc le lien fort avec l'éducation nationale, donc on en conclusion, je vous invite, chers collègues à voter les crédits de la mission et j'en profite pour remercier l'ensemble des services du Sénat et de votre ministère, Madame la Ministre, merci à tous. La parole est La parole est à madame la rapporteure pour avis de la commission des affaires sociales, madame Jocelyne Guidez. Madame la ministre. Mon cher Marc, monsieur le rapporteur spécial, mes chers collègues, malgré la baisse de 7,4 % des crédits de la mission en raison d'une diminution des bénéficiaires des prestations service aux anciens combattants, le budget prévu pour 2023 permettra de revaloriser de 3,5 pour 100 des pensions militaires d'invalidité et la retraite du combattant après une revalorisation exceptionnelle de 7 % en 2022, je salue la décision du gouvernement de répercuter dès 2023 la hausse de la rémunération des fonctionnaires sur le point de PMI, alors que les règles de calcul aurait conduit un en tenir compte, qu'en 2024 compte tenu de l'inflation, cette revalorisation, qui représentera un coût de 41 millions d'euros demeure toutefois insuffisante pour soutenir les pensionnés, nous devons donc être attentif à ce que les pensions servies aux anciens combattants ne subissent pas le même décrochage que celui constaté entre 2005 et 2021, mais là-dessus, je vous fais confiance, je veux saluer l'adoption en première partie du PLF 2 l'amendement de la commission des affaires sociales qui accordent une demi-part fiscale au conjoint survivant de plus de 74 ans, quelle que soit l'âge du décès d'anciens combattants, cette mesure de justice renforcera le soutien de la nation, aux familles d'anciens combattants et je sais aussi que ça a été votre combat, madame la ministre, je m'interroge toutefois sur l'âge à partir duquel le conjoint survivant d'un ancien combattant peut bénéficier de cette demi-par le fait qu'ils doivent attendre ses 74 ans, ne me paraît pas justifié sa tâche ne correspond à aucune autre ouverture de droit, il pourrait être envisagé d'accorder cette demi-part des 67 ans, soit l'âge du taux plein pour la retraite, alors je sais que ça a un coût, mais je pense qu'il va falloir faire enfin bon, faut savoir où on va avec ça, combien ça peut coûter, on y reviendra, je n'ai pas déposé d'amendement parce que je pense qu'il faut qu'il y ait une discussion autour de tout ça, nous devons donc poursuivre nos travaux sur ce dispositif afin d'en évaluer les effets et de le rendre à terme plus juste pour les enfants, l'ensemble des familles de combattants, soulignant que l'augmentation de 3,8 millions d'euros de la subvention versée à l'ONAC VG permettra de financer la pérennisation des maisons à tous qui offre un accompagnement très utile aux blessés psychique et à leurs familles, et là je tiens vraiment à remercier le gouvernement qui vont construire une supplémentaire, le maintien de 25 millions d'euros de la dotation d'action sociale de l'ONAC DG malgré la baisse du nombre d'anciens combattants, permettra à l'Office de soutenir ses ressortissants en difficulté d'accompagner les pupilles de la nation et les victimes de terrorisme, les moyens consacrés au armée jeunesse à la mémoire progresseront pour assurer le financement des journées de défense et de citoyenneté, l'entretien de plus dur de guerre et de lieu, de la mémoire nationale ainsi que la commémoration lié au 80ème anniversaire de la seconde guerre mondiale, or ces moyens alloués à la jeunesse et la mémoire devrait progresser bien plus significativement en tout cas je l'espère, il me paraît nécessaire pour le musée consacré au monde combattant soit à terme sanctuariser et que les actions en faveur du lien armée-nation et de la mémoire combattante soit renforcée, les nouvelles générations du combattant de combattants, dont les besoins évoluent devront être accompagnés par l'ONAC en outre fils pourrait renforcer les Liens armée-nation en valorisant l'engagement citoyen en faveur du monde combattant et en soutenant davantage la transmission de la mémoire notre cohésion nationale en dépend, alors que les témoins des grands conflits qui ont marqué notre pays disparaissent progressivement au nom de la commission des affaires sociales, je vous invite à adopter les crédits de la mission et j'aimerais remercier bien sûr mon collègue Marc avec qui je travaille vraiment en bonne cohésion et avec aussi, madame la Ministre, où on est toujours, comment dire, à discuter, échanger et vouloir avancer ensemble, c'est ensemble qu'on ira beaucoup plus loin, merci à vous tous. Bien, nous allons passer l'addition générale je vous rappelle que le temps de parole attribués à chaque groupe comprend l'intervention d'addition générale et l'explication de vote et on commence par Madame Katia pour polie pour quatre minutes pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste. madame la présidente, madame la ministre madame et monsieur les rapporteurs, chers collègues, à l'heure d'examiner le budget relatives à aux anciens combattants et plus encore à l'heure où la guerre est aux portes de l'Europe, je veux rendre hommage à ces femmes et ces hommes qui se sont battus pour que nous soyons libres si les derniers résultats électoraux inquiète au groupe CRCE nous faisons le voeu de construire une société progressiste et humaniste chers collègue alors que les anciens combattants, été de nouveau doté d'une Ministre délégué, le gouvernement a décidé de redonner la prérogative des anciens combattants, un secrétariat d'État si cela peut paraître être un détail : nous sommes convaincus qu'un ministère en tant que tel demeurera utile tant que les contentieux ne seront pas totalement réglé, c'est le souhait des associations d'anciens combattants à la lecture du rapport budgétaire relative à cette mission, nous constatons une fois encore une baisse du budget, elle atteint 154 millions d'euros pour 2023, soit une baisse de 7,4 % par rapport à 2022, une fois encore, cette baisse de crédits est justifiée par la diminution naturelle du nombre de bénéficiaires des pensions militaires d'invalidité de la retraite du combattant, madame la secrétaire d'État, je souhaite me faire le porte-parole des associations pour vous dire qu'il suffirait de garder un budget constant d'une année sur l'autre pour satisfaire pleinement les revendications du monde combattant, toutefois je veux noter 2 avancée majeure : la première concerne les Harkis, avec une augmentation de 3 millions d'euros de leur dotation portant sur le droit à réparation du fait des préjudices subis en raison de l'indignité et de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français, la seconde était certainement la plus attendue, je veux bien entendu parler de l'octroi du bénéfice de la demi-part fiscale pour les veuves, quelle que soit l'âge de décès de l'époux, il s'agissait d'une discrimination par l'âge, contraire à nos principes constitutionnels, nous nous félicitons donc de ces 2 mesures, en revanche, au rayon des insuffisances et manque la valeur du point de PMI s'établira au 1er janvier 2023 à 15 58 contre 15 05 euros en 2022 en tout état de cause, cette augmentation de seulement 3 52 % est largement inférieur à l'évolution des prix à la consommation,

dans ces conditions, un rattrapage du retard constaté sur la valeur du point de PMI, serait une bonne mesure, comme vous le savez, la valeur du point PMI n'est pas indexé sur l'inflation, mais sur l'indice d'ensemble des traitements bruts de la fonction publique de l'État, sans même revenir sur le passé et l'érosion du pouvoir d'achat des anciens combattants, résultant d'une inflation et d'un gel quasi totale de l'indice entre 2012 et 2018, la situation apparaît préoccupante, madame la secrétaire d'état, il est impératif de rattraper le retard rapidement, y compris en mettant un pied sur un calendrier de rattrapage, je vous remercie.

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur, madame la rapporteure chers hein Jocelyn, mes chers collègues permettez-moi de saluer le travail de nos rapporteurs Marc Laménie mais également ma collègue Jocelyne qui Days, dont je salue le sérieux de son travail et la qualité de ses analyses, mes chers collègues, nous avons la lourde tâche dans le cadre d'un projet de loi de finances d'octroyer de la fiscalité et des moyens à l'inestimable sacrifice au service de la patrie par le sang versé et ce que nous devons à celles et ceux qui victimes ou persécuté doivent être indemnisés, disons-le, la trajectoire par le gouvernement et porté par Madame la Ministre, Patricia Mirallès est acceptable, voire même encourageante, ce que nous disent les chiffres, je pense à la baisse du nombre de bénéficiaires de pensions militaires d'invalidité et de prestations octroyées aux anciens combattants, du fait de l'érosion démographique, c'est que la guerre, les guerres françaises s'éloigne et que le devoir de mémoire n'est plus qu'urgent, ce que nous disent les Français et les associations, c'est que le devoir de mémoire ne doit oublier personne, et être le plus juste possible, y compris dans les moyens alloués aussi ce que nous pouvons observer, c'est que la mission Anciens combattants, mémoire et Liens avec la nation est un point de bascule dont nous devons avoir conscience, les demandes de financement de cette mission seront d'année en année élargit paradoxalement à mesure que les guerres s'éloigne du fait de l'élargissement du Champ de reconnaissance de ce que doit une nation à ses combattants à leurs familles et aux victimes et des moyens que l'État doit mettre en place pour instaurer du lien entre son armée et son peuple, de plus, l'évolution des définitions que nous déterminons par exemple de ce que veut dire être victime être mort pour la France du du Champ d'application que revêt la mémoire ou les mémoires l'évolution du nombre de jours fériés, auront des conséquences notables sur les Budgets à venir à louer à la mission Anciens combattants, mémoire et Liens avec la nation lorsque pour la première fois cette année, nous décidons que le parcours du soin complet et complémentaire avec le service de santé des armées des maisons Athos prennent aussi en compte les blessures psychiques en accompagnant aussi les familles de militaires souffrant de ces troubles, nous faisons évoluer la définition et la reconnaissance de ce qu'est une blessure, autre exemple, la reconnaissance des préjudices en faveur des harkis, supplétifs et rapatriés témoignent aussi de la finement avec lequel l'État prend mieux en compte la question des préjudices je salue d'ailleurs l'action du gouvernement ce sujet car en un an, les moyens de la politique de reconnaissance et de réparation en faveur des harkis ont presque été le le montant moyen attribué par bénéficiaire est en moyenne de 8784 euros depuis les premières auditions des harkis, Madame la Ministre, que de chemin parcouru et c'est tant mieux, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre voit le montant de sa subvention pour charges de service public, augmenté de 3 8 millions d'euros pour l'année 2023 pour supporter non seulement le travail de la commission nationale indépendante sur les harkis, mais aussi la revalorisation du point d'indice de la fonction publique, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre voit aussi sa dotation d'action sociale de 25 millions d'euros préserver cette dotation est essentielle afin de verser des aides financières aux anciens combattants à leur conjoint survivant mais aussi de soutenir les pupilles de la nation, comme l'a rappelé ma collègue rapporteure Jocelyne 10 Days l'ONAC VG doit pouvoir avoir les moyens d'élargir et de développer ces actions destinées à promouvoir les Liens entre armée Nation en valorisant l'engagement citoyen auprès de nos armées, Jean Faure mille aussi le veut par ailleurs, je tiens à saluer les augmentations du budget relatives au lien armée jeunesse notamment le soutien au service militaire volontaire, le financement des journées de défense et de citoyenneté les JDC ainsi que la promotion du lien armée jeunesse des classes de défense et des cadets de la Défense, faisant progresser les crédits alloués de 4 % en 2023 pour atteindre une enveloppe de plus de 24 millions d'euros concernant la politique mémorielle, les crédits demandés par la politique de mémoire progresse de 17 2 % par rapport à 2022 le crédit de financement des actions de mémoire était en 2022 de 17 85 millions d'euros, certes en légère hausse ce budget n'était pas suffisant et il conviendrait de savoir quelle aurait été la volonté du gouvernement pour 2023 hors inflation, en matière de financement des actions mémorial j'en viens maintenant aux crédits en faveur des anciens combattants aux pensions militaires d'invalidité et aux retraites de combattants qui constituent l'essentiel du budget alloué à la mission concernant la retraite du combattant là aussi la diminution démographique du nombre de bénéficiaires aujourd'hui, en moyenne, âgé de 85 ans est estimé à 7 % en 2023 cette diminution permet notamment à l'État de financer différemment les pensions militaires d'invalidité et de revoir sa politique en matière d'octroi des demi-parts, nous devons reconnaître que le gouvernement en fait de choix essentiels répercuter la hausse de 3 5 % du point d'indice de la fonction publique en juillet 2022, sur le point de PMI de janvier 23 au lieu de 24 41 millions d'euros supplémentaires qui permettront de mieux soutenir les anciens combattants, face à la hausse des prix, l'octroi de la demi-part supplémentaire pour le calcul de l'impôt sur le revenu, je tiens ici à saluer et remercier la rapporteuse, une fois de plus, Jocelyne qui Days qui a proposé par amendement que la demi-part fiscale supplémentaire soit accordé au conjoint survivant, quelle que soit leur âge et je te soutiens ces évolutions ainsi dans le cadre de ce projet de loi finances 2023, le groupe Union centriste que je représente pour cette mission votera favorablement l'adoption des crédits de la mission Anciens combattants, mémoire et Liens avec la nation, je vous remercie. pour le groupe RDSE. Madame la présidente, madame la ministre madame et monsieur les rapporteurs, mes chers collègues, chaque année, une réalité s'impose : celle de la disparition des anciennes générations de feu comme l'on dit ainsi en écho à cet état de fait, les crédits de paiement demandé en 2023 pour la mission Anciens combattants, mémoire et Liens avec la nation sont donc en baisse de 7 4 % si le budget de l'État se doit d'accompagner la diminution du nombre de bénéficiaires des pensions et prestations d'anciens combattants, il se doit cependant de demeurer en capacité de proposer à un haut niveau de réparation corollaire à notre au niveau de reconnaissance. Les dispositifs de la ami. Si on ne relève pas de leur du soutien, mais de celui du devoir, devoir moral intangible envers tous ceux et toutes celles qui ont consenti des sacrifices au profit du destin collectif de la France, si j'ai la conviction que les marges budgétaires dégagés mécaniquement par le paramètre démographique doivent être l'occasion de renforcer et de compléter les mesures existantes dans cette perspective, je me réjouis des avancées portées par le projet de loi de finances pour 2023, je pense notamment à la revalorisation des pensions militaires d'invalidité au 1er janvier 2023, le calcul de la valeur du point PMI effectuée en fonction de l'indice d'ensemble des traitements de la fonction publique d'État et mise en oeuvre en 2005 se relève non satisfaisante en période de forte inflation, je salue donc la décision du gouvernement de répercuter dès janvier, la revalorisation de droit commun de 4 % du point d'indice au 1er janvier 2023, il faudra rester cependant vigilants face à un niveau d'inflation sans cesse révisés à la hausse pour l'année prochaine, dans ce contexte, l'extension de l'octroi d'une demi-part fiscale au conjoint survivant d'anciens combattants se également de nature à soutenir le pouvoir d'achat de ses bénéficiaires, nous avons décidé au Sénat lors de l'examen des articles de la première partie d'améliorer le dispositif proposé par nos collègues députés, la suppression de la condition d'âge de décès de l'époux ancien combattants pour le bénéfice par sa veuve d'une demi-part fiscale à ses 74 ans, et pour nous, une mesure d'équité qui était très attendue par le monde combattant, nous souhaitons qu'elle soit conservés par le gouvernement, si la mission met également en oeuvre les dispositifs issus de la loi du 23 février 2022 un texte par lequel la France reconnaît les conditions d'accueil et de vie indigne des harkis et de leurs familles, rapatriés d'Algérie après les accords d'Évian de 1962 la question reste toutefois ouverte s'agissant des personnes qui ont vécu de façon tout tout aussi indignes en dehors des camps et des hameaux de forestage je compte sur le 1er rapport de la commission dite Bockel attendu au printemps 2023 pour nous apporter un éclairage quant à la justesse des critères retenus dans la loi précitée, au sens de la mission, le programme 158 entièrement dédié à l'indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la se Seconde Guerre mondiale, voix et c'est normal, là aussi, ses moyens, suivre la baisse tendancielle du nombre de ses bénéficiaires, aux côtés de la politique de réparation, il est bien entendu fondamental de poursuivre les actions en direction de la mémoire, je suis fier d'avoir représenté le Sénat à Auschwitz le 7 novembre dernier lors de la cérémonie d'hommage aux victimes de la tragique nuit de cristal, une manifestation qui a réuni des délégations de parlementaires du monde entier la résurgence d'un antisémitisme banalisé et dangereux, doit nous conduire à être particulièrement soucieux du devoir de transmission aux jeunes générations, notamment sur ce qu'a représenté la déportation et les camps de la mort, l'ignominie absolue au fil du temps, les témoins ou les ayants droit des grands conflits disparaissent, il nous appartient donc de conforter la politique de mémoire qui concentre et je le regrette vivement, seulement 1 virgule un % des ressources du programme 169 de ce que, de 14 comme les avait qualifiés Maurice Genevoix jusqu'à nos soldats en OPEX opérations extérieures, sans oublier nos valeureux combattants de l'ombre que l'année 2023 mettra à l'honneur autour de la figure de Jean Moulin, aucune des victimes de la guerre ne doit être oublié dans le Champ de nos actions, la mémoire dans doit s'entretenir le groupe RDSE votera favorablement pour les crédits de la mission, je vous en remercie. Madame la présidente, madame la ministre, madame, monsieur, les rapporteurs, chers collègues, celui qui ne sait pas d'où il vient, ne peut savoir où il va, car il ne sait pas où il est en ce sens, le passé et la rampe de lancement vers l'avenir, cette citation résume assez bien la mission budgétaire que nous examinons ce cet après-midi, mais aussi et surtout les enjeux qu'elle ton plus que jamais à l'heure où ce qui nous rassemble, semble se réduire à une portion congrue, tant les tensions qui agitent notre société oublions ces repères sont importantes et diverses faire vivre cette mémoire collective revêt une dimension toute particulière, se souvenir de notre histoire avec lucidité mais sans fausse honte avec un orgueil mais sans méchanceté, se souvenir de ceux qui ont combattu, parfois jusqu'au sacrifice ultime est fondamental, nous le voyons dans les communes de France commémoration après commémoration ou cette flamme doit être entretenu ou cette flamme doit être transmise aux générations suivantes : et si la mission Anciens combattants, mémoire et Liens avec la nation voit ses crédits baisser de manière constante, année après année, l'année 2023 se démarque par l'ampleur de la baisse, comme l'ont rappelé les rapporteurs de cap symbolique sont franchi cette année, les crédits de la mission sont désormais inférieures à 2 milliards d'euros et pour la première fois le montant consacré par l'État à la retraite du combattant est inférieur à celui qui est consacré à la demi-part fiscale des anciens combattants et de leurs principal crédit d'impôt en faveur des anciens combattants et lu ici l'amendement de la rapporteure adopté dans la première partie qui élargit encore le dispositif ainsi les crédits affectés au pension viagère la retraite du combattant et des pensions militaires dans mes Didite poursuivent leur inexorable baisse tant en valeur absolue que rapporté à l'inflation, la revalorisation exceptionnelle au 1er janvier 2022 du point d'indice des pensions militaires d'invalidité 10, PMI n'a pas atteint son objectif de rattraper l'effet de l'inflation entre 2018 et 2021 à cause d'une hypothèse d'inflation trop fait pour 2021 d'autant moins que le point d'indice indexé sur les rémunérations publiques décroche face à l'inflation depuis 2012, de la même manière, la revalorisation de droit commun de 4 % vont avoir lieu au 1er janvier 2023 est inférieure à l'inflation de l'année 2022 les crédits des autres actions sont au contraire en hausse notamment, mais pas que, en raison de l'inflation, c'est le cas pour le budget de la Journée défense et citoyenneté qui connaît une légère hausse, millions d'euros, du fait d'un non plus important de jeunes pour l'accord 2023, bien que l'année 2023 marque un retour à la normale pour le fonctionnement de la JDC le coût moyen par jeune devrait rester stable par rapport à 2022, les crédits du service militaire volontaire sont eux stable dans un cas comme dans l'eau, ces augmentations sont peu significatifs car l'immense majorité, plus de 75 % des crédits effectivement utilisée pour ces dispositifs n'apparaît pas dans les crédits de la mission Anciens combattants et sont supportés par la mission Défense le Fonds social européen et par des collectivités territoriales, j'y reviendrai pour résumer les dotations la mission sont installés sur une trajectoire fortement dès son nom en ce qui concerne les actions de la budgétisation initiale le PLF pour 2023, bien qu'il comprenne quelques revalorisations liées à l'inflation qui n'inverse pas cette tendance, cette revalorisation ne fait que que limiter l'incidence budgétaire de la réduction inexorable de la population des bénéficiaires des rentes viagères constat s'appliquant à celles relevant du programme 169 comme revenons du programme 158 causée par l'âge très avancé d'une majorité des bénéficiaires, les rapporteurs ont ainsi appelé à l'adoption des crédits de la mission, appel auquel mon groupe souscrit mais qu'il me soit permis de rappeler que nous examinons cette mission à quelques encablures du bruit des bombes et des cris qui résonne en Ukraine sur un continent ayant déjà connu tant de guerres et de souffrance, cela appelle donc 2 principales observations, l'un des enseignements de la guerre en Ukraine et l'importance fondamentale des forces morales de la nation dans ce contexte, une réflexion est engagée dans le cadre de la prochaine LPM sur le rôle et le redimensionnement des réserves, il serait donc intéressant qu'on parallèle notamment dans le cadre de la généralisation annoncée du service national universel, une réflexion plus poussée soit menée sur les moyens et les outils les plus efficaces pour en créer et renforcer le lien armée jeunesse car force est de reconnaître que celui-ci fait encore trop largement défaut alors qu'il est pourtant la première brique de ce lien armée-nation dont on redécouvre aujourd'hui le caractère fondamental la baisse tendancielle des crédits de la mission, porté par la démographie déclinante des bénéficiaires des différentes allocations de reconnaissance de la nation pourrait permettent de dégager des marges de manoeuvres supplémentaires à cette fin, l'autre enseignement et la faiblesse du nombre d'armes opérationnelles et des munitions qui leur sont dévolues dont dispose l'armée française, nous l'avons vu avec l'envoi des canons Caesar, or son budget important mais justifie au regard des menaces et souvent la source de dépenses qui ne devrait plus le palu directement imputés comme la JDC le CMV cet arrangement budgétaire m'apparaît n'efface d'abord en terme de lisibilité, mais aussi et surtout car ces crédits lui sont indispensables, par souci de clarté et de sincérité sur les moyens effectivement attribués à la défense nationale, les crédits mobilisés pour ces 2 dispositifs s'il restait opérée par le ministère des Armées devrait ainsi intégralement relever de la mission Anciens combattants, mémoire et Liens avec la nation, cette double action : le renforcement des moyens et des outils consacrés à la jeunesse et à la politique de mémoire grâce à des crédits stable et surtout sortir certaines dépenses du budget de la mission Défense me semblait des pistes nécessaires à explorer, je vous remercie. Merci, la parole est à Madame Vanina Paoli-Gagin pour quatre minutes pour le groupe des indépendants. Madame la présidente, madame la Ministre, méthane et messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, Reconnaissance de la nation en faveur du monde combattant, transmission de la mémoire, renforcement du lien entre l'armée et la nation, indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie commis pendant la Seconde Guerre mondiale, les objectifs poursuivis par cette mission nous oblige et l'examen de ces crédits nous invite à une certaine solennité. Mais lister les programmes prévus par cette mission ne suffit pas en dire toute l'importance, car l'essentiel n'est pas là l'essentiel, c'est le soutien que l'État apporte à tous les hommes et toutes les femmes qui sont prêts à donner leur vie pour la nation, les crédits de cette mission finance principalement, vous le savez, mes chers collègues, des pensions, vous avez des prestations destinées aux anciens combattants, ils évoluent donc en fonction du nombre de bénéficiaires, cela a été dit, parce que le nombre des anciens combattants diminue, pour des raisons démographiques, ces crédits baissent encore cette année, ils s'établissent un virgule 9 milliards d'euros pour 2023, soit une baisse de plus de 7 % par rapport à la loi de finances initiale pour 2022 je tiens néanmoins à saluer un certain nombre d'avancées, la dotation créé par la loi de reconnaissance de février 2022 prévu pour le dispositif de réparation à destination des harkis et de leurs familles et portée à 60 millions d'euros, ce montant représente une augmentation de plus de 33 % par rapport à 2022 les crédits consacrés à la politique de la mémoire augmente de 3 millions d'euros, cette hausse permettra de financer des travaux de restauration nécessaire pour préserver notre Patrimoine mémoriel je salue cet effort important conserver ses lieux de transmission en bel état, c'est en effet soigner la mémoire que nous livrons aux générations futures. Je tiens également à saluer la progression des moyens consacrés aux opérateurs accompagnant les combattants et les blessés de guerre, cette progression est légère, certes, mais c'est une progression tout de même pour l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, cette augmentation est la bienvenue, elle permettra de supporter la revalorisation du point d'indice de la fonction publique, elle permettra aussi d'assurer le fonctionnement de la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et leurs familles, cette hausse permettra également de financer la pérennisation des maisons à c'est un dispositif expérimental de grande valeur qui procure un soutien aux blessés psychologique désarmé et je me réjouis que leur accompagnement souhaite ainsi renforcer Madame la Ministre, mes chers collègues, sur l'ensemble des crédits de la mission, seuls les crédits liés aux allocations viagères de la mission connaissent une baisse en 2023, mais cette baisse et là encore principalement liée à la démographie des bénéficiaires pour le reste, tous les crédits des autres actions sont en hausse aussi ce budget, nous, me semble-t-il, répond aux attentes des anciens combattants et le groupe les indépendants votera les crédits de cette mission, je vous remercie. Merci madame, la parole est à Madame Raymonde Poncet Monge pour le groupe Écologie Solidarité territoire et pour quatre minutes. Madame la présidente, madame la ministre madame et monsieur le rapporteur, chers collègues, la mission Anciens combattants, mémoire et Liens avec la nation voit ses crédits diminuer comme chaque année, mais plus que chaque année, cela s'explique bien sûr par la diminution du nombre de bénéficiaires mais justement il faudrait légèrement accroître le nombre des bénéficiaires, car certains harkis attendent toujours de bénéficier de ces crédits 22 supplétifs de statut civil de droit commun, attendent toujours une aide de seulement 4150 euros, cette question se pose chaque année et chaque année, le gouvernement avance un certain nombre d'arguments contestable mesure non applicable car il n'existe pas de base juridique impossibilité des mesures rétroactives, ou encore : avis défavorable du Conseil d'État et de la Cour européenne des droits de l'homme, les amendements parlementaires fournissent une base juridique à cette extension, pourtant la jurisprudence du Conseil d'État relative à la désignation explicite ou implicite des bénéficiaires d'une mesure adoptée par le Parlement en est en leur faveur, pourtant, enfin, le Conseil d'État et le CD CEDH n'ont pas rendu de tels jugements nous parlons ici de seulement quelques dizaines de milliers d'euros d'ailleurs ce que demandent ces hommes, ce n'est pas une aumône ou le suivi social que le ministère des Armées met en place, c'est la reconnaissance aussi nous remercions le rapporteur Marc Laménie t'avoir déposé un amendement en ce sens et pour lui donner plus de force, nous nous sommes permis de le déposer à l'identique, vous avez tant à si le gouvernement à lever le gage et à conserver l'amendement lors de la nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, sinon ces personnes vont inexorablement disparaître sans jamais avoir été reconnu par l'État en 2019, le Parlement a élargi aux veuves de plus de 74 ans, le bénéfice d'une demi-part fiscale supplémentaire à la condition que leurs maris décédés soit lui-même titulaire de la carte du combattant ou d'une retraite du combattant mais quid des veuves de moins de 74 ans, cet effet de seuil crée crée une rupture d'égalité malvenu, le Sénat a corrigé cela par amendement lors de l'examen de la première partie et nous nous en félicitons de la même manière, nous invitons le gouvernement à conserver cet ajout à l'Assemblée nationale, nous nous interrogeons aussi sur les crédits de la Journée défense et citoyenneté qui n'augmente que d'1 1000000 d'euros, alors que l'année 2023 doit marquer le retour à la normale après 3 années de pandémie ainsi la dépense par participant devrait rester la même qu'en 2022 hou la JDC étaient le plus souvent réduites de moitié, comment, avec un tel budget organiser correctement séjourné ou les jeunes Français, Françaises et Français doivent découvrir les enjeux géopolitiques qui conduisent la France a développé un appareil de défense les caractéristiques de ce dernier, effectuer des tests de langue française, à prendre les gestes de premiers secours et suivent une formation de sécurité routière. un mot de mémoire, pour finir, alors que les derniers poilus se sont éteints, tout comme les derniers compagnons de la Libération, la question de la transmission de la mémoire des guerres mondiales, et plus largement de la mémoire du 20ème siècle devient de plus en plus prégnante l'État bien- sûr ne remplacera jamais la transmission qui pouvait s'opérer par les témoins Directs du siècle passé, néanmoins, il est temps d'envisager une nouvelle ambition de politique mémorielle tourné vers les jeunes générations pour conclure madame la Ministre, le groupe écologiste solidarité territoires votera les crédits de la mission Anciens combattants, telle que modifiée, je l'espère, par l'amendement de notre rapporteur. Merci, la parole est maintenant Monsieur André Gattolin pour le groupe RDPI. Madame la présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, l'heure où la guerre fait rage à l'Est de l'Europe dans un mélange de nouvelles technologies et de guerre de positions qui nous rappelle les pires moments de la première guerre mondiale à l'heure où d'aucuns s'interrogent sur la nécessité de sacrifier un peu les dividendes tirés de 70 années de paix pour défendre notre liberté et nos valeurs fondatrices alors où les derniers combattants de la Seconde Guerre mondiale s'éteignent comme avant eux lors est née de la première guerre mondiale, le travail de mémoire n'est décidément pas un luxe dans notre société, emporté par l'immédiateté et l'hypertrophie du présent au détriment du regard méthodique peu porter sur notre passé et de la volonté aussi de se projeter dans le futur contente, a jugé trop incertain, le travail de mémoire n'est donc pas qu'aux commémorations événementiel, le temps d'une journée pour retourner dès le long de vingt aux affaires courantes quand les repères s'affaiblissent et que l'avenir paraît menaçant, il est indispensable de savoir d'où nous venons pour savoir où nous voulons aller ensemble, concrètement, il convient ici de dans le cadre de ce débat budgétaire de saluer l'augmentation de 20 % des montants qui seront l'an prochain, consacré à la mémoire 2023 et 2024 en effet marqueront des anniversaires particulièrement important et cet effort budgétaire et bienvenue et puisque nous parlons de la seconde guerre mondiale je veux ici, vous remercier, Madame la Ministre, pour votre présence le 19 août dernier à Dieppe, à l'occasion du 80ème anniversaire du du raid allié de 1942 qui vit malheureusement la mort et la déportation de milliers de jeunes Canadiens souvent engagés volontaires, est venu sur notre continent, comme déjà leurs aînés en 1914 pour défendre notre liberté et nos valeurs communes, le prix du sang payer par nos concitoyens ne doit jamais être oubliée, il ne faut pas non plus oublier le sang versé par nos Zannier et tous les peuples du monde entier qui se sont battus à ne compter côté parfois en lieu et place de nos propres troupes, c'est avec ces briques mais Muriel du passé que nous solidifiant au long cours, nos relations avec des nations qui ont si activement contribué à notre histoire et à notre liberté, j'étais au début de ce mois à Ottawa pour assister à la projection au musée de la guerre de Canadiens du documentaire du Français Laurent Mathieu sur la mémoire du raid de Dieppe, un travail exigeant, très apprécié de nos amis canadiens et je peux témoigner ici combien ce type d'engagement Mauriel cette reconnaissance collective n'en M2 l'événement troupes oublié de nous concours intensément à la qualité des relations que nous entretenons entre nos 2 pays, le travail de mémoire consolide le présent et devient ainsi un travail commun d'échafaudage de l'avenir à ce sujet, je formerai madame la ministre, et pour conclure de voeux, le 17 mai 2024, cela fera 80 ans que Félix Eboué, 3ème, compagnon de la Libération nous aura quittés panthéonisé depuis 1949 il demeure cependant trop méconnu de nombreux de nos concitoyens, même la place qui porte son nom, ici à Paris continue, avec la complicité involontaire de la RATP à être usine réellement dénommée place Daumesnil, faire savoir à nouveau aujourd'hui l'engagement exceptionnel de Félix Eboué dans la France libre serait je crois reconnaître aussi l'apport immarcescible de la Guyane à notre pays, enfin, discrète, la diaspora indienne qui compte plus de 200000 habitants en métropole et bien davantage dans nos territoires d'outre-mer, hé bien pendant la première guerre mondiale et furent plus d'un 1000000 de sa à s'engager auprès des alliés et plus de 120000 à combattre dans l'est de la France, là encore, leurs descendants, se battent pour leur mémoire, de notre nord de ne pas les oublier pour conclure je dirais bien évidemment que le groupe RDPI votera en faveur des Budgets de cette mission, je vous remercie. Merci madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mesdames et messieurs les rapporteurs, c'est un immense respect pour ceux qui se sont battus, qui se battent encore pour la France, ici même au à l'étranger et c'est avec ce respect que j'étais revient ici au nom du groupe socialiste, écologiste et républicain sur le projet de loi de finances de la Mission interministérielle Anciens combattants, mémoire et Liens avec la nation cette mission budgétaire se veut la traduction financière de la solidarité et de la reconnaissance de la nation envers les militaires et les anciens combattants en raison de leur engagement ou de leur sacrifice, la Mission interministérielle Anciens combattants, mémoire et Liens avec la nation est une passerelle entre la société civile et le monde combattant, elle est également l'occasion de créer des Liens intergénérationnels qui sont fondamentaux pour le devoir de mémoire et la cohésion sociale, cette mission s'articule de de programmes complémentaires depuis le PLF 2022 le programme 69 Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et Liens avec la nation et le programme 158 et d'armes nisation des victimes de persécutions antisémites et les actes de barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale,

passe en dessous de la barre de 10 milliards d'euros avec une diminution de, de 161 millions d'euros en autorisations d'engagement et 154 millions d'euros en crédits de paiement ces baisses ont lieu malgré une revalorisation de 4 % du point d'indice, le point de pension militaire des validité au 1er janvier 2023 c'est la diminution des crédits de la mission peut se justifier par le cycle naturel de la démographie en ces temps de crise, il aurait été souhaitable que les marges de manoeuvre ainsi libérés, bénéficient à des mesures de revalorisation des pensions, notamment au regard de l'inflation, de fait, année après année les crédits consentis aux anciens combattants ne cesse de s'amoindrir certaines avancées sont toutefois a salué, dans le cadre de la discussion budgétaire comme la décision du gouvernement de répercuter dès le 1er janvier 2023 la revalorisation du point d'indice de la fonction publique sur celle du point de PMI afin d'atténuer partiellement les effets de l'inflation pour les anciens combattants, autre point positif, la pérennisation des maisons d'Athos pour renforcer l'accompagnement des militaires blessés psychologiquement et des familles, en complément des autres programmes de réhabilitation psychosociale

de plus de 74 ans, quelle que soit l'âge du décès de la l'ancien combattant et la grâce à notre collègue rapporteur Jocelyne Guidez, hé bien unanimement l'ensemble du Sénat a reconnu qu'il était nécessaire de le faire en effet nous ça a voulu en l'article 41 qui propose de le de lever le critère temporel existant dans le droit à pension des des victimes de terrorisme par cet par cet article, ce droit n'est plus lié à la date de l'acte de terrorisme dont les personnes ont été victimes, par ailleurs, je tiens à cette occasion, une fois de plus, de saluer le caporal Loïc Liber, seul survivant du terrorisme dur terroriste mais Mohamed Merah aujourd'hui tu t'appeler Pejic et encore aux invalides, en dépit de ces avancées, le monde combattant en raison de la crise sociale et financière

l'évolution de l'appellation retraite du combattant en allocation de reconnaissance du combattant et également scruter la valeur du point PMI reste cependant nettement insuffisant au regard au regard au regard des préconisations de la commission tripartite pour le rattrapage du retard accumulé et pour compenser le niveau d'inflation 2022, par ailleurs, notre groupe souhaite également avoir l'assurance que la dite commission sera à nouveau appelés à se réunir pour le trimestre, la 1er ce qui Metz 2023 pour étudier cette question, enfin le nombre de points de retraite combattants qui est depuis 2017 de 52 d'ailleurs, je tiens à rappeler que le passage de 48 à 50 puis 52, étaient des mesures fortes des gouvernements de François Hollande, il serait donc souhaitable que le cette mandature, le nombre de points, il sera portée à 60 à raison de 2 points par an dès 2024 je souhaite par ailleurs conclure mon propos en insistant sur d'autres revendications plus qu'ancienne qui aurait toutes les raisons d'être satisfaite car elle concerne la mise en lumière et le devoir de mémoire et mon collègue gaga tous vient de faire partie de, en quelque sorte, c'est le devoir de mémoire que nous devons envers les combattants originaires des outre-mer et des régions vraiment d'outre-mer, dont le nombre, je le nombre de jeunes s'engagent encore dans nos armées parce qu'il faut saluer tous ces combattants qui sont venus en tant que dissident et grâce à eux, à ne pas si ils ont été mis en lumière, Jeanne, qui est une cinéaste qui vient d'avoir, d'ailleurs un Oscar, aux États-Unis, alors que pour le moment, la France ne connaît pas cette histoire, les dissidents, je veux également mettre en lumière le travail avec eux à pas assis, mais d'une autre martiniquaise Arlette, qui a également fait un film sur la situation de l'Indochine, tous ceux qui ont contribué à la guerre de l'ombre à à la guerre d'Indochine, hé bien ils sont méconnus et ils ont beaucoup souffert, parce qu'il y a ce film de Arlette pas quitte et je vraiment Madame la Ministre, que vous contribuez à ce que cette histoire, la vraie histoire soit connue parce que ce sont des personnes qui ont répondu à l'appel du général De Gaulle avec la FFR pour libérer la France, en espérant que ces pistes de réflexion seront prochainement étudiée par le gouvernement, le groupe socialiste écologique et le comité émet un avis favorable pour la mission Anciens combattants, mémoire et Liens avec la nation dans les termes du projet de loi de finances pour 2023 je vous remercie. Patricia Mirallès, secrétaire d'État chargé des Anciens combattants et de la mémoire, vous avez la parole.

Madame la présidente, madame et messieurs les rapporteurs, mesdames et messieurs les sénateurs, c'est le 1er budget que j'ai l'honneur de porter de présenter au Parlement, je le fais avec émotion et fierté ce budget, celui du monde combattant de la mémoire du lien entre les armées et la nation, et celui de la reconnaissance de la transmission, reconnaissance de l'engagement au service de la France des Françaises et des Français et transmission des valeurs républicaines, de la culture de défense et des forces morales, représentant de la nation à l'écoute des anciens combattants qui sont très présentes dans vos territoires vous entretenez des relations étroites avec eux, je vous c'est comme moi, attaché aux enjeux de ce budget, c'est aussi pour entretenir et enrichir cette proximité que j'ai entamé et que je mène un dialogue nourri et fructueux avec leurs associations, il est inconcevable que mon action que je veux ambitieuse et déterminée ne les associent pas, j'ai reçu les associations nationales et depuis le 4 juillet je vais à leur rencontre à chacun de mes déplacements, l'objectif que je me suis fixé de préserver et d'améliorer les droits du monde combattant de consolider la reconnaissance de la nation à son égard et de nous assurer que les dispositifs existants sont pleinement déployer et perfectionner lorsque ça paraît nécessaire tout d'abord le budget que je vous présente aujourd'hui garantie et même augmente les droits du monde combattant, il est doté de 1,8 milliards d'euros au titre de la mission Anciens combattants mémoire il y a avec la nation, le gouvernement poursuit ainsi l'effort qui consiste à limiter l'évolution des crédits à due proportion de la diminution du nombre de bénéficiaires de la dette viagère tout en maintenant un niveau inchangé, les crédits de solidarité, c'est dans cet esprit que j'ai proposé à la première ministre d'accélérer la revalorisation de la valeur du point de pension militaire d'invalidité pour que soit intégrée dès le 1er janvier 2023 et non en 2024, l'effet de la revue de l'organisation des traitements des fonctionnaires décidée par le gouvernement le 1er juillet dernier comme je l'ai annoncé lors de mon audition devant le Groupe d'études le monde combattant et mémoire de de votre assemblée, la première ministre a arbitré en faveur de cette proposition, le Conseil d'État étudiera cette semaine le décret qui a une qui introduira cette modification dans le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre en ce qui concerne un sujet majeur pour le monde combattant la demi-part fiscale des conjoints survivants, j'ai travaillé étroitement avec le Ministre délégué chargé du Budget Gabriel Attal pour pour atteindre une mesure plus juste, plus solidaire et plus sociale qui marque notre profonde reconnaissance à l'égard du monde combattant, je tiens donc à saluer l'adoption de votre assemblée, le 18 novembre de l'amendement gouvernemental et de 3 autres amendements similaires dans celui de la présidente du Groupe d'études monde combattant et mémoire Jocelyne Guidez, cela va permettre d'accorder la demi-part fiscale supplémentaire à toutes les veuves, âgé de 74 ans, quelle que soit l'âge du décès de l'ancien combattant, dès 2023, il s'agit d'une demande récurrente des associations d'anciens combattants, ces dernières années, je pense que nous pouvons toutes et tous nous féliciter de cet acquis à l'égard de celles qui se qui se sont battus pour la nation, ce budget porte encore d'autres mesures nouvelles, qui traduisent mon ambition pour le monde combattant, la première d'entre elles concerne et les blessés psychiques les sans blessure apparente, comme on les désigne parfois l'expérimentation par l'armée de terre, des maisons Athos et pérenniser, elles seront désormais financés par ce programme, il en existe 3 aujourd'hui dans deux vont être réinstallés dans des locaux plus adaptés, la construction d'une 4ème sera en outre lancé cette année, autre mesure nouvelle, nous allons étendre la la période de prise en compte de la qualité de victime d'acte de terrorisme, les victimes d'attentats survenus avant 1982 et bénéficieront en bénéficieront désormais les dizaines de blessés de l'attentat de la synagogue de la rue Copernic, en 1980 sont par exemple concernés une enveloppe d'un 1000000 d'euros, il est consacré, enfin, de 4 millions d'euros supplémentaires seront dédiés à l'entretien et à la rénovation du Patrimoine mémoriel. Et l'attention toute particulière sera accordée aux harkis et à leurs familles, vous savez, mon attachement à ce sujet, il est de notre devoir, que la nation connaissent pleinement les anciens combattants qu'ils furent, et qu'il reçoive réparation des préjudices qu'ils ont subi ce quinquennat et l'occasion de poursuivre les avancées significatives qui ont été amorcées à ce sujet à la fin du mandat précédent la dotation pour le financement du droit à réparation prévue par la loi du 23 février 2022 sera augmenté de plus de 30 % et portée à 60 millions d'euros, contre 46 millions d'euros en 2022 j'ai en outre demandé à ce qu'on renforce les moyens humains et matériels pour l'instruction des dossiers concernant les harkis, notamment pour permettre de solder en 2023 les dossiers déposés au titre du Fonds de solidarité et dans l'Ain, l'instruction est complexe, l'ONAC mobilisera dès le mois de janvier 2023 6 agents supplémentaires pour cette mission, aucune de ces démarches ne pourrait être concrétisée sans concéder les opérateurs du ministre du ministère des Armées chargé du monde combattant dans leur action et dans leurs moyens, qui sont donc reconduit en ce qui concerne l'ONAC léger, le contrat d'objectifs et de performance est en application. Le sujet du maillage départemental a beaucoup inquiété le monde combattant, souvenons-nous que pendant la la, l'épidémie de la Covid, les services départementaux de l'Office en même lien constant et précieux avec l'ensemble de leurs ressortissants, certains particulièrement fragiles et isolées, je veux ici à cette tribune les remercier, à l'heure où le gouvernement entend renforcer l'accès aux services publics de proximité, ce maillage ne saurait être remis en cause, le sujet est donc clos le budget que je vous présente prévoit une augmentation de la subvention de fonctionnement de l'ONAC deux 3 8 millions d'euros pour atteindre 60,2 millions d'euros. Ouais. Et nous maintenons son budget d'action sociale à un niveau élevé de 25 millions d'euros, gage de la capacité de l'Office a accompagné ses ressortissants les plus fragiles, qu'ils soient anciens combattants ou orphelins de guerre, de son côté, la subvention de fonctionnement de l'Institut National des invalides est accru de 700 millions d'euros pour Athènes 13 7 millions d'euros, la subvention de l'Ordre national de la libération est en légère hausse à 1,74 millions d'euros pour intégrer le coût de la revalorisation du point d'indice de la fonction publique en 2023, le ministère des Armées reste en pointe du travail de mémoire et de valorisation culturelle nous confirmons en 2023 notre politique de hausse du budget consacré à la mémoire qui atteignent donc presque 21 millions d'euros, le Patrimoine mémoriel, placé sous la responsabilité du ministère des Armées est extrêmement riche et porte la mémoire de notre nation, il fera l'objet d'vue une attention renforcée à hauteur de 10 37 millions d'euros en 2023, soit une augmentation de crédit de 28 % par rapport à 2022, un budget d'un 1000000 et demi d'euros sera par ailleurs consacré en 2023 aux commémorations concernant les 12 journées nationales et les célébrations liées aux thématique mémorielle largement consacré l'année prochaine au 80ème anniversaire de plusieurs grandes épisodes de la seconde guerre mondiale, je souhaite également que cette année 2023 mettent davantage en valeur les combattants en opérations extérieures, cette 4ème génération du feu, j'ai la volonté de travailler avec l'ensemble des acteurs pour mieux faire vivre et pour mieux faire connaître le le monument aux opérations extérieures installés dans le parc André Citroën à Paris la politique culturelle du ministère des Armées est ambitieuse et volontariste et prendre de nos modes de nombreuses formes en effet. Ce ministère et le 2ème, acteur culturel de l'État en touchant tous les domaines de ce secteur qui va du Patrimoine immobilier à la bande dessinée une directive culturel triennal guide pour la période 2021 2023 la mise en oeuvre de cette politique, elle a d'abord pour objectif de conserver de valoriser l'important Patrimoine culturel du ministère des Armées bâtiments historiques musées archives et bibliothèques et d'intensifier la recherche historique en soutenant notamment les jeunes chercheurs, par le biais d'allocation de thèse ou des contrats doctorant ces différents leviers renforce le lien entre les armées et la nation, ils soutiennent l'évocation et l'engagement des militaires et favorisent le recrutement en cela la politique culturelle du ministère des Armées développe les forces morales de notre pays, en s'adressant, nos concitoyens et appuie activement la politique de défense. Mesdames et messieurs les sénateurs, je suis au travail ce budget ouvre un mandat qui perpétuera au niveau de l'ambition au service du monde combattant de la mémoire et du lien armée nation jeunesse ce budget est donc celui de la résilience de la nation, enjeu fondamental de cette année qui a vu réapparaître un conflit de haute intensité sur notre continent, l'augmentation des moyens et les choix stratégiques, je vous présente, avec ce budget, sans les outils nécessaires pour impulser un élan nouveau à la politique de soutien au monde combattant et de transmission de la mémoire, que j'entends mener à l'avenir dans un dialogue permanent avec les associations, avec les territoires, et avec les élus, sachez compter sur moi. Oui merci madame la présidente, madame, madame la ministre, salut, monsieur le président de la commission défoncé, Affaires étrangères. Cher collègue rapporteur et mes chers collègues, alors cet amendement au nom de la commission des finances qu'on si sont l'indemnisation de 22 supplétifs de statut civil, c'est un sujet un sujet relativement ancien qui mérite aussi respect, reconnaissance et réparation donc 22 supplétifs de statut civil de droit commun de la guerre d'Algérie, qui se sont vu refuser l'allocation de reconnaissance sur le fond de monde une disposition législative déclaré depuis anticonstitutionnelle et donc il s'agit d'un mouvement de crédit concernant cet amendement, mouvement de crédit qui conduirait à confier à l'ONAC VG, qui a déjà pris contact avec ces personnes, titre de sa mission d'opérateur le programme 169 auteur de 92920 euros pour indemniser ces 22 personnes soit 4195 rapatriés et cette demande d'indemnisation est porté par les associations des rapatriés en faveur de ces personnes, dont 3 sont malheureusement déjà décédé, donc voilà, donc, et l'avis de la commission est favorable bien entendu. Quel est l'Asie du gouvernement Monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les sénateurs, l'amendement que vous proposez, vise à traiter la situation des anciens membres des forces supplétives de statut civil de droit commun, vous savez que les gouvernements successifs ont voulu réserver l'allocation de reconnaissance aux anciens supplétifs de droit local dans les conditions de rapatriement furent extrêmement dur au cours de ces dernières années, ces conditions d'éligibilité ont été consolidées juridiquement et validé par le Conseil constitutionnel, en 2013 concernant le cas des supplétifs de droit commun que vous évoquez dans votre amendement toutes les demandes ont été identifiés, toutes les situations, le nécessitant ont d'ores et déjà été traitées via l'action sociale de l'ONAC VG, je rappelle que ma prédécesseur Geneviève Darrieussecq, alors ministre déléguée en charge des anciens combattants, avait demandé aux services départementaux de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre de contacter chaque personne qui lui a été signalé, afin de pouvoir les intégrer dans les dispositifs d'aide de l'ONAC VG les 26 anciens supplétifs de statut civil de droit commun, signalé à l'époque en donc bien été contacté trois étaient décédées, si ce n'avait pas souhaité donner suite aux sollicitations, cette personne n'avait pas exprimé de besoins particuliers dans un ayant déménagé ne répondent non plus si ce n'était pas des anciens combattants déjà accompagné par l'action sociale de l'ONAC. Qu'il poursuivra ce soutien actif et IV avait reçu une aide pour un montant global de 9800 euros, une seule, une nouvelle demande est apparu en 2020 finalement retirée par l'intéressé et aucune demande en 2021, dans ces conditions, l'objectif que vous appeliez de vos voeux et déjà satisfait donc je vous donnerai ou un ou un avis défavorable ou un retrait de votre amendement merci.

Madame la Ministre. vous savez que j'avais porté la loi l'année dernière, celle du 23 février et si l'objectif poursuivi n'avait pas été satisfait, croyez-moi que je me serais engagé pour qu'ils le soient, je tiens d'ailleurs, mon cabinet à votre disposition afin que vous puissiez faire un point directement avec eux, si ça peut vous rassurer, merci. dans votre présentation, madame la ministre, on dirait qu'effectivement, enfin on traite ça comme autant de cas individuels avec différentes situations, nous, nous avons reçu quand même une sollicitation d'une association, c'est-à-dire que d'une personnalité morale qui défend ces ces 22 personnes, je ne sais pas si elles sont pas enfin il faudrait peut-être que veut on pourra vous donner leurs coordonnées que vous l'écriviez que leur demande leurs revendications sont satisfaites, mais en tout état de cause, je voulais pointer le fait que ce ne sont pas 22 situation individuelle mais aussi qu'elles sont portées par des associations d'anciens combattants. Oui, dans le droit fil de ce qui a été dit par ma collègue Madame pour Simon mais aussi par monsieur la Mini, Madame la Ministre, peut-être que vous avez quelques cas, mais pour avoir rencontré des associations et, lors de nos différentes auditions, hé bien ce n'est pas le même langage, donc il faudrait peut-être répondre puisse pour qu'elle puisse répercuter sur leurs différents mandats, mais pour le moment, je prends préfère que nous puissions voter et les amendements qui ont été proposées, merci Oui, cher Marc, tu connais ma position là, là-dessus, c'est vrai que moi ça fait plusieurs années que que je défends, ça, ça fait plusieurs années qu'on reçoit de la même association de monsieur Hamouri d'équipe harponner quelqu'un, on y a droit donc moi j'aime à se tenir là-dessus parce que, par contre, où je te rejoins victoire c'est que faudrait écrire quand même à ces associations et et leur expliquer et je pense qu'il y a vraiment un problème de communication,

je, je pense vraiment pas, je veux dire, on a vraiment travaillé en bonne Intelligence, à chaque fois avec avec madame la la Ministre, donc moi je je m'abstenir, quoi, je veux dire, on aura encore le même amendement l'année prochaine avec d'autres personnes qui vont le déposer parce que à chaque fois, il les gens, mais par contre, c'est peut-être un problème vraiment de communication là-dessus,

fait vous le demande, pourquoi pas, mais moi c'est qu'une seule association et c'est toujours la même personne d'accord et puis simplement une chose, c'est que nous avons le nom des gens, nous avons les noms des des personnes qui ont été indemnisées celles qui n'ont rien demandé et celles qui ne pouvait pas l'avoir. Parce qu'il y a quand même je crois trois 3 ou 4 personnes qui ne voulaient pas la voir alors soit que alors moi je peux pas vous donner les noms parce que c'est vrai que ça reste confidentiel, quand même, il faut, il faut le comprendre mais je, je pense que si vous vous me faites confiance, moi je peux en tout cas vous fournir les noms de ces personnes-là parce que le dossier entier je ai voilà

Alors je vous rappelle qu'il n'y a pas d'explication de vote sur les crédits d'émission, vous ne pouvez vous exprimer que sur les amendements, donc, Monsieur le Président, quand bon est-ce que vous voulez vous exprimer sur ce ah, à l'occasion de cet amendement. Je fais ce que je peux pour vous. la ministre des Anciens combattants, avec laquelle j'ai eu l'occasion d'aller à Verdun et surtout ces lieux de mémoire et et et saluer votre engagement personnel sur ces sujets, je voulais juste dire que quand on parle, anciens combattants et nous les les élus, ancien maire, on a souvent l'habitude et l'impression de parler pour ceux des grandes guerres, je ne voudrais pas qu'on oublie les anciens combattants qui résultent des OPEX, car nous sommes saisis de beaucoup de demande d'intervention de militaires qui se demande et s'ils vont pouvoir bénéficier de ce statut d'anciens combattants, nous avons laissé des morts, beaucoup de blessés et je voulais simplement profiter de la discussion de ce budget pour attirer l'attention sur ses soldats qui dans sur plusieurs continents, continue à nous représenter à défendre les libertés et nos valeurs et leur dire qu'il ne faudra pas les oublier, maintenant et dans l'avenir et le budget que nous allons voter aujourd'hui est aussi le garant des conditions de reconnaissance qu'on leur réserve pour plus tard, je vous remercie. Rapidement, peut être rassuré le président Cambon effectivement ont le droit à être reconnu ancien combattants toute tout soldat qui aura fait 120 jours au combat, et donc on parle, on parle bien des de nos soldats qui partent en opérations extérieures au combat et à ce moment-là, ils ont le droit effectivement à avoir la carte du combattant et il est tous les avantages qu'ils peuvent avoir en tant qu'ancien combattant quant à à l'amendement, je le redis, hein, puisque j'ai été moi-même député, donc j'ai connu cet amendement pendant 5 ans précédemment et c'est toujours Monsieur Maurice qui le dépose et je vous le redis je mets à disposition mon cabinet pour que vous ayez l'explication parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas donner directement ici, mais je, je, je vais mon cabinet à disposition pour vous donner la réalité et les personnes qui, il y a, il y a quatre personnes qui n'avaient pas le droit, parce que elle ne sont pas reconnus anciens combattant. Bien, je vous remercie, je vais donc mettre aux voix ces deux amendements identiques qui ont reçu un avis défavorable du gouvernement qui est pour.

Qui est contre qui s'abstient sont adoptés, j'appelle en discussion : les articles 41 et 41 bis, je me vois l'article 41 qui pour. Qui est contre qui s'abstient, il est adopté l'article 41 bis, un amendement du rapporteur de la commission des finances, vous avez la parole monsieur la. Oui merci madame la présidente, madame la ministre, chers collègues, alors concernant cet amendement, il s'agit. Pour l'article 41 bis prévoit la remise par le gouvernement au Parlement d'un rapport dans les conditions dans lesquelles l'État travers son opérateur l'ONAC VG assure le dénombrement, le soutien des pupilles de la nation des orphelins de guerre, cette information est déjà rendu public par l'Office via son rapport annuel, il serait toujours loisible aux parlementaires de demander tout complément d'information par le biais des questionnaires aussi le présent mon amendement propose la suppression de cette demande de rapport et vise à la suppression de du présent article et article et je sais qu'après il y a un autre amendement alors comme on dit, ne la commission des finances, nous on n'est pas complètement fermé, je crois qu'il a un esprit d'ouverture

un amendement de suppression de l'article, bon après il y a l'amendement suivons qu'il sera présenté par par nos collègues sur lequel ben je dirais je ne on va je demanderai l'avis de Madame la Ministre. Madame la Ministre, quel est votre avis sur cet amendement. dans lesquelles l'État via l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, assure le dénombrement et le soutien des pupilles de la nation et des orphelins de guerre, comme vous le savez l'article que vous souhaitez supprimer résulte d'un amendement parlementaire que le gouvernement a accepté d'inclure dans le dans le texte, voté en première lecture à l'Assemblée nationale, en vertu de l'article 49. Alinéa 3 de la Constitution, le rapport annuel de l'Office auquel vous faites référence dans votre amendement ne distingue pas les orphelins de guerre au sein de la population plus large que les pupilles de la nation dans les bilans globaux des interventions. Le rapport que le gouvernement a accepté de mettre au Parlement apportera donc une information complémentaire éclairant les parlementaires sur un sujet qui fait depuis plusieurs années l'objet de demandes récurrentes, cela me perds me paraît un objectif auquel nous pouvons tous souscrire de plus, je suis l'objet d'un grand nombre de sollicitations, soit par voie de courrier soit par voie de questions écrites soit par voie d'amendement sur les conditions d'accompagnement par l'état des pupilles de la nation et des orphelins de guerre, il me paraît donc nécessaire de mesurer l'efficacité du dispositif à travers ce rapport demandé à l'Assemblée nationale, en conséquence, je vous propose de retirer votre amendement ou alors ça sera un avis défavorable. Donc, monsieur le rapporteur, la. Oui merci madame la présidente, la Ministre va écouter, je dirais, puisque, en plus, dans la continuité de l'amendement suivant, je dirais, on reste bien entendu ouvert là à l'heure à la discussion tout à fait, tout à fait, je crois que tous les sujets sont importants, je crois que et franchement collectivement les on les on les respecte toutes et tous ces gens profitent sincèrement pour remercier tous les

je, on le en l'occurrence dans sous couvert de du rapporteur général de la commission des finances, des présidents de commission, je dirais, qui font l'honneur aussi de d'être là Monsieur Cambon et puis une autre collègue, présidente de la commission

ça, simplement je, je pense que c'est une bonne chose que tu l'aies enlevé mais par contre, Madame la Ministre, il faut qu'on ait ce rapport non, parce que voilà le le souci aujourd'hui, c'est que si on enlève les rapports ici, c'est parce que généralement on n'en a pas, voilà, on a on a pas le retour, donc moi je suis pour, pour ça, parce que vous avez raison, on a plein de de questionnement par rapport à ça et notamment moi j'ai été interpellé sur le pupitre de France, c'est-à-dire si on est ancien combattant, en effet, les enfants sont plus de de de France, il décède et par contre quelqu'un qui a fait de la résistance et qui est décédé ou qui a été tué lors d'une intervention ces enfants là ne sont pas considérés comme publics de France, donc il y a vraiment un réel travail à faire là-dessus, mais faut-il que le rapport vraiment nous reviennent voilà merci beaucoup.

dont je connais l'intérêt approfondie pour ces questions mémorielles et et précisément ce n'est pas un rapport par rapport c'est un rapport pour préciser dénombré, on est dans une situation hein les, les, les, les survivants de la seconde guerre mondiale sont en train de disparaître, il y a des nouveaux anciens combattants, il y a des nouvelles pupilles de la nation et donc un état et une mesure permanente est importante et c'est le sens précisément

et les orphelins de guerre, qui concerne les malgré-nous c'est pas Pascal Ory le le grand historien spécialiste de la période qui dit l'occupation allemande de l'Alsace et de la Moselle de 39 à 45 a été si violente qu'elle a paradoxalement fait plus pour l'intégration de cette région au sein de la plaine, culture et intégrité nationale française que des décennies et des siècles de tentative dans ce sens et là précisément nous avons vis-à-vis de ces personnes qui ont été enrôlés de force, de 1939 à 1945 surtout à partir de 42 plus de 113000 alsaciens et 31000 mosellan, il est absolument indispensable à la suite de la reconnaissance, qui avait engagé par le général De Gaulle en 1963 de ces malgré-nous de ces gens forcés de combattre contre la France et dans les l'armée allemande, voire nazis, il est important qu'on ait cette pleine reconnaissance de leurs droits, le plein dénombrement et c'est le sens de cet ajout qui rendra encore ce rapport, on compte plus merci donc je vous appelle, hein, merci l'approuver, merci. Quel est l'avis de la commission sur cet amendement. Oui merci madame la présidente, la mamie ce cher collègue écoutez on peut évoluer, je dirais, positivement, ce sera un un avis favorable et puis j'en profite pour remercier je dirais tous les collègues qui sont présents, vos services, madame la ministre, et puis l'ensemble des services du Sénat, tous services confondus pour l'engagement et le dévouement merci. L'avis du gouvernement. Monsieur le sénateur Gattolin mesdames et messieurs les sénateurs, donc je vais donner évidemment un avis favorable puisque, il me semble que dans ce rapport,

incorporés de force donc par l'armée allemande des orphelins qui ont été des incorporés de force peuvent se voir attribuer la qualité des pupilles de la nation, si leurs parents a reçu la mention Mort pour la France, leur sort spécifique justifie en outre qu'une attention distinctes soit porté à leur situation, il paraît donc pleinement justifié de leur consacrer un chapitre dans un rapport consacré aux conditions dans les, dans lesquelles l'État au travers de l'Office de de nationale des combattants et des victimes de guerre, assure le dénombrement et le soutien des pupilles de la nation et des orphelins de guerre, donc je je je donnerai un avis favorable à cet amendement. qui est contre qui s'abstient, il est adopté et l'ordre du jour appelle maintenant l'examen des crédits de la mission culture. Merci madame la ministre, vous voulez vous exprimer avant qu'on je vous en prie. Juste rapidement je voulais remercier donc madame la présidente, je voulais vous remercier, je voulais remercier tous les sénateurs d'avoir d'avoir voté ce budget qui est si important pour nos anciens et pour le sacrifice et qu'ils qu'ils ont, pour la nation, merci beaucoup. La parole est à monsieur Eblé, rapporteur spécial de la commission des finances.

Madame la présidente, madame la Ministre. Mes chers collègues. Le montant global des crédits demandés dans le cadre du présent projet de loi de finances pour la mission culture s'élève à plus de 3 milliards 700 soit une progression dépassant 7 % celle-ci est supérieure à l'hypothèse d'inflation retenues, il y a quelques semaines pour 2023 en projet de loi de programmation des finances publiques la quelle hypothèse devrait cependant rapidement être remise en cause, si l'on observe le niveau déjà constatés et les perspectives d'inflation dans un proche avenir j'aborderai dans un 1er temps le programme 131 dédié à la création sa dotation est majoré de 10 % pour dépasser le milliard d'euros, cette progression des crédits peut être en première analyse, salué, dans un contexte de reprise délicate de l'activité, et singulièrement de l'activité culturelle elle ne lève cependant pas toutes les inquiétudes pour l'ensemble du secteur confronté à un effet de ciseau entre redémarrage progressif mais l'de l'activité et hausse du coût des dépenses contraintes notamment bien sûr énergétique pour les opérateurs de l'État ces surcoûts ne seront pas intégralement compensée en loi de finances, ce qui devrait induire une réduction des marges artistiques 30 pour 100 en 2023 la fermeture de certains opérateurs à la rentrée 2023 est une hypothèse malheureusement crédible, faute de pouvoir produire certains spectacles, la perspective des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 constituent également une source supplémentaire d'anxiété avec la probabilité renforcée d'annulations de festivals et de concerts en raison d'un manque de forces de l'ordre et de sociétés privées pour en assurer la sécurité, je relève en outre que l'action du ministère dans le domaine de la création peut apparaître brouillées, la multiplication des objectifs assignés 16 sous-actions pour les actions, hein, le recours soutenu à la labellisation fragilise en effet sa lisibilité, j'observe par ailleurs le caractère résiduel pour ne pas dire marginal qu'elle peut revêtir dans les territoires où elle se résume à un financement complémentaire des politiques territoriales pour conclure sur ce programme, je m'attarderai sur 2 mesures : la première vise la poursuite du programme de commande publique monde nouveau mise en place dans le cadre du plan de relance 10 millions d'euros seront dédiés à ce dispositif qui vise notamment à faire entrer la culture dans des zones où elle n'est plus assez présente espaces ruraux périphéries urbaines ou Coeur de ville dégradés, il conviendra cependant d'être vigilant sur la réalité de l'accompagnement des artistes, la complémentarité avec le un pour 100 culture et le droit de suite que le ministère doit avoir sur les Oeuvres ainsi financer s'agissant notamment des arts visuels. mise mesure les 12,7 millions d'euros qui viennent abonder le soutien à l'emploi, dont 7 millions d'euros fléché vers le Front national pour l'emploi pérenne dans le spectacle, son peps cette progression des crédits s'inscrit dans une trajectoire haussière révélatrice d'une sous-budgétisation constante depuis 2019 dans ces conditions, nous nous interrogeons sur la fiabilité de la prévision budgétaire pour 2023. Venons-en désormais au programme 175 dédié au Patrimoine, au pluriel, et qui devrait être doté de 1,1 milliard d'euros en 2023 soit une production là une progression là encore de plus de 7 % par rapport à 2022 ce financement est complétée par des soutiens hors budget, mobilisant nos concitoyens dont pour Notre-Dame de Paris, dont le montant 849 millions d'euros devrait dépasser le coût des travaux actuellement estimé à 703 millions d'euros et le tour du Patrimoine, pour lequel le ministère des gels, la réserve de précaution chaque année ce jeu comme l'augmentation prévue des crédits du fonds incitatifs partenarial vient d'ailleurs compenser la tendance à la baisse des crédits déconcentrés, près de la moitié de la progression des crédits dédiés au programme 175 relève de mesures destinées à tenir compte de l'inflation et de la hausse des coûts sur les 37 4 millions d'euros dédié à cet objectif, près des 2 tiers sont fléchés vers les opérateurs, la majoration des coûts et déjà constaté sur plusieurs chantiers, encadré par l'État s'agissant précisément des chantiers, nous avons noté que 2023 devrait être marquée par l'ouverture de la Cité de la francophonie à Villers-Cotterêts, le coût du chantier était initialement évalué à 185 millions d'euros avant d'être porté à 209 millions d'euros, sa réalisation n'a d'ailleurs été permise que par la mise en oeuvre du plan de relance cette expérience coûteuse doit servir de point cardinal dans la réflexion à mener sur d'autres grandes opérations d'investissement et je pense en particulier à l'aménagement du site de Clairvaux Clairvaux qui se voit doté de 15 millions d'euros en autorisations d'engagement pour 2023 démarrage assez modeste, chacun en conviendra, en regard du coût global de cette opération, au-delà de la hausse des dépenses contraintes nous relevons une hausse importante des prix d'acquisition d'Oeuvres les plus importantes qui aurait vocation à enrichir nos collections publiques, les niveaux d'adjudication dans les ventes aux enchères s'établissent désormais très régulièrement à un niveau 4 à 10 fois supérieurs, voire davantage à celui des estimations. Enfin, si la reprise de la fréquentation des établissements publics dédiés au Patrimoine a été plus importante que prévu en 2022 l'horizon ne semble pas pour autant totalement dégagée en raison de plusieurs incertitudes, l'effet de l'inflation bien sûr sur les dépenses culturelles, l'absence de retour de certaines clientèles, on pense en particulier à la clientèle des touristes chinois et la perspective d'une fermeture, le temps des Jeux olympiques et paralympiques en 2024 je sais maintenant la parole à mon collègue Didier Rambaud pour les programmes de 124 et 361. Comme le rapporteur, la commission des finances vient de le dire, c'est donc. Ouais, sénateur Rambo de prendre la la suite. Madame la présidente, madame la ministre, messieurs les présidents de commission mesdames les rapporteurs pour avis, mes chers collègues, ce projet de loi de finances pour 2023 prévoit une majoration de la dotation du programme dédié à la transmission des savoirs et à la démocratisation de la culture de près de 6,5 % en crédits de paiement par rapport à 2022 les crédits devrait ainsi atteindre environ 800 millions d'euros, les moyens financiers dédiés aux établissements d'enseignement supérieur culturel et à l'insertion professionnelle devrait progresser de 32 millions en CP afin de répondre à 4 objectifs évaluation des bourses sur critères sociaux, le renforcement des subventions de fonctionnement et des et d'investissement des écoles d'art et d'architecture, la mise en oeuvre des grands projets d'investissement de ces mêmes écoles et enfin le soutien aux établissements territoriaux d'enseignement supérieur, en ciblant notamment le statut des enseignants au sein de ces écoles

d'art dramatique de Paris et autres au Théâtre national de de Strasbourg qui organise rencontres et auditions prend en charge une partie des jeunes artistes engagés à la suite des auditions, programme des maquettes du 1er spectacle et élabore un annuaire des artistes issus des 11 écoles nationales d'art dramatique, par ailleurs, 13 millions d'euros sont fléchés vers des établissements structurant au sein des écoles de la création et du Patrimoine, cet apport doit être salué ce qui ne doit pas nous empêcher de rappeler l'importance des restes à payer sur des chantiers, couverts par le programme 361 venons en maintenant un dispositif auquel je suis attaché le passe culture déployés dans toute la France depuis mai 2021 étendu en 2022 au jeune de 15 ans et plus, et aux élèves, à partir de la quatrième le passe culture sera ouvert aux jeunes 6ème et 5ème en 2023 208,5 millions d'euros sont prévus en 2023 pour le financement du dispositif qui est, rappelons-le, aujourd'hui, le 2ème, opérateur du ministère de la culture, derrière la Bibliothèque nationale de France, plus de 2 1 1000000 de jeunes sont aujourd'hui inscrits sur l'application et 14 millions de réservations de produits culturels ont été opérés via le passe pour un montant total de 235 millions d'euros concrètement 87 % des jeunes concernés ont acquis un bien culturel par cette intermédiaire, le Pass culture est un dispositif qui, à mes yeux et pertinent et je continuerai de soutenir mais comme vous le savez, madame la ministre, je reste attentif à sa mise en oeuvre pour que l'efficacité puisse être amélioré le Pass ne peut se résumer à une simple plateforme d'achats de biens et de services et doit être éditorialistes en vue de mettre en place un véritable parcours culturel lors des prochains des prochains mois, avec mon collègue Vincent emblée nous allons vérifier que le Pass ne serve pas au financement d'achat lié au au parcours scolaire et qui puissent contribuer à faire évoluer des pratiques culturelles l'accent pourrait être ainsi mis sur l'accès aux spectacles vivants, par exemple, j'en profite également pour pour tordre le cou à quelques rumeurs, j'ai entendu récemment sur le fait que le Pass culture ce rééligible dans le au parc de loisirs, non ce n'est pas le cas pour en revenir aux puces aux pistes d'amélioration du Pass culture je crois également que nous devons renforcer l'accès des jeunes non ce qui l'a scolarisé au Pass, seuls 3,7 % des inscrits sur l'application ont déclaré ne pas être scolarisés, or ce ratio est plus faible que le nombre de jeunes non scolarisés rapportée à l'ensemble de la population visée et, bien sûr, sans oublier les les zones rurales et périurbaines où l'offre culturelle et là ce n'est pas la même et où les questions de mobilité, j'ai eu l'occasion de vous le dire, se posent en tout état de cause, le passe culture de doit pas résumer aussi l'effort de l'État en faveur de l'éducation artistique et culturelle, autrement dit la montée en charge budgétaire de l'application ne doit pas s'effectuer au détriment des moyens qui lui sont traditionnellement dédiée, nous ne pouvons que déplorer le fait que les indicateurs rattaché au programme mettent d'ailleurs en avant une réduction de la part des enfants, il a et adolescents ayant bénéficié de bénéficier d'une action d'éducation artistique et culturelle et une baisse de l'effort en faveur des territoires prioritaires pour conclure je souhaite revenir sur le programme 224 soutien aux politiques du ministère qui devrait être doté d'environ 810 millions d'euros en 2023, comme lors de l'exercice précédent, la masse salariale devrait devrait croître en 2023, atteignant ainsi 516 millions d'euros, 67 % de cette progression résulte de mesures catégoriels dont le plan de rattrapage indemnitaire, celui-ci doit permettre de renforcer son attractivité et d'éviter des vacances de postes prolonger le projet immobilier Camus, lancée en 2019 prévoit la rénovation des locaux et l'aménagement de nouveau bureau au sein du ministère de la culture devrait ainsi en 2023, passer de 7 à 3 sites initialement établi à 36,6 millions d'euros, le budget prévisionnel a été actualisé en 2022 pour être porté à 55 43 millions d'euros, l'exercice 2023 devrait voir la dotation numérique du ministère, continuer à progresser 26 52 millions d'euros seront ainsi dédiés au renforcement de la transformation numérique et de la cybersécurité et à la mise en place d'outils permettant de renforcer et de fiabiliser le suivi économique de l'activité des secteurs qui le subventionne en ciblant notamment la fréquentation au sein des opérateurs ou là où la

pardon, compte tenu des moyens supplémentaires dédiés à la culture que je souhaite souligner une nouvelle fois la commission des finances, a décidé d'approuver les crédits de la mission culture. Merci. La parole est maintenant Madame Sabine Draxler, rapporteur pour avis de la commission de la culture, l'éducation et de la communication. Madame la présidente, madame la Ministre, le monde du Patrimoine appréhender le niveau des crédits en 2023 après les aides exceptionnelles dont il a bénéficié pendant la crise sanitaire, nous sommes satisfaits de constater que l'État maintient son effort dans ce secteur, nécessite des investissements qui s'accommode mal d'un financement par à-coups, le niveau de l'inflation reste néanmoins un motif d'inquiétude, tant pour les musées que pour la poursuite des chantiers de restauration car le budget 2023 ne compense que partiellement les les effets, à cet égard, la Commission de la culture, regrette que les crédits destinés à la restauration des monuments historiques ou à la rénovation des équipements patrimoniaux, les collectivités territoriales ne soient pas revalorisées, à l'exception du fonds incitatifs et partenariale, compte tenu de l'effet ciseaux auquel les collectivités sont confrontées, des problèmes d'ingénierie qu'elle rencontre, il aurait été utile que celle-ci soit davantage accompagner. Nous souhaitons vous interpeller madame la Ministre, sur la situation préoccupante des effectifs des services déconcentrés en charge du Patrimoine qui ne leur permet plus d'assumer correctement leurs missions de conseil et d'expertise auprès des collectivités territoriales et des propriétaires privés, il y a urgence à recruter et à revaloriser l'attractivité de ces postes, nous sommes également préoccupés par le faible niveau des crédits alloués à l'architecture et aux espaces patrimoniaux remarquables face aux enjeux de régénération des centres anciens et de transition écologique et énergétique, il ne faudrait pas que le Patrimoine se retrouve la victime collatérale de ces politiques, faute d'avoir pris en compte suffisamment tôt à quel point il constitue au contraire un levier de revitalisation comme de sobriété énergétique, nous sommes convaincus que la réhabilitation du bâti ancien constituent d'un point de vue durable, l'avenir de la construction, parmi vos priorités, Madame la Ministre, figure à juste titre la transition énergétique de votre ministère si nous saluons les efforts destinés à améliorer les performances des bâtiments, des opérateurs, nous pensons que votre accent doit aller plus loin dans la mesure où il est aujourd'hui avéré que la transition, telle qu'elle est amorcée va affecter la pérennité de tout le Patrimoine dont votre ministère et pourtant chargé d'assurer la préservation madame la Ministre, les dispositions de la loi climat et résilience vont entraîner ni plus ni moins que la disparition des caractéristiques architecturales française car ni les nouvelles modalités de calcul du DPE ni les solutions de rénovation thermique préconisées ne sont adaptées au bâti d'avant 1948 sans vouloir soustraire le Patrimoine aux impératifs de transition écologique, nous sollicitons votre intervention pour que les travaux de rénovation énergétique ne se traduise pas par la perte du Patrimoine et du savoir-faire de notre pays, ainsi que par un gaspillage d'argent public, il y a urgence à engager un travail interministériel pour mieux concilier préservation du bâti ancien et transition écologique, nous avons identifié dans notre rapport plusieurs leviers d'action et nous espérons vraiment Madame la Ministre, pouvoir compter sur votre engagement pour les mettre en oeuvre, très vite, car de nombreuses maisons partout en France, ont déjà fait les frais de ce malentendu réglementaire, je vous remercie. Madame Sylvie Robert, rapporteur pour avis si également de la commission culture, éducation, communication. Madame la présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, la nouvelle progression des crédits des programmes Création et transmission des savoirs et démocratisation de la culture constitue bien évidemment un réel soulagement nous vous remercions madame la ministre d'être parvenu à convainc l'ensemble du gouvernement que le secteur culturel devait rester une priorité pour 2023 et le secteur de la création encore besoin d'accompagnement si les collectivités publiques long aussi très largement soutenu pendant la crise sanitaire sa situation demeure fragile, il faut le dire qu'il est affecté depuis 7 ans par des crises successives, les attentats 2015 la pandémie de Covid 19 et désormais la hausse des prix de l'énergie, malheureusement, aucune de ces crises n'est encore véritablement surmonter la vague d'attentats s'est traduite par un relèvement durable est considérable des coûts de sécurité des établissements quant à la crise sanitaire, ses effets reste encore palpable, que ce soit sur la fréquentation ou sur les recrutements avec une vraie crise des vocations observables sur l'ensemble des différents emplois à cela s'ajoutent les changements profonds des comportements des publics qui mettent de plus en plus à mal les modèles traditionnels traditionnels économique des établissements, que ce soit d'ailleurs des établissements publics comme privés, dans ce contexte, on comprend que la crise énergétique et l'inflation généralisée cristallise les inquiétudes puisqu'elles affectent non seulement les dépenses des établissements mais aussi leurs recettes, les Français réduisent leurs dépenses de loisir, le mécénat est en baisse et les collectivités territoriales sont tentés de réduire leurs engagements financiers pour faire face à la hausse de leurs dépenses pour faire face à ces difficultés, nous vous savons gré d'avoir choisi de faire porter la priorité en 2023 sur l'emploi ainsi que sur le renforcement des marges artistiques des établissements leurs marges de manoeuvre sont effectivement réduites et la hausse de leurs tarifs ou la révision à la baisse de leur programmation aurait des effets désastreux tant sur la fréquentation que sur la création, il reste néanmoins désormais accompagner cet effort financier par un renforcement du dialogue entre votre ministère les acteurs culturels et les collectivités territoriales, il s'agit d'un besoin essentiel pour ce secteur qui nécessite de disposer de visibilité très en amont du fait des contraintes, on le sait, de leur programmation c'est vrai aussi pour les crédits d'impôt mais je pense que l'on en parlera, il est vrai par exemple que l'affaire autour des possibles annulations de festivals en 2024 du fait des jeux Olympiques aurait peut-être pu être évités si des concertations préalables était intervenus alors la commission de la culture est convaincu que le soutien à la création artistique, à l'éducation artistique et culturelle et aux établissements d'enseignement passe par Ray meilleur dialogue et par le développement de nouvelles modalités de contractualisation avec les collectivités territoriales, je vous remercie et je vous propose donc de donner un avis favorable à l'adoption de ces crédits,

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission Culture mesdames et messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, c'est une longue période chahutée que le monde de la culture traverse depuis 3 ans et si quelques éclaircies ont pu parcourir son ciel, les nuages s'amoncellent à nouveau, et avec eux leur cortège inquiétude en 2020 débuter la crise sanitaire les confinements les restrictions et la cruelle sanction de ne pas faire partie des essentiel depuis, on le sait, et parce qu'il a fallu qu'elle nous manque pour qu'on fasse cela soit compris, la culture est un bien vital, or la guerre aux portes de l'Europe, l'inflation, la crise climatique le retour prudent différents des publics nous ordonne d'anticiper, de crainte que nous quitte à nouveau dépenses entier de la vie culturelle, les Budgets examiné aujourd'hui sont pleinement concernés par ces crises et nous saluons ici, Madame la Ministre, de réels efforts budgétaires réalisées, c'est un marqueur de la reconnaissance du rôle majeur joué par la culture dans cette bien rude période néanmoins des inquiétudes demeurent pour aujourd'hui mais aussi pour demain, comme souligné par nos 2 rapporteurs Sylvie Robert et Sabine Draxler nous savons tous que cela nécessitera à coup sûr un suivi budgétaire attentif pour réagir à temps, via des projets de loi de de finances rectificative, que ce soit les programmes 175 patrimoines 361 transmission des savoirs et démocratisation ou 131 création de grands défis attendent votre ministère en 2023 d'abord l'inflation et le coût de l'énergie, l'hypothèse de plus qu'à 3 % et déjà caduque et la hausse des crédits 7 % pour le 133 7 pour le 175 et 10 pour le 131 devait devrait en être atténué d'autant le soutien aux opérateurs est en progression, mais le surcoût énergétique estimé Laurent déjà bien insuffisant pour les établissements d'enseignement supérieur d'art, les conservatoires, où les écoles d'architecture même constat en matière de Patrimoine, c'est en plus à une forte hausse du coût des matières premières des chantiers qu'il faut faire face la réalité rattrape vite les établissements structure et 5 s'imposent à leurs arbitrages budgétaires, mettant en péril la programmation artistique, les horaires et durée d'ouverture, le calendrier des créations les tarifs et les délais des chantiers des annulations sont envisagées des reports des fermetures à ces mesures extrêmes de voir devra répondre un soutien extrême ensuite la gestion des ressources humaines, sur le terrain, festival établissements culturels, constate un manque criant des métiers nécessaires à leur fonds de qu'ils soient techniques, administratifs ou artistiques, même constat pour l'enseignement, les écoles d'architecture, elles ont besoin de moyens supplémentaires, car il va falloir mettre en place des fourmis, des formations initiales et continues pour répondre au défi de la mise aux normes énergétiques dans les Drac, le manque d'attractivité pointé, il existe ainsi des postes vacants dans le secteur du Patrimoine sur 12 postes ouvertes en en sorti à l'école de Chaillot, ce que seuls 4 sont pourvus, le recours aux contractuels ne pallie pas les manques à cette crise de la ressource en matière de professionnels s'ajoutent celles liées au coût des revalorisations salariales liées à l'inflation, le ministère fait un réel effort pour compenser, quel que soit le secteur, mais tout l'écosystème culturel dans sa très grande diversité de statuts et de métier n'en bénéficiera pas les collectivités et les acteurs privés sont eux aussi concernés les arbitrages ne vont pas toujours vers la compensation et l'offre culturelle dans sa diversité en effet fragilisé, outre ces 2 sujets, Madame la Ministre, 3 autres nous air le 1er concerne l'éducation artistique et culturelle, et le rôle du Pass culture on s'étend, ou les choix budgétaires sont complexes, on ne peut que s'étonner de son montant représentant 25 % du programme 361 ceci dénote singulièrement avec la sobriété budgétaire qui s'impose aux acteurs de la culture, l'ASS Pass culture ne connaît pas la crise, ensuite si la peur collective et tu n'as à une avancée pour faciliter l'accès à des actions culturelles dans les établissements scolaires du second degré, elle interroge sur son usage et sa mise en oeuvre en matière de assez le passe à une logique d'offre à laquelle les établissements répondre on crée la demande, alors que le assez est avant tout un projet, une médiation vers la culture, c'est pourtant cette médiation entre enseignants, élèves, structure créateur et collectivités construite dans le temps qui fait la réussite de l'EAC, la labellisation proposé tend à exclure certaines actions ou artistes et à diminuer les interactions avec les collectivités, la simplification à l'extrême du process de commandes confine à une uberisation de l'EAC, nous ne souhaitons pas qu'elle se résume au Pass culture, la transformant en un système d'achat dans une boutique d'action d'artistes et d'événements le second point concerne les festivals, ils subissent une loi des séries, la crise sanitaire, la crise énergétique, les surcoûts de programmation la crise climatique et maintenant la menace d'annulation de décalage liés aux JO à tout cela s'ajoute le retour hésitant du public, le Fonds festival ne suffira pas, les organisateurs attendent enfin la nomination d'un référent au ministère et de référent dans les Drac, ils entendent être défendue lors de tous les arbitrages qu'ils sont faits et qui les concernent, si les plus grands et les plus solides parviennent non sans difficultés à tenir tous les autres sont en danger, or par leur nombre, leur diversité et leur présence dans tous les territoires, ils sont des moteurs de la vie culturelle, singulièrement sur la période estivale, les JO sont évidemment un rendez-vous exceptionnel et une phrase, une fierté pour notre pays, mais les festivals ne doivent pas en être la victime désignée à cause d'un manque de moyens logistiques ou de compétence phagocyté par ce grand événement, enfin le 3ème point concerne la situation du Patrimoine confrontée à l'arrivée de du diagnostic de performance énergétique le DPE si la transition écologique et l'amélioration énergétique du bâti sont des nécessités, cela ne doit ni nuire au Patrimoine ni détériorer la qualité de nos communes, en écho à l'intervention de notre rapporteur Sabine dressèrent je ne peux que vous alerter sur ce qui se passe en ce moment le DPE celui des règles inadaptées au bâti conçu avant 1949 il lui est même délétère or nul besoin d'être spécialiste pour comprendre que l'isolation par l'extérieur sur un bâti ancien en Pierre ou en torchis, par exemple, est une erreur technique, c'est aussi une faute vis-à-vis l'identité de nos villes et villages, effaçant les particularismes locaux nuisant à la qualité du cadre de vie,

pour conclure, Madame la Ministre, vous l'avez compris dans ces moments où tout confine à l'urgence ou il est nécessaire de faire des choix, dégager des priorités ou le temps du dialogue évite raccourcis voire inexistants, le ministère de la culture doit être fort voix entendu ces propositions retenues et ce quel que soit l'interlocuteur ministère COJO Adem, par exemple, trop nombreux sont les annonces ou décisions ou la culture et le Patrimoine sont concernés et pour autant, le sentiment est donné que le ministère et peu concertée, Madame la Ministre, le groupe UC votera favorablement ce budget, mais au delà de ce vote, parce que nous soutenons ardemment la culture et le Patrimoine et que l'essentiel est bien là, le groupe UC témoigne ainsi de sa vigilance et de ses inquiétudes, préservons la poésie de notre pays, le Patrimoine et les paysages en sont les craint la culture et l'air qu'on y respire Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Défendent le budget de la culture pourrait seulement consisté à relever ses externalités positives sur l'économie, en particulier en particulier touristiques et son rôle social, en réalité, l'État doit se comporter en promoteur sans attendent l'exacte contrepartie comptable de son investissement, notre pays a la responsabilité de soutenir la culture qui fait tout simplement partie de notre système de valeurs républicaines, elle nous oblige, elle est l'expression de la liberté selon une formule Cantiliens en cela, si j'ose dire la culture. Par essence essentielle elle a d'ailleurs trouvé sa place dans le plan de relance qui a permis à nos acteurs et institutions du monde culturel de traverser la crise liée à la pandémie de Covid je salue cet effort et sa pérennisation à travers le programme de commande publiques monde nouveau qui se poursuivra avec un 1er soutien de 10 millions d'euros en 2023 en direction du spectacle vivant et des arts visuels, j'en profite pour rappeler notre amendement de bonification du crédit d'impôt pour le spectacle vivant, adopté en première partie du projet de loi de finances et nous espérons qu'il survivra à la navette parlementaire, en attendant, mes chers collègues, la culture devra affronter d'autres difficultés, je pense bien entendu au coût de l'énergie, ainsi qu'à la baisse du pouvoir d'achat de nos concitoyens qui pourrait les comptes hein craindre à sacrifier les activités culturelles en outre la question des Jeux olympiques et par olympique de 2000, vingt-quatre est un sujet d'inquiétude, madame la Ministre le monde culturel attend des réponses car certains de ces acteurs ont besoin de se projeter dans le temps, pour des raisons évidentes de programmation pour faire face à tout cela, le projet de loi de finances pour 2023 affichent une progression globale d'environ 7 % des crédits de la mission culture c'est un effort significatif mais l'action publique doit respecter l'objectif d'équité, la culture, c'est pour tous et sur tous les territoires s'agissant tout d'abord nos territoires je souhaite évoquer la question du Patrimoine, un levier essentiel du dynamisme local et surtout un marqueur fort de l'identité de nos villes, départements ou régions les crédits du programme 175 augmenteront de 7 5 % en 2023, c'est une bonne chose mais ce programme ne reflète pas l'ensemble de l'effort de l'État en faveur du Patrimoine, j'ajouterai qu'il est fortement concentré sur les monuments historiques et les musées, par conséquent, il n'est pas inutile de souligner l'action très volontaire des collectivités locales, selon la Cour des comptes, elles investissent en moyenne chaque année 650 millions d'euros en direction du Patrimoine avec un regard appuyé sur le petit Patrimoine de proximité qui est aussi. Mais tous les moyens réunis, y compris ceux de la Fondation du Patrimoine et de la mission Bern dont le fameux lotos suffiront-ils à couvrir les défis auxquels est confronté notre Patrimoine : le renchérissement des chantiers de restauration et la nécessité d'accélérer la transition énergétique sont deux enjeux imminents et le 1er va clairement oblitérer une partie de la hausse des crédits budgétaires s'agissant de la transition énergétique, il convient d'éviter de mettre dos à dos, Patrimoine et développement durable dans les 2 cas, il s'agit de conserver notre héritage. Aujourd'hui, nous disposons des et des outils technologiques pour concilier les mesures de protection du Patrimoine et les objectifs de développement durable, il faudra bien sûr bien former les architectes pour cela les moyens déconcentrés de l'État, en charge du Patrimoine doivent être à la hauteur, or ils sont très contraint actuellement. Enfin, je souhaite souligner un 2ème point, celui de la démocratisation de la culture, l'égal accès à la culture est un objectif de la politique publique du ministère à travers le programme 361 dans ce cadre, le passe culture focalise beaucoup l'attention pour ne pas dire les crédits puisqu'il absorbe jusqu'à 25 pour 100 du programme. Moi je me réjouis de sa montée en charge et de son ouverture à de nouvelles classes d'âge, mais je m'interroge également sur le fait que le spectacle vivant et les musées recueille une bien moindre attention il y a donc un effort à faire pour inciter les jeunes à plus de diversité dans leurs pratiques culturelles, il faut, comme l'avait rappelé Malraux en 66, je cite, faire ce que la 3ème République avait réalisé dans sa volonté républicaine pour l'enseignement, il s'agit de faire en sorte que chaque enfant de France puisse avoir droit au tableau au théâtre, au cinéma, et caetera, comme il a le droit à l'alphabet dans cette perspective, il me semblerait souhaitable de ne pas négliger les autres volets du programme dont les actions plus traditionnelles d'éducation artistique et culturelle, mes chers collègues, je le répète parce qu'elle est au coeur de notre projet républicain : la culture doit toujours être soutenu le groupe RDSE approuvera donc les crédits de la mission. Merci madame Laure Darcos pour le groupe Les Républicains. Merci madame la présidente, madame la Ministre, mes chers collègues, avec le projet de loi de finances, vient le temps des promesses, celui de 2023 n'échappe pas à la règle, les moyens de la mission culture sont abondés à 205 de 250 millions d'euros, ce qui représente une augmentation de 7,4 % par rapport à la loi de finances initiale pour 2022, il s'agit évidemment d'un motif de cette. Six actions et nous aurions tort de considérer cet effort budgétaire comme négligeables mais est-il pour autant suffisant, je n'en suis pas certaine, tous ceux qui sont investis de cette mission essentielle de préserver la pâte de Patrimoine, de favoriser l'acte de création de promouvoir la culture pour tous, s'arme de l'augmentation exponentielle des coûts énergétiques, la filière du spectacle et le Patrimoine sont particulièrement impactées, certes l'État est intervenu puissamment dans un passé récent, afin d'aider le monde de la culture, à faire face aux conséquences de la crise sanitaire par un certain nombre de mesures transversales, le mystère de la culture, a pour sa part, apporter une réponse forte et singulière, il faut saluer et qui se prolongera en 2023, afin notamment de permettre aux structures de surmonter les difficultés actuelles, mais l'augmentation des crédits apparaît d'ores et déjà absorbées par l'inflation, chaque programme de la mission bénéficie d'un amendement le programme 175 consacrée au Patrimoine finances comme vous le savez, les politiques de préservation et d'enrichissement du Patrimoine. Sur le français dans ce cadre, il est prévu l'accroissement des moyens alloués au fonds incitatifs et partenariale pour les collectivités, a fait le potentiel financier, le renforcement du plan de sécurité cathédrale et un soutien renforcé à la politique d'archéologie préventive, ce sont des propositions que nous pouvons approuver l'action de l'État se traduira également par un investissement accru dans la rénovation et la modernisation des établissements culturels avec notamment l'augmentation de trois millions d'euros de la subvention d'investissement du Centre des monuments nationaux ou le renforcement des capacités d'investissement du musée d'Orsay avec 1 virgule 5 millions supplémentaires, je m'en réjouis, ah tu te personnel la création, à travers le programme 131 bénéficie d'une attention particulière avec l'ambition de soutenir l'emploi artistique et les artistes, auteurs, près de 13 millions d'euros sont consacrés à cette action, je voudrais aussi souligner le renforcement des moyens alloués aux opérateurs de la création et la poursuite des projets d'investissements ambitieux dans les institutions emblématique de ce secteur à hauteur de 13,5 millions d'euros, enfin la transmission des savoirs et la démocratisation de la culture, qui doivent être au coeur de notre pacte républicain bénéficie elle aussi d'un soutien renouvelé le Pass culture a désormais trouvé son rythme de croisière et il était censé que chaque jeune collégien ou lycéen, puissent bénéficier d'une offre diversifiée sur l'ensemble du territoire l'effort en faveur de ce dispositif ne doit cependant pas se traduire par la diminution concomitante des moyens alloués aux territoires prioritaires et à l'éducation artistique et culturelle telle ne semble pas pas être le cas concernant cette dernière, à ce jour, elle recouvre des réalités plus très hétérogènes, par les formes qu'elle revêt la pluralité des acteurs impliqués, la diversité des territoires où elle se déploie parce qu'elle est indispensable à la démocratisation de la culture et renforce, égalité des chances, elle doit être soutenue sans réserve, je suis par ailleurs heureuse de constater les efforts budgétaires destinées à améliorer l'attractivité de l'enseignement supérieur, culture, son insertion dans le paysage de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'insertion professionnelle des jeunes diplômés pour autant des difficultés persistantes fait la création, je pense au spectacle vivant privé confronté à de fortes contraintes conjoncturelles, notamment la hausse généralisée des coûts mais aussi des contraintes structurelles avec des pénuries de main-d'Oeuvres récurrente après 2 années catastrophiques en termes d'activité et de recettes, l'année 2022 a été synonyme de reprise en demi-teinte l'équilibre économique des festivals est quant à lui particulièrement dégradée, c'est toute une filière qui s'interroge sur son avenir et son modèle de développement dans ce contexte, il a été demandé, malheureusement sans succès une prolongation du crédit d'impôt, spectacles vivants, au delà de ce crédit d'impôt, il sera judicieux nécessaire de réfléchir au renforcement de la filière musicale et du Centre national de la musique, cependant je ne n'anticiperaient pas sur les propositions que notre collègue Julien Bargeton pourrait être amené à formuler dans le cadre de la mission parlementaire que lui a confié la première ministre. Je ne veux pas conclure cette intervention sans émettre un regret à propos des réserves du gouvernement sur les crédits d'impôt destiné aux différentes filières de la culture, que j'ai défendu en séance samedi en 8 en raison de l'orthodoxie budgétaire, poussé à l'extrême, la plupart d'entre eux n'ont n'a pas pu être prolongée, mettant à mal de nombreux acteurs, il s'agit d'un véritable sur sujet d'inquiétude, même si j'ai obtenu une avancée importante pour les éditeurs de services de vidéo à la demande, mais avouez que c'est une bien maigre consolation, voici mes chers collègues, à grands traits les réflexions que je souhaitais vous soumettre compte rendu compte tenu des mesures positives que comporte le budget de la mission Culture les sénateurs du groupe Les Républicains émettront un avis favorable, je vous remercie. Merci, la parole est maintenant Madame Vanina Paoli-Gagin pour le groupe, les indépendants. Une

Madame la présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, le programme Création dépasse pour la première fois le milliard d'euros de budget c'est une excellente nouvelle, à l'image de la hausse de 7 % des crédits dédiés à la mission Culture les aides exceptionnelles arrivent à leurs fins, mais plusieurs mesures fiscales sont pérennisées jusqu'en 2024 comme le crédit d'impôt pour les représentations théâtrales d'Oeuvres dramatiques par exemple la fréquentation moyenne des lieux de spectacles vivants et des arbitres du visuel restent inférieurs aux niveaux observés en 2019, il est essentiel de consolider la reprise d'activité après la crise Covid et pendant la crise de l'énergie, je souligne les 10 millions d'euros destinés au dispositif feront de nouveau dont l'un des objectifs est de faciliter l'accès à la culture en milieu rural, ce qui nous importe tous ici au Sénat, chers collègues, notre groupe est particulièrement attachée à la démocratisation de l'offre culturelle pour tous et partout. Je rejoins, en revanche, les rapporteurs de la commission qui alerte au sujet de la multiplication des objectifs et des labels qui peuvent souvent brouiller l'action du ministère auprès des professionnels de la culture, nous devons également rester en alerte sur la possibilité d'annulation ou de report de festivals et grands événements de la culture en 2024 causée par l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques, les établissements publics dédiés au Patrimoine nous alerte également sur la probable fermeture pendant les Jeux, ces événements majeurs ne doivent pas causer une crispation de l'offre culturelle, je sais que mes collègues de la commission culture, éducation et communication sont particulièrement mobilisés en ce sens, concernant les mesures en faveur de la transmission des savoirs et de la démocratisation de la culture, je souligne les 50 millions d'euros de mesures nouvelles qui ciblent principalement la jeunesse, c'est une très bonne chose, la jeunesse est notre priorité, la revalorisation des subventions destinées aux écoles nationales est un point très positif, cela permettra de participer à la rénovation thermique des bâtiments, il ne faut pas oublier les écoles d'art territoriales qui nécessite des mesures similaires, les collectivités qui en sont les propriétaires n'ont pas toujours en effet les moyens d'engager d'importantes rénovations, c'est très important pour nos territoires, Madame la Ministre, je me réjouis de la progression du Pass culture la dotation augmente de 9,5 millions d'euros pour atteindre 208 5 millions d'euros pour 2023, rien n'est plus précieux que d'offrir à nos jeunes les moyens d'assouvir leur curiosité en matière d'offre culturelle, les élèves de classes de 6ème et de 5ème, qui s'ajouteront à la liste des bénéficiaires en 2023 pourront en témoigner le programme patrimoines enfin sera doté de 1 virgule 10 milliards d'euros en crédits de paiement pour 2023, soit une augmentation de 7,5 c'est considérable parmi les derniers crédits de paiement qui reste du plan de relance 10 millions d'euros sont destinés au plan cathédrale comme l'ont souligné les rapporteurs, le financement des travaux de conservation et de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris proviennent quasi exclusivement du mécénat, cette situation, Madame la Ministre, m'amène à mentionner la reconversion du site de l'abbaye de Clairvaux, qui se trouve dans mon département de l'Aube, vous le savez, un appel à manifestation d'intérêt a été lancé 3 candidats ont été retenus sont en lice dans le cadre d'un dialogue compétitif l'état Madame la Ministre, prend en charge une partie des travaux avec 2 millions d'euros engagés dans le PLF 2023 pour restaurer le grand le grand cloître mais cet exemple nous appellent à réfléchir sur les moyens de mobiliser davantage les donateurs privés dans le cadre de rénovation du Patrimoine aussi j'ai porté deux amendements concernant le financement de la culture dans ce projet de loi de finances, qui malheureusement n'ont pas prospéré le 1er vise à mobiliser l'épargne des Français par la création d'un livret c'est comme culture pour financer la création artistique et le Patrimoine culturel en région, le second vise à lancer une souscription nationale un peu sur le modèle en l'adaptant, de ce qui a été fait pour la rénovation de Notre-Dame afin de soulager, en fait, le coût des travaux engagés par l'État pour la reconversion Clairvaux j'appelle de mes voeux une réflexion sur le sujet dans les prochains mois, enfin je souligne l'urgence à soutenir la rénovation thermique des bâtiments du Patrimoine qui doivent bénéficier de l'engagement de l'État en faveur de la sobriété énergétique, vous le savez, le coût de l'inaction en matière de transition écologique est astronomique, plus on attend, plus ça coûte cher, les chantiers sont colossaux, mais sont essentielles pour conclure l'augmentation des crédits et bienvenue, les défis sont nombreux et j'appelle de mes voeux un engagement fort de la part du ministère de la culture, notamment pour réduire les inégalités territoriales en matière d'accès à l'offre culturelle et à la création, nous devons également rester vigilant sur les conséquences de la flamme de l'inflation et de la flambée des coûts de l'énergie sur les acteurs culturels les plus fragiles, notre groupe, les indépendants, accueille favorablement ces crédits Culture je vous remercie. Merci, ma parole et maintenant monsieur Thomas Dossus pour cinq minutes pour l'Europe Écologie Solidarité territoire. Madame la présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, l'examen des crédits de la mission Culture s'établit une nouvelle fois dans un contexte d'extrême fragilité d'un secteur en pleine convalescence la crise Covid a profondément bouleversé les pratiques et les fréquentations du public si les fermetures totales les jauges et les débats entre activités essentiels et non essentiels sont aujourd'hui un mauvais souvenir, la fréquentation n'a toujours pas retrouvé son niveau d'avant-crise, moins 15 % par rapport à 2019, que ce soit pour les musées ou les spectacles vivants ou les arts de la scène et ce chiffre n'est qu'une moyenne des écosystèmes culturelle déjà fragiles, sont toujours en pleine incertitude les menaces que font peser les JO sur la saison culturelle 2000 vingt-quatre n'aide pas à retrouver des perspectives rassurantes à cette situation déjà difficile, est venue s'ajouter une autre crise non plus sanitaire mais énergétique et d'approvisionnement, l'explosion des coûts et des factures d'électricité et de gaz ainsi que des matériaux de construction impact très durement les équipements culturels et leurs opérateurs et là encore, les plus petits sont les plus exposés, face à cet état de crise multiple, il faut le reconnaître, l'État a répondu présent, en témoignent les 2 milliards d'euros débloqués pour la culture durant le plan de relance ainsi que les Budgets de la mission culture à proprement parler, en constante augmentation, c'est d'ailleurs toujours le cas cette année, avec une augmentation de 7 % des crédits alloués, bien sûr, ce soutien est loin d'être parfait, on ne peut que regretter les efforts de relance plus important sur le Patrimoine que la création, l'absence de prise en cause de la relation systémique entre acteurs, surtout pour les petites structures associatives ou culturelles ou encore la place de la rénovation énergétique encore limitée dans les Budgets détaillons maintenant, thème par thème, les grandes composantes du budget sur le Patrimoine, tout d'abord, près de la moitié de l'augmentation du budget du programme 175 est due à l'augmentation des coûts et de l'inflation sur toute la chaîne de valeur culturelle, on y retrouve ainsi des coûts en augmentation très forte sur les chantiers de plusieurs sites, comme la cathédrale de Soissons ou de Saint-Louis, de Versailles, ainsi que les dépenses d'électricité qui pourrait augmenter entre plus 128 % et plus 200 85 %, selon les estimations des rapporteur sur la création, ensuite, là aussi, l'effort est présent pour la première fois le budget dépasse désormais la barre symbolique du milliard d'euros, et il faut le saluer l'augmentation vise aussi bien à préserver les marges artistiques des opérateurs et des acteurs culturels face à l'inflation que soutenir l'emploi vient là via la revalorisation du Fonds peps ou encore de plusieurs projets d'investissement et d'aménagement comme le Théâtre national de Chaillot ou la Cité du théâtre la transmission des savoirs programme dans lequel 25 % du budget est consacré au Pass culture à hauteur de 208 5 millions d'euros, alors oui, cette politique du chèque, y compris dans la culture n'est pas l'idéal, il pourrait être en effet mieux cibler, mieux accompagner l'enveloppe pour être aussi plus importante mais tout ce qui concourt à l'éveil culturel de la jeunesse à lui offrir un accès simple à la diversité culturelle du pays, même sans médiation doit être salué, nous l'avons vu dans chacun des programmes, la crise énergétique est une donnée majeure ce qu'on l'on parle de facture énergétique, il ne faut pas oublier les collectivités territoriales, celles-ci représentent en effet 75 % de l'investissement public en direction de la culture 9 8 milliards en tout, contre 3,5 milliards pour l'État, or les directeurs des affaires culturelles en collectivité anticipent des cadrages budgétaires strictes pour l'exercice 2023 et laisse craindre une baisse du budget des collectivités dédié à la culture de 10 à 20 cette situation fait craindre que le volet culturel soit une variable d'ajustement pour les collectivités, si celles-ci ne sont pas suffisamment soutenues en raison de la faible reprise du secteur et malgré les filets de sécurité et autres plans de soutien, voilà pourquoi nous vous proposons, par le biais d'un amendement de soutenir davantage les collectivités pour absorber l'augmentation des factures de leur équipement culturel. nous nous compterons pas de gérer la casse, puisque nous vous proposons aussi également d'aller plus loin dans dans la planification, ce que ne fait pas ce budget, nous souhaitons les l'émergence d'un fonds correctement doté pour enfin enclencher la rénovation énergétique des équipements culturels, plusieurs acteurs culturels ont fait part de leur volonté de s'engager dans cette voie et nous voyons au-delà au-delà de l'aspect climatique que la crise énergétique leur a donné raison, nous soutiendrons naturellement le revendication enfin, Madame la Ministre, je tiens ici à me faire le relais de plusieurs inquiétudes concernant la planification culturel sur le long terme de l'État même si formol formellement, cela n'est pas rattachée à cette mission,

sans fin, comme en témoigne aujourd'hui la situation de métal là chez ma mère de Facebook, madame la ministre, il y a mieux à faire, ne serait-ce que pour la musique, nous en parlerons plus tard dans l'après-midi mais le soutien au CM2 doit être renforcée, que ce soit par le biais d'une fiscalité affectée plus diversifié, ou par un soutien de l'État renforcée, nous attendons ainsi les conclusions de la mission confiée à notre collègue Julien Bargeton le budget que nous examinons, aujourd'hui, est un budget de rémission, un budget qui tentent par encore de pallier des difficultés d'un secteur à l'écosystème, certes riche dans notre pays, mais qui se révèle aussi d'une infinie fragilité, il lui manque le souffle d'une grande relance culturelle nous déterminerons notre position de vote sur le budget culture en fonction des débats sur les amendements, je vous remercie. Merci, la parole est maintenant monsieur Julien Bargeton pour le groupe du Rassemblement démocratique progressiste et indépendant. Merci madame la présidente, mais monsieur le Président, Madame la Ministre, c'est un budget inédit en hausse très forte après déjà des périodes d'augmentation 3,7 milliards de crédits de paiement, soit une hausse record de 255 millions d'euros, presque 7 et demi pour % tous les crédits augmentent d'ailleurs, c'est-à-dire que, effectivement, on pourra avoir parfois des hausses différencier, etc c'est une hausse qui est global : 7,6 pour le Patrimoine, plus de 10 % pour la création, je note que pour la première fois de son existence, ce crédit ce ce ce cette cette enveloppe dépasse le milliard d'euros uniquement pour la création, c'est la première fois depuis que le ministère de la culture existe 6,7 % pour la transmission de la démocratisation 4 virgule 7 % pour le soutien aux politiques transversales, bref ce sont des une hausse globale du ministère et, en plus des eaux ce qui concerne tous, tous ces secteurs. Alors même que l'an dernier les crédits était déjà en augmentation de 8 % il y a donc une hausse structurelle du budget du ministère de la culture, et nous nous en nous nous en réjouissons, alors oui c'est vrai ça intervient dans un contexte d'inflation de crise énergétique qui a été soulignée par les différents interlocuteurs, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a aussi les mesures qui concernent évidemment le le traitement et la réponse à ces, à ces problèmes, des mesures ciblées, cela a été dit, notamment pour faire face au surcoût dans les chantiers a été évoqué la cathédrale de Soissons 20 pour faire face au surcoût mais aussi bien sûr 13 millions de plus pour le château de Villers-Cotterets parce que, hé bien les chantiers culturels avec la hausse des coûts de l'énergie et et l'inflation hé bien sont de plus en plus cher, mais également des hausses pour le pouvoir d'achat des des agents 15 2 millions d'euros pour des mesures catégorielles pour les agents du ministère, la poursuite du plan de rattrapage indemnitaire en direction des corps de catégorie A, plus la mise en oeuvre de la revalorisation de la rémunération des agents contractuels et la mise en place d'un régime indemnitaire pour les enseignants chercheurs des École nationale supérieure d'architecture, donc il y a aussi des mesures qui concernent les personnels des des ministères des hausse globale de hausse pour faire face au contexte et des mesures innovantes dans cet ensemble. Le la phase de de monde nouveau, c'est un programme novateur qui s'adresse aux créateurs qui jouent dans de tous les champs, dans tous les champs de la création contemporaine, le spectacle vivant, les arts visuels, la musique, le Design et etc 10 millions d'euros en plus en 2023 également, bien sûr, les métiers d'art sont concernés 5 millions et demi de plus pour les métiers d'art et puis, il faut rappeler que, en dehors bien sûr sûr des crédits strict du ministère, il y a des dispositifs innovants comme le Loto du Patrimoine qui a permis de lever 100 millions d'euros en 4 ans pour le Patrimoine, dits de proximité, je crois aussi que nous pouvons le le ranger dans la catégorie des dispositions innovantes et utiles pour le secteur culturel, cela permet la poursuite d'investissements dans les institutions emblématiques comme sénateur de Paris, je voudrais bien sûr citer les 5 millions d'euros pour la salle Jean Vilar au Théâtre national de de Chaillot ou encore l'extension de l'institut du du monde arabe, son son agrandissement son réaménagement, un peu plus de de 2 millions d'euros, mais également 15 millions d'euros pour le Palais de la cité, bref, les grands chantiers qui sont effectivement très important, hé bien se poursuivent et prennent de l'ampleur en 2023 grâce à des photos à cet effort budgétaire, alors il a souvent été évoqué, mais je voudrais parler moi aussi du Pass culture parce que le Pass culture sert à gager

il faut vraiment considérer que c'est bien sûr lié à la loi organique relative aux lois de finances, il faut bien trouver un gage mais je regrette que ce soit un peu systématiquement ce gage là qui soient c'est vrai qu'il y a eu des crédits importants en plus de 108 millions d'euros, 9 millions et demi par rapport à la finance 2022, c'est parce que l'expérimentation a montré qu'il qu'il fonctionne et les statistiques parlent d'elles-mêmes en la matière de un 1000000 de jeunes qui sont inscrits sur l'application 14 millions de réservations de produits culturels, qui ont été faits

d'un bien culturel par ce biais, donc c'est une une réussite, alors évidemment, c'était une expérimentation audacieuse et qui a évolué, d'ailleurs, et je crois qu'on peut se s'en sont félicités, beaucoup pensaient que cela allait échouer mais finalement ça a rencontré son son public, elle est aujourd'hui d'ailleurs étendu et le sera encore en aux élèves de 6ème et de 5ème en 2023 le fait de d'avoir accru la part collective du Pass et va dans le bon sens parce que bien sûr le Pass doit être accompagnée également d'une d'une médiation culturelle croit à l'expérience, écrivait William Butler Yeats, prix Nobel de littérature en 1923 il a presque il y a 100 ans, pas tout à fait mais, bientôt, je sais que vous aimez la poésie, Madame la Ministre, en la matière, c'est une alliance entre l'audace et l'expérience, c'est-à-dire que l'expérience peut fournir le fait que même si on tente au début quelque chose par audace, hé bien on en on prend en compte la façon dont l'expérimentation réussi ou non, et on a fait évoluer le passe culture je pense que c'est ensemble comme cela qu'il faut continuer et c'est pour toutes ces raisons, l'augmentation globale et puis les éléments plus particulier que j'ai souligné que notre groupe votera les crédits de la mission, je vous remercie. Monsieur Lucien 100 pour le groupe socialiste, écologiste et républicain, vous avez la parole. C'est Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission, mesdames et messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, le droit de participer à la vie culturelle est rarement considéré comme un droit d'égalité en France la crise sanitaire a pour Avantage d'avoir rendu évident, ce qui est considéré comme essentiel et ce qui ne l'est pas, les crédits alloués à la mission culture a enregistré une hausse remarquable oui les priorités définies pour 2023 semble en phase avec les besoins du secteur est-ce que cela est vraiment le reflet d'une politique ambitieuse, peut-être, Madame la Ministre, ces moyens supplémentaires sont les bienvenues est-ce suffisant, hé bien non, face à l'inflation et à la fin de l'aide de Covid, l'effort doit être plus grand, la France est forte de sa richesse culturelle nous sommes reconnus dans le monde entier, soyons à la hauteur, il y a urgence, les voyants sont au au rouge, l'inégalité face à cette reprise, a de quoi nous inquiéter, il y a un manque de visibilité nos festivals ne sont plus que jamais menacée par la crise énergétique, les petites structures, se demandent si elles survivront à l'hiver, pourquoi le quoi qu'il en coûte si les fermetures définitivement des établissements surviennent en 2023 et peut être bien en 2024 la première source de financement de la culture en France, ce n'est pas l'État, ce sont bel et bien les collectivités territoriales, on le sait, les Budgets de la culture sont généralement les plus concernés et les plus touchés, il est donc plus que jamais nécessaire de soutenir nos nos territoires dans leurs pratiques culturelles oui au fond d'innovation territoriale de 2022, il reste tout de mômes, bon de souligner que sa conception ne répondent pas toujours au renforcement de la contractualisation entre l'État et les collectivités que nous demandons, plusieurs mesures fiscales, ça a été évoqué, visant à favoriser la reprise d'activité sont annoncées outil phare de votre budget le passe culture verra ses crédits augmenter afin d'être accessible dès la 6ème il ne remplacera jamais une politique forte d'éducation et de sensibilisation à la culture, l'utilisation du Pass culture reste fortement inégal en fonction des territoires, il profite encore trop aux industries culturelles, le Pass culture doit être ne doit pas être substitut à l'action de l'État madame la Ministre, vous avez fait de la jeunesse, l'une de vos priorités, nous nous en félicitons, mais attention à l'inachevé, la réforme des Elsa qui suscite l'inquiétude sur nos bancs en est un exemple à la modernisation de ses établissements est indispensable, nous déplorons que de nouveaux moyens mis à disposition pour les bourses ne baissent 10 physique aux étudiants des écoles nationales et pas à celle des écoles territoriale, bien que l'amener 2022, et vu le retour à un format normal des festivals leur avenir n'en est pas moins compromis dépense énergétique inflation des montants des cachets prestations extérieures, absence de personnel qualifié, raréfaction des bénévoles pénurie du matériel, la, la liste des difficultés ne cessent de s'allonger : quelle est la réponse, un engagement de l'État modeste et une coordination avec les collectivités trop faible, la dotation du Fonds festival ne sera injustement pas revalorisée en 2000 23 au regard de l'inflation du coût de l'énergie pire et l'annonce par le ministre de l'Intérieur des possibles annulations et reports des festivals en 2024 en lien avec l'organisation des Jeux olympiques, sans concertation préalable avec les organisateurs Prodiss SMA Syndeac mais également les lieux de festivals, le Hellfest les Vieilles Charrues des Eurockéennes le festival d'Avignon et tous les autres, il est envisagé de changer les dates et d'annuler certains festivals, ceci a jeté le plus grand doute sur les perspectives de ces manifestations, l'inquiétude notre commission est très forte : n'opposons pas le sport à la culture, Madame la Ministre, nous sommes à vos côtés pour que vous fassiez entendre raison au ministre de l'Intérieur et encore plus à la première ministre pour qu'en 2024 le le sport ne soit pas l'opposé à la culture, ce n'est pas l'un ou l'autre mais c'est bien le sport et la culture en même temps, la culture, vecteur d'émancipation, d'épanouissement anime la vie des quartiers et évite les errements à certains de nos jeunes, c'est la culture qui doit venir aux Français et non l'inverse, malgré ces quelques remarques et réticences que vous prendrez sûrement à votre compte et l'évolution positive des moyens mis en oeuvre, mon groupe se prononcera favorablement pour votre budget, je vous remercie de votre attention. Merci, la parole. Est ensuite à monsieur Pierre Ouzoulias pour le groupe communiste, républicain, citoyen écologiste. Madame Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, notre époque est celle de la crise de la médiation, les élus de la République que nous sommes là vivent en permanence et sont ainsi troublé quand l'exécutif décide de consulter directement la nation par l'intermédiaire de citoyens tirés au sort ce déconstruction Nice social est aussi à l'oeuvre dans le domaine culturel et le Pass culture on est l'un des symptômes, il participe de l'illusion qu'un jeune peut être sans médiation, l'acteur de sa propre formation culturelle, réduit à sa fonction de consommateurs, il est douteux qu'il puisse s'extraire de son habitus social pour mettre à profit toutes les potentialités émancipatrices de la culture, la médiation culturelle telle qu'elle avait été pensé par André Malraux, aux origines du ministère de la Culture reposer sur le principe que l'accès à la culture était entravée par des déterminismes sociaux et géographiques et qu'il fallait pour les dépasser, je cite. Allez au devant de ceux qui ne savent pas encore que l'offre culturelle l'est accessible en s'affranchissant de leurs conditions sociales, culturelles, les citoyens accéder alors au droit constitutionnel de l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à la culture, pensé comme une oeuvre de libération, la médiation devait s'exercer au plus près des publics par une étroite collaboration avec les collectivités et les acteurs privés, porté par l'essor des maisons de la culture, cette politique doit aujourd'hui être reconsidérée pour s'adapter aux nouveaux usages ainsi l'enquête réalisée en 2008 sur les pratiques culturelles en France, a montré que le téléphone est devenu le 1er terminal culturel nomades et donc la porte d'entrée principale vers de nombreux univers culturel l'efficacité technique de cet outil et sa large diffusion dans la pompe lation ont beaucoup apporté apporter comme bénéfice ainsi elle expliquent la progression spectaculaire de l'écoute musicale journalière qui a doublé en 10 ans, elle était de 9 % en 1973 et elle est proche aujourd'hui de 60 cette banalisation des supports Audio cache une socialisation de leurs usages, par exemple, les modules en baladodiffusion sont beaucoup plus écouté par les diplômés de l'enseignement supérieur que par les autres, à l'inverse, l'utilisation de l'outil numérique semble préjudiciable à d'autres pratiques culturelles, sans doute parce qu'elles exigent une participation plus active, c'est le cas de la lecture des livres qui en constant déclin ou de la visite des musées et des monuments historiques, je doute que le passe culture puisse contribuer à inverser ces évolutions pour les musées, les monuments, la visite scolaire seraient sans aucun doute plus efficace pour rapprocher les jeunes publics d'un Patrimoine qui leur est de plus en plus étranger je pense personnellement que la crise actuelle du cinéma trouve peut-être certaines de ces causes dans cette particule Ariza Sion de la pratique et dans la perte d'une culture cinématographique, ouverte à la diversité de ses formes d'expression avec une certaine nostalgie, je me demande par quoi ont été remplacés les ciné-clubs des lycées d'antan en 2023, le budget de la culture connaîtra une hausse qui est absolument indéniable, néanmoins, on peut se demander si elle pourra contribuer à la nécessaire adaptation des politiques publiques aux évolutions multiples des pratiques la crise pandémique a montré la fragilité des modèles économiques des grands établissements fondé sur l'illusion qu'ils pourraient trouver leur équilibre sans dotation du ministère l'indispensable régénérescence de la médiation culturelle oblige à s'interroger sur les modalités de la participation de tous les opérateurs du ministère à une politique nationale qui se donnerait pour suprême dessins de rapprocher tous les publics de la culture, autrement dit en termes plus techniques, quelle est la capacité de la délégation générale à la transmission au territoire et la démocratie culturelle de votre ministère, madame la Ministre a influer sur les multiples politiques sectorielles mises en neuf par des agences autonomes et financé par des taxes affectées depuis plusieurs années, la commission de la culture du Sénat alertent les ministres successifs sur la nécessité de redonner du sens au principe du droit d'accès à la culture, l'évolution des pratiques culturelles fait de cette refondation une impérieuse nécessité, je vous remercie. Merci. La parole est maintenant à monsieur Max Brisson pour le groupe Les Républicains. Madame la présidente, madame la Ministre, méthane et messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, j'ai intervient en lieu et place de ciné Boulay-Espéronnier empêchée au dernier moment, je voudrais, Madame la Ministre, que vous fait ce qu'il y ait quelques maladresses à mon propos, je voudrais vous interroger dans 3 directions : et d'abord, la fréquentation des lieux culturels, ce n'est pas l'Automne prometteur que vous annonciez en juin, le bilan est très contrastée, il y a ceux qui sont bien redressés et les autres qui prennent de plein fouet les nouveaux modes de consommation et les nouvelles approches numérique après la dure période de la pandémie pour ne rien arranger, le ministre de l'Intérieur a récemment annoncé pour 2024 l'annulation de toutes les manifestations culturelles en marge des jeux, des 2 questions me viennent alors comment avons-nous pu en arriver à une mesure si radicale, quelles garanties pouvez-vous donner aux organisateurs de manifestations culturelles pour 2024, madame la ministre, il faut les défendre, se tenir à leurs côtés pour leur donner les moyens de faire face à ces défis et pour qu'il puisse aussi s'engager dans une transformation stratégique durable votre projet de budget prend-il vraiment compte un fléchage des crédits alloués pour répondre à la diversité de ces situations on peut parfois en douter d'autant plus qu'à ces évolutions structurelles s'ajoutent les conséquences de la crise de l'énergie et de l'inflation qui ampute amputeront aussi bien les Budgets des organisateurs que ceux des publics et surtout de ceux qui sont les plus fragiles, j'aurais donc vivement que vos crédits ne sont pas mieux fléchées en fonction de cette diversité, je regrette également que de la danse des crédits, on ne sent une inflexion des aides pour aider les acteurs de la culture, à faire face à ces mutations, les aider à Soglo dans ces transformations stratégique durable je voudrais ensuite dire d'homo sur le Patrimoine, j'ai compris que vous n'avez guère apprécié mon commentaire sur la rénovation du château de Villers- Cotterêts, entendons-nous bien : sa réhabilitation n'est pas en question mais vous ne pouvez pas m'empêcher de penser que le projet Cultural culturel est arrivé après la décision présidentielle et le programme légitime de réhabilitation, j'ai eu comme l'impression qu'il fallait remplir une case et que le modem Lyon, pas un projet culturel au coeur de cette réhabilitation, le rapporteur a dit le reste quant aux dépassements budgétaires sur la question du Patrimoine, je voudrais aussi vous rappeler que notre commission était attaché au rôle des ABF et qu'il est souhaitable dans un pays comme le nôtre que le déploiement nécessaire des ENR ne nous conduisent pas aux mêmes erreurs de défiguration des patrimoines et des paysages comme nous avons pu le connaître lors du déploiement d'autres réseaux, il faut donc préserver leur rôle, leur mission et leur présence sur le terrain surtout, comme l'a très bien dit notre rapporteur Sabine très ce réseau exceptionnel ne doit-il pas être renforcée face à l'ampleur de la tâche qui l'a devant lui sa réduction génère des lenteurs et des prises de décisions parfois peu argumenté qui contribuent sur le terrain à des tensions avec les maires, et donc à remettre en cause la pertinence même de leur expertise et de leur raison d'être, j'appelle à votre vigilance espérer que l'excellent rapport de nos collègues admettent talons et Pierre Ouzoulias retiennent l'attention du gouvernement oui dans notre pays une partie de notre Patrimoine est menacée, oui, il est urgent que s'élabore un travail partenarial avec les autorités religieuses, les communes et l'État l'acceptabilité des financements publics communaux et départementaux qui qui est à ce prix et la préservation de ce Patrimoine, l'est également, de même nous regrettons qu'une politique adaptée en matière de rénovation énergétique du Patrimoine historique n'émerge pas de ce budget, comme l'a souligné, notre rapporteur je finirai par Domo sur le Pass culture sa montée en charge, nous comme ou pas une discrimination sociale préoccupante finalement ce Pass culture, prophétise-t-il vraiment à à ceux qui en ont le plus, peut se voir, de se retirent pas nécessaire d'y introduire des conditions de ressources, de même, ne faut-il pas relativiser son succès au vu des inscriptions groupés dans certains nombres d'école voilà quelques mots pour évoquer les crédits de l'une des de mission culture de votre ministère, ils sont en hausse, il faut le saluer, comme l'a fait, Sylvie Robert, notre rapporteur pour avis, je voudrais ajouter un coup de chapeau pour le dialogue que vous souhaitez instaurer avec la Haute, y compris sur le sujet sensible des restitutions et de la préservation des collections nationales, vous trouverez ici une assemblée intransigeante sur les principes et ouverte sur les modalités, je vous remets. Merci, la parole est maintenant madame. Marie-Pierre Meunier pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, les difficultés incertitude de la période actuelle n'épargne aucun secteur, y compris celui du Patrimoine, la crise sanitaire avait été l'occasion d'apporter des réponses justes, notamment en matière de soutien public aux activités les plus fragilisées ainsi le plan de relance a permis à la fois d'accroître fortement les crédits alloués au Patrimoine et d'engendrer une dynamique générale dans les activités du secteur bénéficiera encore en 2023 aussi, nous saluons l'augmentation des crédits du programme 175 à un rythme équivalent à celui de l'ensemble de la mission, soit de 7 % par rapport à l'an dernier, néanmoins, cette hausse doit être relativisée car ces crédits ne seront plus complété par ceux du plan de relance qui avait permis de dégager 227 millions d'euros supplémentaires pour le Patrimoine et la hausse qui représente 77 millions cette année ne compensera que partiellement ce montant, cette situation fait donc naître des inquiétudes quant à la capacité de ce budget à pouvoir accompagner des acteurs du Patrimoine qui vont devoir faire face à l'inflation à l'explosion des tarifs de l'énergie mais aussi à la poursuite de la dynamique d'investissement initiée par le plan de relance ainsi l'envolée des prix de l'énergie va continuer à peser fortement en 2023 sur l'équilibre financier des structures telles que les musées et les monuments parallèlement pour de nombreuses collectivités et notamment les plus petites d'entre elles, le Patrimoine ne sera peut être pas parmi les premières priorités, elles auront besoin d'un soutien plus affirmé de l'État pour assurer la sauvegarde et l'entretien du Patrimoine dont elles ont la charge mon défendant lors de chaque PLF une répartition plus équilibrée sur les territoires des crédits cette année, nous notons avec satisfaction que l'augmentation des crédits en faveur de l'entretien de la restauration des monuments historiques hors grands projets profite essentiellement en moyenne mise à disposition des Drac pour la restauration de monuments historiques appartenant à l'État parallèlement les moyens, les moyens du fonds incitatifs et partenariat pour les monuments historiques des collectivités à faibles ressources sont inscrits de 2 millions nous souhaitons néanmoins attirer votre attention sur le mode de répartition de l'enveloppe de crédits locaux entre les différents projets, en effet, il semble que les grosses opérations quoi en ce moment, parfois plus de 50 % de l'enveloppe sont favorisés, or une telle choix est nécessairement au détriment d'autres opérations de dimension plus restreinte peu de travaux d'entretien des monuments sont réalisés et les communes et le moins versé sur le Patrimoine ne sont pas encouragés à déposer des dossiers notre point de vigilance et celui des moyens humains, des services déconcentrés de l'État départementaux des Drac et des dac car moins de personnel qualifié, c'est forcément moins de soutien aux petites collectivités ne pouvons que regretter une nouvelle fois que les crédits pour l'architecture et les espaces protégés soit en stagnation, qu'il s'agisse de reconquête des centre-ville ou de transition énergétique de l'habitat ancien le dispositif site patrimonial remarquable est un outil très efficace qui mériterait que le ministère s'en saisisse réellement j'en terminerai avec les crédits en faveur du Patrimoine archéologique qui exprime un soutien continu de l'archéologie préventive et des missions de service public, réalisée par l'Inrap et les services d'archéologie des collectivités territoriales, toutefois le surcroît d'activité d'aménagement qui suit le plan de relance nécessite des fonds supplémentaires afin de pouvoir continuer de repeindre, répondre aux demandes sans allonger les délais délais de chantier, enfin nous saluons les augmentations des crédits à destination des de conservation et d'études et pour le soutien aux fouilles archéologiques programmés en partenariat avec le CNRS et les universités, pour conclure, si ce budget reste un budget de soutien aux actions de valorisation et de protection du Patrimoine, nous émettons des réserves quant à sa capacité à répondre totalement aux difficultés auxquelles sont confrontés ces actes. Si la parole est maintenant madame elle se Joseph pour quatre minutes et pour le groupe Les Républicains. Madame la présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, malgré 2 années difficiles, l'accès à la culture, le soutien au Patrimoine doivent pouvoir connaître un rebond, nous sommes dans la suite des actions menées dans le cadre du plan de relance avec une reprise timide et des pratiques culturelles qui change le mécénat diminue et certaines aides de nos régions aussi si nous saluons la hausse des crédits, nous regrettons le risque qu'elle soit neutralisée par l'inflation, nous ressentons une certaine déception ces surcoûts annoncés sont rédhibitoires éloigneront certains publics de l'accès à la culture. Si nous saluons bien sûr, l'augmentation des crédits du programme patrimoines, il faut réfléchir à quelque chose de plus ambitieux dans les rénovations et réhabilitations dans nos territoires, il y a quelques mois, avec mon collègue Olivier Paccaud nous avions rappelé l'importance du Patrimoine privé et du Patrimoine local, les crédits doivent aussi bénéficier à ce Patrimoine de proximité, l'innovation culturelle se fait dans les territoires, c'est une clé pour la reprise et pour le soutien à la vie locale, un vrai signal. Il faut encourager toutes les solutions qui permettent aux citoyens de financer des projets, le Loto du Patrimoine, on a été une mais il ne doit pas rester la seule les circuits courts, cela peut aussi fonctionner dans le Patrimoine, il faut permettre un financement Direct, les services de l'État doivent pouvoir parler aux acteurs locaux sont filtrés appuyer les projets de nos collectivités, même s'il faut saluer la prise en compte de la crise énergétique, il faut aussi constater la majoration des coûts dans les chantiers, l'avenir de la culture, c'est d'abord la question à son accès. La reprise des accès au musée est un signe positif, mais des incertitudes pèsent sur leur fréquentation et sur l'amplitude d'ouverture, cela vaut aussi pour la jeunesse, ce qui nous amène au Pass culture et la question de la création et la découverte du patrimoine c'est une aide appréciable mais la médaille a son revers, je dirais même que fâcheusement : on se rapproche un peu de la politique du carnet de chèques, c'est quelque chose qui profite à tous, mais la difficulté que cela Avantage les initiés, c'est-à-dire ceux qui savent déjà ce qu'ils vont faire le jeune qui aime les livres qui aiment les musées, essayer de quelle manière il va utiliser le Pass mais celui qui n'a pas d'idée ne saura comment recourir à cette aide, c'est donc plus une démarche confirme matrice que créatrice de démarche culturelle et du point de vue de l'éducation artistique, on ne peut que déplorer une baisse des fonds et ainsi une démarche qu'construite avec l'éducation nationale, plutôt que des fonds qui s'additionnent me paraît plus judicieuse. Je souhaite bien sûr attirer l'attention sur les festivals, ils ont bien résisté malgré 2 années rudes comme les acteurs de ce secteur, l'ont indiqué, ils ont été les premiers à fermer les derniers à ouvrir au bout de ces 2 années, les publics sont globalement restés fidèles au rendez-vous et c'est heureux, même si nous déplorons la disparition de certains festivals, l'offre est restée abondante, mais pour combien de temps encore. à peine est-on sorti de cette crise que de nouvelles difficultés pointent leur nez avec un heureux événement : l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques 2024 sans pour autant opposer le sport à la culture et sont créés, bien sûr, de rivalité entre les événements nos regrettons un manque de visibilité et une absence de dialogue entre tous les partenaires concernés, les festivals sont tributaires d'aléas et leurs répétitions de toutes sortes, interroges, il a été envisagé de réfléchir à un système d'assurance qui prendrait non seulement les risques artistiques mais aussi climatique peut être est-ce une piste à explorer je ne pose pas le risque à la protection, mais comment se lancer durablement, si les perspectives sont sombres sans cette assurance, et cela vaut dans tous les sens du terme, le risque est tout simplement que les festivals fasse les frais de la loi du marché qu'on essayé des bénévoles de l'engagement des collectivités territoriales, avec ce manque de visibilité et de perspectives un festival se prépare au minimum 2 ans à l'avance, soutenons festival qui ne doivent pas faire les frais de ces nouvelles contraintes, nous regrettons toujours l'absence de référent festival tant au niveau national que régional, alors que c'est un sujet brûlant pour l'orientation des politiques culturelles et la défense de l'accès à la culture sur tout le territoire quelle place voulons-nous donner à la culture dans notre société, soyons ambitieux et inventif, nous voterons les crédits de la mission Culture malgré certaines insuffisances et de nombreuses réserves, nous comptons sur vous pour gagner ses arbitrages nécessaires. Si Madame la Ministre, c'est à vous. Madame la présidente, monsieur le président de la commission, cher Laurent Lafon, messieurs les rapporteurs spéciaux cher Vincent Eblé Didier Rambaud mesdames et messieurs les rapporteurs pour avis, mesdames et messieurs les sénateurs, j'avais mon masque, je l'ai enlevé parce que je viens d'avoir mon résultat de test PCR qui est négatif, juste pour vous expliquer et que vous n'ayez pas d'inquiétude. Hormis cette bonne nouvelle, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour la vraie. Bonne nouvelle de la journée, ce budget du ministère de la culture que nous allons étudier pour la première partie, la mission culture qui est en hausse assez historique, je voudrais avant de commencer ma présentation vraiment vous remercier pour tous les échanges constructifs. Et très précis que nous avons eu au fil des derniers mois, que ce soit en commission ou lors des rendez-vous bilatéraux que nous avons pu avoir ce sont à chaque fois des moments très utile et je salue aussi la qualité de vos rapports qui sont des sources d'inspiration pour nos travaux au quotidien, vous l'avez tous dit : Le monde de la culture vient de traverser 2 ans de pandémie. Dont on ressent encore les effets aujourd'hui mais il reste plus résiliant plus fort que dans de nombreux pays, y compris de nos voisins européens, grâce à toutes les aides qui ont pu être déployés par l'État pendant la crise grâce aussi à cette capacité d'innovation permanente et de lien avec les publics que les lieux culturels, l'ensemble de l'écosystème de la culture, a pu porter et et maintenir. Mais bien avant cette crise sanitaire, une autre révolution est venue impacter le monde de la culture, depuis même 10, 20, un peu plus que ça, au moins 20 ans c'est la révolution numérique qui est à la fois porteuse d'opportunités, mais aussi de menace pour la création, pour les auteurs pour les créateurs. La crise sanitaire, au fond, est venue accélérer ces mutations qui était déjà en germe notamment elle à amplifier la puissance des géants du numérique et à la souligné les inégalités sociales, de l'accès à la culture. Nous, si nous regardons les études décennale du ministère de la culture, c'est un outil très précieux pour voir les évolutions structurelles cette étude sur les pratiques culturelles des Français, a montré en réalité une fracture générationnelle qui se creuse certes accélérée par la pandémie mais présente bien avant qu'on pourrait résumer ainsi aux plus âgés, une culture de sortie vers les musées, les spectacles et cetera et aux plus jeunes une culture qu'on pourrait qualifier de salon avec cette addiction aux écrans qui se développe mais qui ne se limite pas qu'à la jeunesse, c'est vraiment aujourd'hui à toute la population qu'on doit donner et redonner envie de culture en Chair et en os. C'est l'ambition, en tout cas que je porte au ministère de la culture et c'est pour ça que ce budget est historiquement haut puisque il est aujourd'hui à 3 7 milliards d'euros de crédits pour la mission culture soit 7,4 pour 100 de plus que l'année passée, vous le savez, au-delà des crédits de la mission culture, on y reviendra plus tard dans la journée puisque nous allons étudier les les crédits de la mission Médias livre et industries culturelles qui s'élève à 704 millions d'euros, plus 3 virgule 8 milliards d'euros consacré à l'audiovisuel public, j'ajoute à cela 769 millions d'euros de taxes affectées et près de 2 milliards d'euros de dépenses fiscales, j'ai bien entendu vos inquiétudes chère Laure Darcos au sujet de la pérennité de certains crédits d'impôt, vous savez qu'aujourd'hui la position du gouvernement est de permettre une évaluation la plus précise possible avant de pouvoir en rediscuter mais nous serons très vigilants au total si j'additionne toutes ces enveloppes, ce sont 11 milliards d'euros de financements dont le ministère de la culture à la responsabilité et qui permettent d'injecter toute l'ambition que nous voulons porter pour la politique culturelle de ce pays, le budget que je vous présente se veut réellement un budget de résilience et d'action résilience que vous l'avez tous dit nous sommes encore en convalescence post-pandémie et nous devons accompagner l'ensemble des secteurs culturels pour faire face à ces défis dans dans ces défis du présent, il y a également la crise énergétique, vous l'avez largement mentionné, c'est une priorité de ce budget avec 56 millions d'euros débloqués pour répondre aux besoins, aux besoins immédiats du contexte énergétique que nous connaissons mais c'est aussi un budget d'action pour préparer l'avenir et, si je reste sur cet exemple de la sobriété énergétique et de cette priorité pour la transition écologique, ce budget permet d'investir à plus long terme pour des travaux assez significatif dans cette perspective d'une meilleure isolation thermique des bâtiments et d'une amélioration des performances énergétiques des bâtiments culturels, c'est pour ça que le budget d'investissement de la mission Culture s'élève en 2023 à 627 millions d'euros, en augmentation de 70 millions avec notamment des exemples que certains d'entre vous citer par exemple les travaux du musée d'Orsay du Théâtre national de Chaillot, je pourrais citer aussi l'école d'architecture de Limoges ou celle de Lille, tous ces travaux se sont que quelques exemples, vise à améliorer la performance énergétique des bâtiments donc baisser à terme leur facture d'énergie et à à engager cet énorme chantier de décarbonation de la culture, que j'ai placé au coeur de mes priorités décarbonation de la culture et conciliation, je vous rejoins totalement sur cette nécessité de concilier le Patrimoine sa préservation sa valorisation et le développement des énergies renouvelables, nous sommes en ce moment en train de travailler sur une instruction par exemple pour l'intégration des panneaux photovoltaïques dans une démarche respectueuse de la préservation du Patrimoine, c'est tout à fait possible de concilier les 2. Ce budget pour ne pas être trop longue, je voulais vous le présentez autour de quelques grandes priorités qui me tiennent à coeur : j'en ai choisi 5 l'éducation artistique, la souveraineté, le Patrimoine, l'emploi et l'international. Concernant l'éducation artistique, je vous remercie tous d'en avoir parlé, car nous sommes réunis je pense ici par cet enjeu crucial, qui est de sensibiliser dès le plus jeune âge, les jeunes générations à tous les possibilités d'émancipation et de développement d'esprit critique et de confiance en soi que permet la culture dans le budget 2023, ce sont 14 millions supplémentaires qui sont dédiés à cette priorité avec 4 millions pour l'éducation artistique, or pas sculptures pardonnez-moi pour le Pass culture, vous vous en avez largement parlé, je voudrais insister sur le fait que ce Pass culture est un nouveau Pass culture depuis quelques mois, c'est un Pass culture plus collectif, plus participatif avec cette dimension de Pass culture pour les classes au collège avec vingt-cinq euros par élève pour chaque enseignant, on peut voir à ce titre d'ailleurs que ce qui arrive en 1er dans les sorties scolaires des tous les chiffres qui nous remonte, c'est bien le spectacle vivant, le théâtre qui avait plus de mal à arriver en tête pour le Pass culture individuelle et nous avons aujourd'hui 2 2 millions de jeunes inscrits pour le Pass culture individuelle la part personnelle du Pass culture ce qui est colossal et vraiment, j'insiste sur le fait, cher Didier Rambaud, que ça n'est pas une plateforme d'achat, je vous rejoins sur cette ambition-là, c'est un outil aussi pour faire participer les jeunes pour les engager en faire des protagonistes, pas uniquement des consommateurs cher aussi monsieur Ouzoulias, vous le savez, à l'époque de Malraux, internet et les smartphones n'existaient pas, donc évidemment que le l'enjeu de la médiation. Il est au coeur de nos politiques, mais aujourd'hui vous avez vous-même démontré à quel point le Pass culture répond en fait à ce nouvel usage qui est que tous les jeunes ont un smartphone d'ailleurs nous aussi les adultes et nous voyons bien cette addiction à ces machines et que ces via ces machines aussi que nous devons les toucher, mais le Pass culture à développer des parcours un cercle d'ambassadeurs des des expériences qui permettent d'aller bien au-delà du simple acte d'achat du clic d'achat je pourrais revenir dans les réponses aux amendements, si vous le souhaitez, je voudrais aussi vous signaler que ce Pass culture devient de plus en plus européen et c'est une très bonne nouvelle, l'Espagne, j'ai été au mois de septembre, a lancé son bonus coup le tour, hein, et l'Allemagne, j'ai été il y a 3 jours, a également décidé de mettre en place un Pass culture un coup tour Pasquier complètement calqué la affirme comme telle sur le Pass culture français plus nous serons nombreux à le porter plus les jeunes Européens seront reliés aussi par cette nouvelle ambition culturelle. 2ème priorité. Qui me tient à coeur et dont je voulais vous parler, c'est celle de la souveraineté culturelle souveraineté que je vois à la fois dans le monde physique pour soutenir la création, soutenir les métiers d'art, soutenir la langue française, soutenir la création avec le programme mon nouveau mais je vois aussi dans le monde numérique et c'est vrai que le plan France 2030 or de ce budget est là aussi pour nous aider à investir sur des studios de tournage sur des formations nouvelles sur des expériences immersives en lien aussi avec les expériences physiques et sur ce que sera plus tard, le métavers, mais dans une approche française une approche sensorielle, une approche aussi qui défend la liberté d'expression et de création, j'y tiens beaucoup, merci en tout cas, Julien Bargeton, d'avoir insisté sur le plan métiers d'art qui me tient très à coeur et dont on voit une amorce dans ce budget 2023, avec une augmentation du soutien aux manufactures nationales Sèvres et le Mobilier national, qui sont un peu les fleurons de nos manufactures pour pouvoir porter une partie de ce nouveau plan pour les métiers d'art sur lequel j'aurai l'occasion de revenir, je voulais insiste également sur l'enjeu de la langue française et dans ce budget, vous avez vu qu'il y a une légère hausse pour accompagner en plus de l'important investissement en travaux, en travaux, le l'ouverture au printemps 2023 de la Cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts j'y été samedi pour faire le point sur le chantier, échanger avec les élus, c'est un projet qui avance très bien et merci monsieur Brisson de redire tout votre attachement à ce projet, je voulais juste vous préciser que, dès le 17 mars 2017. Le les présidents de la République, il était candidat à l'époque, Emmanuel Macron, avait fait un discours à Reims où il l'avait déjà dit que le projet serait un projet dédié à la langue française, donc ça n'est pas venu après, ça a été d'abord une intuition forte de sauver ce château et de le sauver pour un projet dédié à la langue française. étant donné aussi l'histoire de cette ville de naissance d'Alexandre Dumas et de ce château où a eu lieu l'ordonnance de Villers-Cotterêts, le temps file je voudrais vous parler également de l'importance du Patrimoine dans ce budget, qui atteint un budget historique de plus d'un milliard d'euros avec, vous l'avez tous dit l'enjeu des cathédrales leur sécurisation leur restauration, le soutien aux monuments historiques dans tous les territoires des crédits pour des projets emblématiques en région comme la reconversion de l'ancienne abbaye de Clairvaux, avec 15 millions d'euros en en autorisations d'engagement Vanina Paoli-Gagin un effort aussi pour les dispositifs qui accompagne les collectivités territoriales, le fameux Philippe le fonds incitatifs pour le Patrimoine qui en augmentation ou encore la hausse aussi des fouilles programmées et des diagnostics archéologiques auquel nous sommes tous très attachés. 4ème priorité : l'emploi, les compétences, ce budget, j'ai voulu vraiment m'attacher à ce que, ils puissent permettent de d'accompagner les futurs talents et de structurer mieux notre politique d'accompagnement à l'emploi avec une priorité majeure qui est celle des écoles, les établissements d'enseignement supérieur artistique et parmi elles, les écoles d'architecture, c'est quand même un vivier de 20000 étudiants un vivier extraordinaire qui seront les bâtisseurs de demain, les penseurs des villes et des logements de demain, donc il y a un effort très particulier pour les écoles d'architecture dans ce budget, je ne reviens pas, vous l'avez mentionné les bourses, les os des travaux de mise aux normes, les crédits supplémentaires aussi pour hors école l'emploi artistique, les artistes, auteurs, je ne détaille pas tout ce que vous avez déjà dit les moyens du ministère sont eux aussi conforter la masse salariale va augmenter de 38 millions d'euros pour atteindre 532 millions d'euros avec une trajectoire d'emplois stable, le ministère de la culture, c'est 29000 agents dévouée passionnée dont 20705 pour la mission culture qui nous occupe en ce moment quelques mots enfin sur la politique internationale, nous en avons beaucoup parlé en commission et je sais votre attachement à l'action culturelle extérieure de la France, même si elle relève en grande partie du ministère des Affaires étrangères, le ministère de la culture, il y a toute sa part via l'ensemble de nos établissements, qui ont tous pour les plus grands d'entre eux, mais même pour les plus modestes, des équipes qui travaillent en lien avec leurs partenaires internationaux, le budget en en 2023 est en hausse de 17 par rapport à 2000 22 et nous permettra de soutenir la diversité culturelle dans un certain nombre de programmes d'échange avec des pays de plus en plus nombreux, je pense à l'Algérie, je pense au continent africain, je pense au pays du monde francophone et à d'autres, mais aussi d'être au rendez-vous de la solidarité, que la France a toujours montré avec les pays où des artistes sont menacés pour créer, sont menacés dans leur liberté d'expression, ont été contraints de fuir suite à la guerre, je pense à l'Ukraine, je pense à l'Afghanistan, je pense à l'Iran et à tant d'autres pays, voilà, Mesdames et messieurs les sénateurs, les quelques priorités de la mission culture de ce projet de loi de finances pour 2023 sur lesquels je voulais insister, c'est un budget ambitieux, je l'ai dit, en forte hausse, qui nous permettra de répondre aux grands défis du présent, mais aussi de l'avenir de continuer à porter une voix forte dans le monde quinze minutes c'est court pour partager avec vous toutes mes convictions, toutes mes priorités mais avant de passer à l'examen des amendements, je voulais vous adresser un dernier message par le biais d'un poème, c'est devenu notre rituel un poème de Jean Pierre Siméon. Je cherche un mot vaste et chaud comme une chambre sonore comme une harpe dansant comme une robe claire comme un avril un mot que rien n'efface comme une empreinte dans les Corses un mot que le mensonge ne séduit pas un mot, pour tout dire la mort, la vie, la peur, le silence et la plainte l'invisible et le Doubs et les miracles de l'été, depuis si longtemps, je cherche mais j'ai confiance en vous, il va naître de vos lèvres merci. ça. Chers

en conséquence nous si nous n'avions pas terminé l'examen de cette mission à 18 heures 10 elle se poursuivraient à la fin d'émission de cette semaine et nous passerions à la directement à l'examen de la mission Médias livre et industries culturelles en revanche se terminons avant le terme de la durée d'examen de la mission suivante pourra commencer sans attends, nous allons procéder à l'examen des amendements portant sur les crédits de la mission Culture figurant à l'état B et nous commençons avec un amendement du gouvernement, Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, l'amendement que je vous présente à 2 volets : d'une part sur le plan rédactionnel, il vise à annuler la création d'un 5ème programme budgétaire au sein de la mission culture qui était intitulée éducation aux médias hier l'information, et qui était très faiblement dotée il est proposé de repositionner les crédits initialement ouvert pour la création de ce programme budgétaire 500000 euros vers le programme 361 transmission des savoirs et démocratisation de la culture au sein duquel l'éducation aux médias et à l'information constituent un domaine prioritaire d'action et sur lequel les ouvertures sur le programme, nouvellement créée, avait été initialement engagé ça ça fait suite à un amendement de Violette Spillebout, à l'Assemblée, d'autre part, il tire cet amendement, les conséquences de l'adoption de plusieurs amendements parlementaires déposée et adoptée à l'Assemblée nationale en ressent de 3 millions d'euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, le programme, soutien aux politiques du ministère de la culture de la mission culture au titre du développement du Pass culture en Nouvelle-Calédonie, c'était l'amendement de Nicolas Metzdorf, d'une aide pour les collectivités territoriales afin d'assurer l'entretien et la valorisation du Patrimoine local, un amendement de Frédéric Maillot un 1000000 d'euros, là aussi, et enfin de soutenir une politique de recrutement au sein des fanfares un amendement d'Alexandre Portier à un 1000000 d'euros qui vient compléter notre plan fanfare que j'avais annoncé en reconduction à hauteur de 1 1000000 d'euros par an, voilà pour cet amendement du gouvernement, quel est l'avis de la commission. Madame la présidente, il s'agit d'un amendement de coordination budgétaire qui tire les conséquences budgétaires des des amendements retenus par le gouvernement dans le texte adopté à l'Assemblée, donc un avis favorable. Je mets aux voix cet amendement du gouvernement avec avis favorable de la commission qui est pour, qui est contre qui s'abstient, il était adopté, le 507 Monsieur Bruillet. Merci, Madame le Ministre, vous avez évoqué l'enjeu décarbonation culture bienvenue et les moyens consacrés aux équipements nationaux notre amendement vise à soutenir les politiques culturelles des collectivités et des associations qu'elles soutiennent face à la hausse des prix de l'énergie, vous le savez les collectivités dont les finances sont déjà sous tension subissent également l'augmentation des coûts de l'énergie, parfois contrainte d'amputer des politiques culturelles de diminuer les tranches les plages horaires d'ouverture de certains équipements pénalisant parfois des coopérations avec les scolaires, le soutien à des tiers lieux ou à des universités populaires dans les exemples qui me sont revenus, nous vous proposons donc de créer un fonds d'aide pour accompagner les collectivités leur permettent de continuer à soutenir ce maillage culturel local qu'elles assurent quotidiennement les politiques publiques culturelles sont essentielles et nous partageons cet avis à l'essor d'une démocratie culturelle, elles doivent rester fortes et assumées et surtout ne pas devenir une variable d'ajustement dans cette période de grave crise budgétaire. La commission. C'est une demande de retrait puisqu'il nous semble que cet objectif auquel il est possible de souscrire, bien entendu, parfaitement pris en compte par les crédits du plan de relance depuis 2021, par ailleurs, le dispositif est gagé sur l'intégralité des crédits du Pass culture, ça nous semble je serai être un dommage collatéral, donc c'est une demande de retrait sinon défavorable. Madame la ministre, l'avis du gouvernement. Je rejoins merci madame la présidente, l'avis du rapporteur, effectivement, nous avons déjà pris en compte en large partie un certain nombre de situations très difficiles en matière de d'impact de du coût de l'énergie pour certains opérateurs évidemment qu'en priorité, l'État étant seul à financer certains opérateurs, nous devons nous préoccuper de ce que nous sommes seuls à financer, mais dans cette enveloppe, nous regarderons avec nos Drake les cas les plus critiques, y compris pour les structures cofinancé avec les collectivités, donc nous serons au rendez-vous, autant que possible des cas les plus critiques, j'en profite aussi pour vous signaler un appel à projets, qui s'appelle alternative verte dans le cadre du plan France 2030, qui est doté de 10 millions d'euros déjà attribuées et que nous allons reconduire à hauteur de 10 millions d'euros pour financer la des projets de décarbonation de la culture qui permettront à plus long terme, 2 structurellement baisser ses factures d'énergie, je vous remercie avis demande de retrait sinon défavorable merci de ces réponses, pour le rapporteur spécial, à l'évidence le gage n'était pas fait pour diminuer les, les, les crédits, c'est la règle pour échapper à l'article 40 je vais je vais maintenir cet amendement parce que je garde une inquiétude, Madame la Ministre, sur ce que ce que seront le soutien aux collectivités territoriales, après le 49 3 puisque, malheureusement, on n'est pas garantie des résultats, donc, mais j'ai bien entendu la la réponse, c'est l'hypothèse que le fond que vous, consacré aux équipements nationaux puissent éventuellement être utilisé pour d'autres équipements ayant convention avec les Drac, je préfère maintenir l'amendement par précaution. Si je mets aux voix cet amendement double avis défavorable qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient n'est pas adopté le 528 Monsieur dessus. Merci madame la présidente de c'est un abonnement, un amendement complémentaire au au précédent pour un dispositif plus pérenne, donc on le sait, la rénovation énergétique du bâti d'un enjeu fondamental pour la transition avec la défaite, la nécessité de réduire les factures, mais aussi et surtout limiter les consommations pour réduire l'impact environnemental, mais hormis le bâti il y a beaucoup à faire, par exemple sur les déplacements des spectateurs, des artistes ou des prestataires sur les possibles mise en commun des ressources pour éviter des consommations superflues sur le degré de sobriété à mettre en oeuvre en terme de chauffage ou d'illumination et tout cela les les acteurs culturels en sont bien conscients puisque lors du traditionnel débat de clôture du festival d'Avignon, cette année, c'est toute une filière qui a appelé à s'engager pour la transition écologique du spectacle vivant. Ils sont prêts à s'engager mais il demande un soutien, notamment financier de leur ministère et c'est précisément le but de cet amendement et donc nous, nous proposons la mise en oeuvre d'un fonds de 50 millions d'euros pour la transition du spectacle vivant, afin de permettre aux acteurs de réaliser leurs ambitions louables et nécessaires, je vous remercie. La commission a émis un avis de demandes de retrait et il nous semble que là encore le plan de relance, a mis en place un fonds pour les institutions de la création en région sur la période 2021 2022, et donc il apparaît opportun à la commission des finances d'attendent les résultats de l'exécution 2022 pour évaluer les modalités éventuelle de reconduction d'un tel dispositif et évaluer les besoins, les attentes qui pourrait s'exprimer : demande de retrait. Madame la Ministre même avis Vous maintenez je mets aux voix double avis défavorable qui est pour. Qui est contre qui s'abstient n'est pas adopté le 656 monsieur Oui à un amendement de Nathalie Delattre sur le Pass culture qui rencontre un grand succès auprès des jeunes, depuis son lancement en 2019 plus 10 millions de réservations d'offres ont été déposées par près de 11000 acteurs culturels, les achats soutiennent les diverses composantes du secteur culturel cependant les prestataires n'en tire pas tous les mêmes bénéfices on demande en particulier aux acteurs digitaux de proposer une offre gratuite pour être référencé au Pass culture sans contrepartie dans ces conditions, aujourd'hui, quand un jeune utilise son passes s'il achète un livre le compte du jeune et débité en fonction, le commerçant est payé les ayants droit sont payés s'il achète un livre numérique, c'est la même chose, mais s'il achète un compte tenu d'Audio numérique le compte du jeune et débité en fonction mais le prestataire, n'est pas payé et le prestataire payent les droits d'auteur, cette situation fragilise clairement certains modèles économiques de plateformes numériques françaises par ailleurs cette politique l'Audio numérique par rapport aux autres biens culturels, alors qu'il est aujourd'hui le support économique incontournable de l'industrie musicale, l'amendement propose par un fléchage à hauteur de 10 millions d'euros d'inciter le gouvernement à rétribuer les Oeuvres culturelles numériques Audio sur le dispositif du Pass culture de la même façon que les autres offres. La présidente, ce sera clairement une demande de retrait, je veux dire à à Bernard fier que ce cet amendement, ça renvoie à la file de à la philosophie même du du Pass culture le le le Pass culture, c'est un outil qui doit permettre de faire évoluer les pratiques culturelles garage, garantir des des rentes de situation à à des plateformes que connaissent déjà les jeunes en découle donc cette logique de non remboursement et puis notons par ailleurs que la la musique enregistrée ne représentent que 9 % des achats qui sont effectués sur l'application, donc il ne nous sont pas utile de de revenir sur ce point, voilà donc je confirme demande de retrait. Avis du gouvernement. Merci madame la présidente, oui même avis et je voulais vous préciser que les les acteurs numériques monsieur Fiole air quand le Pass culture a été conçu, ont été considérés comme des partenaires de de ce dispositif. Et ont accepté ce principe de non-remboursement avant même de s'inscrire au même sur le Pass culture, ça fait partie de cette petite part d'autofinancement du du du Pass culture par. Au large, budget de l'État qui vient en appui, donc, et vous le savez le le plafond et le les dépenses des jeunes dans le numérique sur le Pass culture sont plafonnés à 100 euros et comme ça vient d'être rappelé, c'est effectivement de très faible montant à à ce stade une évolution ne paraît pas indispensable mais nous resterons évidemment vigilants à l'avenir. Oui, madame la président cet amendement vise à souligner l'insuffisance du financement de l'archéologie préventive, renforcée par l'inflation, si les subventions destinées aux 62 collectivités habilité à réaliser des diagnostics archéologiques ont été accrus, cette augmentation demeure insuffisante, notamment compte tenu de l'inflation pour financer à la hauteur de leurs besoins des opérateurs publics singulièrement les collectivités en charge de cette mission et donc proposé de rattraper ce besoin par un amendement de crédit en abondant le programme 175 patrimoines à hauteur de 8 millions d'euros afin que ces crédits bénéficier ensuite à l'action neuf Patrimoine archéologique sera rate ce rattrapage me semble d'autant plus justifiée que 2 amendements suivront afin d'augmenter les moyens de l'Inrap par parallélisme, ceux des collectivités doivent donc l'être aussi, si les règles de recevabilité budgétaire m'oblige à gager cette proposition par un transfert de crédits provenant d'autres programmes de la mission, en l'occurrence le passe culture je souhaite néanmoins la levée du gage et la pérennité des autres dispositions de cette mission. Je vous remercie, le projet de loi de finances prévoit environ 9 millions d'euros au titre des dépenses de soutien aux fouilles archéologiques programmés réalisés par les collectivités territoriales, en partenariat avec d'autres organismes, ce montant progresse de 4 millions d'euros par rapport à 2022, il a pour ambition une sincérisation des crédits crédits sincérisation, elle va dans le bon sens, elle constitue une première étape et il a semblé à la commission des finances que les résultats de l'exécution 2023, nous donnerons des éléments en vue d'adapter ultérieurement le dispositif, mais en l'état, c'est une demande de retrait sinon défavorable. Madame la Ministre. Madame la présidente, merci madame la sénatrice de la Provoté, c'est que c'est vraiment un des sujets qui a fait partie des des plus fort moment de la négociation budgétaire de. Cet été, et des priorités que j'ai voulu porter, j'en avais aussi parlé plusieurs fois avec François Sauvadet, le président de l'association des départements de France, je sais que de nombreux élus sont soucieux de cet enjeu de l'archéologie préventive, au terme de toutes ces discussions, j'ai obtenu tout de même une hausse de 20 % des crédits par rapport à l'an dernier, je trouve que c'est un un une évolution assez significative, nous pourrons en faire le bilan à l'issue des des prochains mois pour voir comment faire évoluer aussi ces ces arguments budgétaires pour l'avenir, merci à vous demande de retrait également. la situation d'un certain nombre soit de collectivité soit d'entreprises, soit de particuliers qui ont des terrains sur lesquels il y a des vestiges qui sont découverts et la charge de la fouille, une fois que être identifié la potence potentielle présence de de vestiges et particulièrement lourde et il conviendrait que des dispositifs d'accompagnement puisse être mise en oeuvre, parce que, aujourd'hui, alors que le coût de logements par exemple très élevé, hé bien tout cela aboutit à un renchérissement du coût des opérations et ceci est particulièrement préjudiciable à l'accès au logement de tous

avec un engagement auprès de la protection du parc Patrimoine archéologique certains et donc à ce à ce titre-là, elles doivent être considérés comme étant partie pleine et entière de cette politique, je vous remercie. Merci, nous passons 396 Monsieur Madame Monnier. Merci madame la présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, donc sur les exercices précédents, les crédits du plan de relance en constituer une garantie non négligeable pour les acteurs du Patrimoine mais ils ont aussi engendré une augmentation d'activité en manière en matière d'aménagement et de construction, qui devrait se poursuivre en vingt-trois, cette situation a des conséquences directes en matière d'archéologie préventive avec un surcroît d'activité, dont on se réjouit, mais que l'Inrap et les services agréés des collectivités territoriales doivent pouvoir assumer en matière de diagnostic, il apparaît notamment que les aménageurs, publics ou privés sont aujourd'hui satisfaits des délais d'exécution des opérations de diagnostic, ce qui n'a pas toujours été le cas aussi dans le souci de préserver des relations apaisées avec des aménageurs cet amendement propose d'octroyer 5 millions d'euros supplémentaires à l'Inrap afin de permettre à l'institut d'assumer les demandes opérations actuelles est prévue pour 2023 lié à la recrue 10 recrudescence des prescriptions, à la suite de la crise sanitaire, donc on propose d'abonder 5 millions dans l'action neuf programme 175 patrimoines et de minorer, du même montant, l'action cette fonction et soutien au ministère du programme 224. Monsieur Ouzoulias pour l'identique. Merci madame la présidente, madame la miss, mais mes chers collègues, j'ai eu à pratiquer, c'est un souvenir d'ancien combattant, la loi de 1941 sur l'archéologie et je me souviens avec quelles difficultés y compris dans cet hémicycle, la nouvelle loi sur l'arc, le préventive a été votée, présenté je suis très heureux de voir que, aujourd'hui, les élus la défendent et et souhaite même que l'Inrap participent davantage à cette mission de service public,

à l'encontre du du Patrimoine et je je reprends les mots très justes de mon collègue Max Brisson à propos des des énergies renouvelables, là en l'occurrence ce qu'on ce qu'on aimerait, c'est que les aides de l'Inrap pour réaliser le diagnostic soit beaucoup plus dynamique qu'elle puisse s'adapter, presque en deux de façon continue au à l'énorme cahier des charges auxquelles l'Inrap et et les services des collectivités parce qu'ils sont complémentaires et très souvent dans les départements, ils ont passé des conventions pour travailler ensemble, donc j'ai compris aujourd'hui que Bercy, vous demandez à un bilan, ce qui serait intéressant, c'est que dans une future loi de, de, de finances rectificative on puisse ajuster cette subvention à l'Inrap pour lui permettre de réaliser les les diagnostics et afin de ne pas ralentir les travaux, je pense que c'est tout à fait essentiel pour continuer à faire que l'archéologie préventive au jour aujourd'hui soit politiquement acceptable merci d'un président. ainsi que sur l'amendement précédent de notre collègue de la Provoté, nous avons une évolution des crédits prévus dans le projet de loi de finances sur ces questions, mais là il s'agit de financer l'Inrap, il est indiqué que les 4 8 millions d'euros supplémentaires sur l'exercice 2023 couvre pour deux millions six l'inflation et pour 2 millions de la progression des salaires des agents, donc ces nouveaux crédits ne couvre pas l'augmentation du nombre de diagnostics réalisés et donc la charge pour l'opérateur, qui était déjà en évolution importante puisqu'on en avait 1842 en 2020 et 2019 en 2021, nous souhaiterions donc savoir comment le ministère envisage avec l'opérateur, cette augmentation du nombre de ses interventions de nouvelles règles sont-elles envisagées pour alléger cette charge, nous avons dans notre rapport de contrôle sur le financement de la recherche patrimonial avec Didier Rambaud publié en février dernier, insisté sur la nécessité de renforcer, par exemple, les Liens entre le Drassm et l'Inrap au sujet des diagnostics archéologiques subaquatiques nous appelions notamment à la systématisation de conventions d'évaluation archéologique tarifée entre les opérateurs et le Drassm pour éviter le risque d'intervention à perte pour l'Inrap, qu'en est-il, et donc notre avis et l'avis de la commission des finances sur ce sujet : être un appel à la vie du gouvernement. Madame la Ministre. Merci madame la présidente, vous êtes, je suis ravi de voir autant de spécialistes de l'archéologie au Sénat c'est réjouissant, été samedi à Villers-Cotterêts. Après j'ai changé d'ailleurs avec les agents de l'Inrap qui m'ont montré les résultats de leurs fouilles et c'est impressionnant, nous aurons là de magnifiques découvertes qui vont enrichir notre découverte de l'histoire là effectivement nous avons un relèvement de 5 % qui permet de d'absorber le contexte de hausse des prix à hauteur de 2,6 millions et d'accompagner la réforme de la revalorisation salariale des agents à hauteur de 2,2 millions comme vous venez de le dire, mais cette mesure vient en complément des hausses intervenues en 2021 et 2022 5 millions en 2021 1 virgule 5 millions en 2022, et surtout des crédits importants du plan de relance, qui était de 34,5 millions déjà avant le plan de relance en 2020 et 20 millions dans le plan de relance, moi je serai vigilante en gestion, parce que là je j'ai pas pu obtenir plus que tout ce que j'avais déjà obtenu sur l'archéologie et qui me semblait suffisamment satisfaisant mais en gestion au ministère, on a bien nous la visibilité des chantiers de ceux qui progressent on je je serais vraiment très attentive à à rééquilibrer, chaque fois que possible, donc c'est une demande de retrait pour le gouvernement. L'avis de la commission après avoir entendu la ministre. On va rester sur un avis de sagesse, madame la présidente, chacun appréciera en fonction des éléments de réponse, on a compris que Madame la ministre avait négocié son budget, elle a pas obtenu satisfaction en tous points, peut-être pouvons-nous l'aider. Très bien, je vais mettre aux voix cet amendement qui a reçu un avis de sagesse de la commission, un avis défavorable du gouvernement qui est pour. Qui est contre qui s'abstient, il est adopté madame Paoli-Gagin pour le le 691. Oui merci madame la présidente, il s'agit d'un amendement qui vise à augmenter les crédits prévus par la mission pour la reconversion de du site de l'abbaye de Clairvaux, je vous rappelle, mes chers collègues, c'est une abbaye qui a été fondée en 115 par Bernard de Clervaux, c'est un site patrimonial, culturel, historique hors du commun, en effet, cette abbaye cistercienne s'est développée pendant près de 8 siècle jusqu'à devenir bien national en 1792 après la révolution, à l'initiative de Napoléon, elle est reconverti au début du XIXe en prison, devenant de ce fait, un au lieu de l'histoire carcérale de notre pays, elle a notamment accueilli Claude Gueux, dont Victor Hugo s'est inspiré pour l'un de ses romans, désormais, l'État engagé la fermeture de la prison et lancé un appel à manifestation d'intérêt comme je le disais tout à l'heure, les premiers résultats ont été annoncés le 12 novembre dernier plusieurs dossiers de candidature sont en lice, partageant tous l'ambition de faire de Clairvaux, un lieu de culture au rayonnement international comme il le fut autant des cisterciens et de redynamisation pour le tissu économique local en exploitant au mieux toute la richesse patrimoniale du site cette reconversion implique ainsi une mobilisation massive de capitaux privés afin d'engager d'importants travaux de restauration et le lancement de nouvelles activités en lien avec le projet qui sera finalement retenu ce flux financiers s'articulera avec les crédits inscrits par la mission culture à hauteur de 15 millions d'euros en autorisations d'engagement et de millions en crédits de paiement prévus par l'action 0 0 monuments historiques et Patrimoine monumental du programme patrimoines le rapport des rapporteurs spéciaux pour la commission des finances, indique que le montant des autorisations d'engagement prévus ne représente au mieux que 10 % du coût total du chantier qui est estimé, je vous le rappelle, entre 150 et 200 millions d'euros. Afin d'augmenter les moyens consacrés par l'État dès 2023 à la reconversion du site, notre amendement prévoit de tenir le même pourcentage de 10 % en l'appliquant à la borne supérieure de la fourchette estimée des travaux en outre afin d'assurer un décaissement rapide de ces crédits et de ne pas provoquer de retard dans le lancement du projet de reconversion, il est prévu de mettre en correspondance le montant des crédits de paiement avec celui des autorisations d'engagement.

pour un projet d'une ampleur considérable, parce que ce monument pour ceux qui le connaissent et est un monument extrêmement important en volume et en qualité patrimoniale néanmoins le les premiers résultats de l'appel à manifestation d'intérêt ont été rendus publics il y a 2 semaines, il va y avoir de nombreux mois d'ajustement évidemment du projet de négociations, de façon à pouvoir définir un montant d'autorisations d'engagement définitif, donc en l'état de l'avancement du dossier 15 millions ne nous paraissent ne nous paraissent pas impossibles à à entendre, et donc c'est un avis de demandes de retrait. Madame la Ministre. Merci madame la présidente, je suis d'accord en tout point à ce que vient de dire monsieur le rapporteur, c'est vraiment un des chantiers qui nous tient le plus à coeur, d'ailleurs je l'avais mis en avant dans mes exemples lors de ma conférence de presse budgétaire tout de même, c'est encourageant, on a 9 candidats qui se sont présentés 9 groupement privé, attendons de voir 3 d'entre eux ont été sélectionnés dans la première short list. Le l'ampleur des travaux, les projets, entrons dans le détail, c'est le budget 2023 on aura aussi les Budgets 2024 et au-delà pour accompagner ce chantier bien sûr donc demande de retrait. Merci madame la présidente, où des résistants, nombreux ont été incarcérés et ont été fusillés et je pense que, aujourd'hui, alors que nous vivons partout une montée des périls, c'est très important de rappeler cette mémoire et vous me permettrez un un commentaire très personnel, c'est là où mon arrière grand-père Maurice Rome Aegon a été fusillé le 7 mars 1942 merci madame président. Merci, je vais donc mettre aux voix cet amendement qui a reçu un double avis défavorable qui est pour.

Qui est contre. il n'est pas adopté

préoccupante des architectes des Bâtiments de France, face aux difficultés pour les collectivités territoriales à assurer l'entretien et la valorisation du Patrimoine local, les effectifs des DAP s'avère insuffisant et ne sont plus en mesure de répondre aux demandes des collectivités, le nombre d'architectes des Bâtiments de France semble décliner progressivement, comme d'ailleurs l'attractivité de cette carrière les places au concours n'arrive plus à être il intégralement pourvus, ce manque d'attractivité réside sans doute dans une rémunération un peu faible des ABF dépendant du ministère de la culture, mais certainement davantage dans les conditions d'exercice est difficile, compte tenu de leur petit nombre et du nombre très élevé d'avis annuel à donner ses moyens humains insuffisants provoque un allongement des délais d'instruction d'instruction des dossiers, il y a un ralentissement des chantiers, mettant ainsi en péril la protection des sites dans les ABF sont les garants, au regard des besoins d'expertise pas tribunal croissant dans les territoires, le recrutement d'un architecte bâtiments de France supplémentaires par département qui doit constituer un objectif à moyen terme, permettrait de renforcer le contrôle scientifique et technique de l'État sur ses projets de restauration et de conservation patrimoniale et d'offrir une assistance à maîtrise d'ouvrage minimale aux porteurs de projet, cet amendement, c'est 3 millions d'euros supplémentaires à l'action, monuments historiques, j'ai conscience qu'il faudra aussi envisager de travailler à une meilleure attractivité du métier, mais comme je viens de le dire, ça serait déjà, elle serait déjà sensiblement améliorée si la charge de travail des ABF étaient moins lourdes. Quel est l'avis de la commission sur cet amendement. nous avions ciblé, d'ailleurs, en 2018, à l'occasion d'une mission de contrôle, le manque de moyens pour les déplacements des agents ou encore la la faible attractivité financière des métiers, une partie du de ce sujet a été résolue par le plan de rattrapage indemnitaire pour autant celui-ci ne résout pas toutes les difficultés, notant cependant que le gouvernement a entendu cet intérêt en acceptant une une majoration des crédits affectés aux Drac à hauteur de 1 1000000 d'euros, en reprenant un amendement qui avait été qui été déposée à la à l'Assemblée nationale dans le texte transmis dans ces conditions, il est peut être envisagé d'attendre les les premiers résultats de l'exécution 2023 pour envisager une nouvelle majoration de crédits aussi, c'est une demande de retrait. Merci madame la présidente, en effet, juste en complément. Préciser que l'effectif, que ce soit pour les architectes des Bâtiments de France, où les ingénieurs ou les techniciens n'a pas diminué ces dernières années, au contraire, le ministère de la Culture s'est attachée à reconstituer cet effectif dans les départements où il y avait eu des baisses et en réalité aujourd'hui notre enjeu est pas tellement un enjeu de de nombre de mais c'est plutôt qu'on fait face à des vacances de postes à un baisse du nombre de candidats quand ton lancent des concours et donc on a un enjeu de travailler sur l'attractivité du métier des architectes des Bâtiments de France, ce dont on a discuté lors d'un séminaire où je les ai tous réunis, il y a quelques jours, travailler avec l'Ordre des architectes, bref on a avancé plusieurs pistes pour améliorer l'attractivité de ce métier, donc pour moi c'est une demande de retrait parce que l'amendement ne répond pas pleinement à la difficulté qui est celle de l'attractivité aujourd'hui mais je profite d'être au micro pour remercier tous les sénateurs, sur ces bancs et ceux qui ne sont pas là mais qui s'était mobilisés récemment dans les débats pour défendent le rôle des ABF, je sais que vous connaissez très bien la, l'importance de leur mission et pour défendre leur avis conforme pour continuer à concilier le développement des énergies renouvelables et la préservation du Patrimoine, merci à vous tous pour cet engageant. Madame Meunier il est maintenu, donc jamais aux voit double avis des femmes Madame Robert. Oui je je voudrais vraiment souligner cet amendement, même s'il ne répond pas complètement à la situation, je voudrais vous dire et on le sait, que la question de l'ingénierie dans les Drac est un vrai sujet pour les collectivités territoriales, la question des ABF, on l'a vu dans le projet de loi sur les énergies renouvelables est venu, c'est vraiment ce serait un signal très important que de voter cet amendement. Ce que je pense que c'est un sujet qui reviendra et qu'il faut vraiment conforté les Drac sur le sujet, merci beaucoup. pour ne pas rajouter je voudrais ça pour dire que je soutiens que j'appuie ce que vient de dire si les Robert. Merci donc je mettre aux voix cet amendement qui a reçu un double avis défavorable qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient, il est adopté, le 356 madame Robert. au niveau de la commission culture, il vise à permettre aux écoles territoriale d'appliquer aux étudiants boursiers, le même niveau d'exonérations que dans les écoles nationales en compensant pour elle, les effets de cette mesure, à hauteur de 2 5 millions d'euros, alors que les écoles nationales et les écoles territoriale délivrent les mêmes diplômes leur étudiants n'ont pas les mêmes droits, aujourd'hui, la revalorisation des bourses sur critères sociaux destinés aux étudiants des écoles nationales en 2023 risque encore de creuser l'écart entre les écoles nationales et les écoles territoriale et d'accroître ainsi les inégalités de traitement entre les étudiants, la diversité sociale et culturelle étant une politique portée par l'État et non par les collectivités territoriales, il m'apparaît logique de prévoir ce transfert de crédits.

je rappelle plus 7,5 millions d'euros, il convient simplement de rappeler à ce stade que les des aides, hein, dit individuels pour le soutien aux pratiques artistiques des élèves de l'enseignement initial dans les domaines du spectacle vivant sont déjà versés aux élèves des conservatoires à rayonnement départemental et régional, dès lors qu'ils sont adossés à à des pôles d'enseignement supérieur du du spectacle vivant une dotation de 1 virgule 6 millions d'euros, est prévue dans le présent PLF la majoration des crédits dédiés de 2 5 millions d'euros prévus dans le présent amendement viendrait donc plus que doublé cette enveloppe nous avions avec Vincent Eblé dans dans notre rapport de contrôle sur l'enseignement supérieur du spectacle vivant, rendu public en février dernier, appelé à une clarification des modalités de financement des des écoles territoriale la règle en la matière peuvent en première, analyste à paraître obscur et jugé et sont jugés inégale selon les les Drac, l'octroi de nouveaux crédits devraient donc être précédée d'une mise à plat du financement de l'État dans le prolongement d'ailleurs de la réforme des conservatoires qui semble peiner à se déployer, compte tenu du contexte inflationniste comme du risque de décalage entre les établissements nationaux et et et les écoles territoriale une majoration immédiate peut être jugée opportune aussi c'est un avis favorable. Merci que de l'avis du gouvernement. Merci madame la présidente. de la situation des des établissements d'enseignement supérieur artistique avec une priorité pour les écoles d'architecture en particulier et, globalement, on n'a pas du tout oublié, les écoles d'art territoriale avec 10 millions d'euros en investissement 21 millions en fonctionnement, c'est ça en fait qui nous a été remonté des besoins d'investissements de mise aux normes des besoins de repassage en fonctionnement avec aussi bas, la relation que que vous connaissez, je vous assure que de tous les échanges ai pu avoir avec l'Association des régions, l'AMF là ce sont des départements même la FNPC, ça ne faisait pas partie des priorités qui qui m'ont été soulevées ni cet été ni cet Automne, à ce stade nous et rappelons quand même que les taux d'inscription sont très bas, hein, dans ces écoles, on est en France parmi les plus bas d'Europe par rapport à d'autres pays, donc pour moi, la priorité n'était pas là j'avoue la priorité était sur l'accompagnement d'investissement, l'accompagnement fonctionnement et on a mis les les Budgets, donc pour moi c'est un avis défavorable. Bien. Je vais donc mettre aux voix cet amendement qui a reçu un avis favorable de la commission est défavorable du gouvernement qui est pour. Le droit. Qui est contre, il est adopté, Madame Robert, le 357. Oui, donc je vais parler des écoles d'architecture, puisque là aussi au nom de la commission de la culture, cet amendement donc vise à revaloriser de 2 2 millions d'euros, le montant des crédits destinés à compenser la hausse des salaires, des entrées saignant contractuels contractuels des ça, en effet, le coût de cette mesure a été évaluée à 4 millions d'euros tous cas c'est ce qu'on nous a dit, dans l'audition et le projet de loi de finances ne comporte qu'un virgule 8 millions d'euros, à ce titre, cette mesure apparaît donc indispensable pour permettre aux INSA qui, c'est vrai, dont le budget a augmenté, vous l'avez dit, et je d'ailleurs, je l'ai dit dans ma DG de retrouver des marges de manoeuvres financières leur permettant de maintenir un enseignement de qualité, car derrière il y a aussi d'autres questions qui viennent impacter leur budget, je vous remercie, quel est l'avis de la commission des finances. Oui, sur ce sujet ne semble pas qu'il y a de désaccords de fond tout le monde convient qu'une revalorisation de la rémunération des enseignants chercheurs dans les écoles d'architecture et nécessaire, mais le processus est engagé dans le présent projet de loi de finance à hauteur d'un 1000000 650 millions d'euros, 650000 euros et donc la commission a considéré considéré que c'était une première étape et qu'il convenait de demander le retrait. Quel est l'avis du gouvernement. Je mais aux voix qui est pour.

Qui est contre. Il est adopté, j'attire votre attention sur le fait qu'il nous reste 15 traitement quinze minutes et 6 amendements à examiner chacun prend les deux minutes ça passe pas, donc tout le monde a compris le message, j'imagine.

la plupart du temps elles sont soumises à des modalités d'application variable 2 jours d'horaires et d'offres artistique notre amendement vise à généraliser cette gratuité, nous sommes conscients qu'elle n'est pas la réponse unique à l'enjeu de démocratisation elle permet cependant de lever le 1er frein, je me permets de souligner que le Val-de-Marne avait mené une étude sur la non-fréquentation sur les gens qui ne fréquentait pas le Mac/Val et que les 2 réponses qui venaient la première était, ça n'est pas pour moi et la deuxième était le coût est trop élevé, élevé, malgré un tarif très peu dissuasif, donc, nous vous demandons d'investir en direction de la jeunesse, évidemment, nous souhaitons que le gage soit levé. Quel est l'avis de la commission. Alors effectivement, on considère que ça va être un amendement d'appel qui est incontestablement séduisant, je me permets de vous rappeler que le Pass culture tente d'y répondre partiellement en intégrant les musées dans son offre dédiée en partie au 18 20 ans ils sont comme néanmoins difficile pour l'État de d'imposer à la totalité des musées notamment privé cette gratuité, fût-elle compensée, donc c'est un avis de retrait. Qu'est l'avis du gouvernement. Même avis d'autant plus que le Mac/Val exemple que vous avez cités et sur le Pass culture et en en bénéficient. Si tous les musées. Ne sont déjà gratuit pour les moins de 25 voire 26 ans, on ne peut pas imposer aux musées territoriaux leur politique tarifaire libre administration des collectivités territoriales en revanche par le Pass culture collectif les sorties au musée se développe par le Pass culture individuelle également et par nos aides via les Drac, un ensemble de programmes comme l'été culturel qui permet aussi l'été, de permettre à des des populations, notamment jeunes, qui ne peuvent pas partir en vacances, d'aller aussi au musée : demande de retrait. moi je mets aux voix cet amendement double avis défavorable qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient n'est pas adopté de 524 monsieur dessus. Merci madame la présidente, donc les associations de réduction des risques sont présentes dans de nombreux festivals ou concerts au concert, pardon, pour 100 le civiliser le public aux risques liés aux usages de drogue leur action permet de réduire le nombre d'overdoses identifiées de sensibiliser les usagers sur les produits les plus dangereux, or cette présence essentielle est loin d'être garanti pour tous les événements à travers cet amendement, nous, nous souhaitons pousser vers la généralisation de la présence de de ces s'association en milieu festif, bien souvent, ce sont les collectivités seuls qui accordent leurs subventions à ces associations, il est temps que l'État s'cage davantage. C'est que, de l'avis de la commission. bien sûr, on peut pas être compte l'objectif mais ce n'est pas le lieu, nous pensons qu'un dispositif créé au sein de la mission Culture contribuerait un essaimage regrettable des moyens budgétaires dédiés à la lutte contre ses addictions et donc c'est une demande de retrait sinon défavorable. Madame la Ministre me ma vie. Même avis : je m'engage à en parler avec mon collègue François Braun, parce que ça relève davantage de la santé, je connais bien l'association. Nos Paul qui notamment a agi de manière très forte sur ces sujets, j'en profite ce que je n'avais pas eu le temps d'en d'en parler tout à l'heure, pardon, madame la présidente, je prends une minute pour vous remercier vous remercier de votre attention sur le sujet des festivals au moment des Jeux olympiques de 2024 nous sommes en plein dans un travail très méthodique, région par région, phase par phase au cas par cas pour permettre à ces festivals de se décaler de quelques jours de revoir leur format, si besoin est de pouvoir se tenir, en fait, seuls sont concernés les festivals, mobilisant des unités de forces mobiles des recours nationaux en unités de forces mobiles, donc déjà on ne parle pas de tous les festivals de France je vous rassurer là-dessus ce pointage a été fait de manière très précise et nous sommes en plein dialogue avec le ministre de l'Intérieur, la ministre des Sports et les préfets concernés et ce ce dialogue et très constructif à ce stade, je voulais vous rassurer là-dessus. Merci, jamais au vote cet amendement double avis défavorable qui est pour, qui est contre qui s'abstient, il n'est pas adopté monsieur Fiole le 657. Oui, je vais vous résumer cet amendement de notre collègue Guilaine Pentel qui vise à soutenir les collectivités territoriales pour l'entretien et la valorisation du Patrimoine local, on sait combien ce Patrimoine du pigeonnier au lavoir en passant par la demeure de maître et le musée ou le musée de proximité signe l'identité de nos villes et visages je vous épargne tous les arguments pour vous dire que sans méconnaître les moyens Philippe qui accompagnent les communes à faibles ressources, nous souhaitons par cet amendement soutenir davantage les collectivités territoriales pour l'entretien et la valorisation du Patrimoine local qui a fait toute la richesse de la France. C'est une demande de retrait en raison de l'existence dans le projet de loi de finances de crédit d'un fonds incitatif et partenariale qui est déjà majoré donc la commission des finances, a estimé que cette demande était déjà satisfaite.

Madame la présidente, cet amendement propose en complément du FIP visant à aider les collectivités à faibles ressources, à financer les travaux d'entretien, de restauration et de mise en valeur des monuments historiques, de créer un fonds d'expérimentation permettant aux Drac de proposer une assistance à maîtrise d'ouvrage à titre gracieux, en direction de ces mêmes collectivités le récent rapport de la Cour des comptes sur la politique de l'État en faveur du Patrimoine monumental établi en effet que cette disposition prévue dans le code du Patrimoine depuis que la maîtrise d'ouvrage des travaux sur les monuments a été rendu au propriétaire, a été très très peu suivi d'effet, en effet, il existe dans de nombreuses collectivités un besoin d'accompagnement technique des porteurs de projets publics dans la non satisfaction contribue à entretenir la sous-consommation des crédits consacrés aux monuments historiques, ce point est corroborée par le dispositif mis en place depuis plus d'une dizaine d'années par la Drac de Bretagne. Qu'est l'avis de la commission. C'est maintenant le président c'est une demande de retrait parce qu'une majoration de la dotation des Drag de un 1000000 d'euros, présenté par amendement à l'Assemblée nationale, a été retenu par le gouvernement dans le texte transmis donc demande de retrait. Madame la ministre, même ma vie ma ma vie. Jamais aux voix qui est pour, qui est contre. Qui s'abstient, il n'est pas adopté, nous allons procéder au vote des crédits de la mission Culture figurant à l'état B, je me vois des crédits de la mission, je vous rappelle que la vie de la commission des finances, est favorable à l'adoption de ces crédits pour. Qui est contre

si pertinent que soient s'angle les pistes d'amélioration du dispositif doivent également concerner l'accès des jeunes ayant quitté les structures scolaires, quelle que soit la zone géographique où ils évoluent les projets et rapports annuels de performances des documents déjà précisément l'évolution du dispositif, le rapport annuel d'activité de la SAS de la SAS Pass culture détaille également les modalités de recours à l'application, en ciblant notamment les actions en direction des publics les plus éloignés, dans ces conditions, il est proposé de supprimer cet article. sagesse je mets aux voix l'amendement de huit qui est pour. Qui est contre qui s'abstient, il est adopté, et l'article et donc supprimer Sans remettre en question la pertinence du sujet de l'accès aux infrastructures culturelles, il est possible, s'interroger sur la nécessité d'inscrire en loi de finances la remise d'un rapport, la commission des finances est traditionnellement assez réservé aux nombreux rapports qui sont sollicités à l'occasion de l'examen de la loi de finances. En l'occurrence celui-ci ne concerne qu'une partie des territoires ultramarins ne vise in fine et que l'action de la seule direction des affaires culturelles de Guadeloupe, puisque les îles, Saint-Martin et Saint-Barthélemy relève du ressort de celle-ci, dans ces conditions, il est proposé de supprimer cet article. La ministre Je mais aux voit cet amendement reçu un avis de sagesse du gouvernement qui est pour. Qui est contre qui s'abstient, il est adopté, et donc l'article est supprimé, nous passons maintenant aux crédits de la mission Médias livre et industries culturelles du compte spécial avances à l'audiovisuel public et du projet loi de finances, considéré comme adopté à l'Assemblée et la parole est au rapporteur spécial de la commission des finances monsieur Karoutchi.

Madame la ministre, madame la présidente, je ne sais pas si c'est utile de faire le tour complet des éléments de de crédits de cette mission, je vais plutôt tout à l'heure, répondre aux amendements, je voudrais juste vous dire que nous avons à la fois un 1er secteur livre et industries culturelles. Qui est un secteur qui a des problèmes à des difficultés liées d'ailleurs essentiellement à la non reprise de la fréquentation des salles malgré une atténuation du Covid que ce soit les cinémas, que ce soit les festivals, que ce soit les théâtres, que ce soit les bibliothèques, la fréquentation n'est plus n'est pas redevenue celle d'avant 2020, donc là nous avons un problème, je le dis tout de suite puisqu'il va y avoir une série d'amendements, nous avons reçu notamment les responsables du CNC, les responsables du CNM, les responsables de la Bibliothèque nationale de France. Chacun a naturellement des difficultés, mais sur le CNC globalement avec des des méthodes diverses globalement le le financement reste conséquent, se pose la question de savoir si le CNC, à raison de financer un certain nombre de films ou de séries que l'on a retrouvé sur Netflix, ça c'est un autre sujet, mais bon le le CNC dispose quand même de moyens conséquents, même si la baisse de fréquentation des salles reste de l'ordre de 20 par rapport à ce qu'elle était en 2019. Le problème du du du CNM est plus compliqué le CNM n'a pas pour le moment trouver réellement sa place ou plus exactement il a pas trouvé, Madame la Ministre, les financements nécessaires, alors pour l'année prochaine je je on a à peu près trouvé ou en tout cas par redéploiement, les financements, mais c'est vrai qu'il faut réfléchir tout de suite à d'autres sources de financement à une autre organisation pour que le CNM ne se retrouvent pas dans une très grave difficulté en 2024 là-dessus il y a un certain nombre de propositions qui ont été faites, nous attendons de votre part de nous dire quelles sont les pistes qui peuvent effectivement renforcer stabiliser le monde de la musique, la BNF c'est un un problème permanent, madame la ministre, pour le moment, alors j'ai bien vu un amendement tout à l'heure mais je je donnerai un avis négatif mais si, mais un Hannover négatif parce que j'allais presque dire il faut ou beaucoup plus où reposer le problème : la BNF a des problèmes d'investissement, d'abord parce que le bâtiment, c'est comme ça commence à vieillir et baffe, vous avez dit mille fenêtre à refaire 16000 euros la fenêtre 160 millions. si vous avez 100 magasin on les attend, mais jusqu'ici, j'ai pas vu, donc c'est clair que, on a un problème, c'est le paquebot de la lecture en France mais un paquebot tellement lourd que je ne sais pas jusqu'où il va falloir aller au niveau des investissements pour maintenir la qualité de service, l'étendue, la BNF et puis soyons francs : au début, lorsqu'on a construit la BNF, tout le monde pensait qu'on allait tellement vers le numérique qu'on allait plus de voir tellement stocker du papier, et c'est comme ça, il continue à y avoir un dépôt de documents de livres extrêmement important : le résultat des courses. C'est que bah on a créé un nouveau centre de documentation à l'extérieur et puis on se dit déjà qu'à l'heure qu'il est même pas construit et même pas livré, il sera probablement probablement insuffisant d'ici 4 5 ans et qu'il faudra peut-être envisager encore un autre, et on se dit bon bah voilà il faut clairement recalibrer le budget lecture dans ce pays, d'autant que, soyons francs, la BNF absorbe tellement de crédit que pardon pour tous les élus de province, il reste pas grand chose pour les bibliothèques de province parce que la BNF est quand même un gouffre bon alors un gouffre utile mais c'est un gouffre donc les bibliothèques de province ont ont du mal L à survivre devant, devant un tel paquebots, enfin, Madame la Ministre, dans les 2 minutes et quel qu'il me reste l'audiovisuel public, alors là, pour ne rien vous cacher, je vous l'avez dit, d'ailleurs, on s'est retrouvé devant la promesse du candidat président ou du président-candidat, de supprimer la contribution de l'audiovisuel public, la présentant sous forme de de finalement de gain pour les citoyens ont pouvoir d'achat, sauf que imprévision doute enfin en réalité rien n'avait été prévu, en contrepartie, et donc on s'est retrouvé avec mon excellent collègue Jean-Raymond Hugonet à faire un rapport pour essayer de trouver des pistes. Sauf que ces pistes certes sont intéressantes mais elles ne sont fondées, madame la ministre que s'il y a une réforme de l'audiovisuel, cette fameuse réforme dont on parle sans arrêt depuis 2017, mais dont nous n'avons pas le commencement de réalisation, on avait bien eu un texte qui est allé à l'Assemblée nationale qui n'est jamais arrivé ici, qui a été visiblement en grande partie abandonné, même si vous en reprenez certains éléments et dans la pratique, on se retrouve avec un élément qui pour moi est franchement une aberration, on ne se remet pas en cause sur le contour, le périmètre du service public sur les missions du service public et on ne parle que d'argent. Combien ben c'est simple : on prend le budget de l'année d'avant on rajoute 2 ou 3 % et puis l'année d'après, on fait la même chose, puis la même chose que la même chose sans jamais redéfinir les missions du service public et ce qu'on attend du service public, il y a donc là un vrai sujet. Moi, j'ai donné en commission des finances, après beaucoup d'hésitations, un avis favorable au budget à 3 milliards 800 millions pour l'audiovisuel public pour ne pas entraver son fonctionnement mais madame la ministre est clairement c'est un avis favorable One shot, si je peux me permettre en anglais pour montrer ma maîtrise de quelques mots One shot, ça veut dire que si vous n'avez pas en 2023, des éléments de réforme permettant de faire progresser les choses, ce ne sera pas la vie pour 2024 ça n'est pas possible franchement et je conclus par là, madame la ministre, on attend beaucoup de votre part en matière d'audiovisuel public. L'avis de la commission d'affaires étrangères, et pour trois minutes. Merci madame la présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, l'audiovisuel extérieur est un puissant outil de rayonnement dans le contexte de tensions internationales fortes alors que les valeurs de la démocratie et de l'état de droit sont attaqués de toutes parts et je voudrais ici félicité et remercié les équipes de France Médias Monde et de TV5 Monde pour leur engagement sans faille et leur courage en soutien de nos valeurs cet audiovisuel répond aussi à une forte attente dans de nombreux pays où les audiences sont significatives, le projet de loi de finances prévoit une contribution de l'État à l'audiovisuel extérieur de 365 millions d'euros, dont 285 millions pour France Médias Monde en hausse de 3,5 pour 100 et 80 millions pour TV5 Monde en hausse de 4 % or compensation des effets de la réforme du financement de l'audiovisuel public, la contribution à l'audiovisuel public a en effet été remplacée par l'affectation au secteur audiovisuel d'une fraction du produit de la TVA, ce mode de financement, confirme que les médias français sont des médias de service public et non des médias d'État, c'est une distinction qui est crucial à l'international pour conforter l'indépendance de notre audiovisuel extérieur et donc en asseoir la crédibilité ce mode de financement n'est toutefois acté que jusqu'au 31 décembre 2024 or, Madame la Ministre votre ministère semblent considérer qu'une budgétisation du financement aurait peu d'impact, il nous semble au contraire qu'une budgétisation, serait très préjudiciable d'ores et déjà, les autorités compétentes du Land de Berlin ont fait savoir qu'une budgétisation du financement pourrait remettre en cause l'attribution et Rachid une fréquence FM, alors que nos chaînes subissent déjà des interdictions en Russie et au Mali une budgétisation risquerait donc d'entraîner des suspicions à l'origine d'un effet domino, c'est pourquoi aussi l'autonomie des chaînes de l'audiovisuel extérieur est essentiel : une fusion des différentes ceci audiovisuel public ferait passer l'actualité internationale au second plan, or la plus grande incertitude continue à prévaloir sur l'organisation de l'audiovisuel public extérieur dans l'attente, les contrats d'objectifs et de moyens sont reconduits sans vision claire de ce que sera l'avenir, la BBC, elle dispose d'une charte royale, approuvé par le Parlement depuis 2016 qui garantit son indépendance, la mise en place d'une charte de ce type serait un facteur de crédibilisation supplémentaire pour France Médias Monde en plus des considérations relatives au financement et à l'organisation des chaînes déjà mentionné sous réserve de ces remarque l'augmentation des crédits est un signe positif et donc notre commission Monsieur Guérini, rapporteur pour avis de la commission des Affaires étrangères pour trois minutes. minutes. La présidente, madame la ministre, mes chers collègues, ça été rappelé dans un contexte de concurrence internationale, les incertitudes pesant sur l'avenir de l'audiovisuel extérieur constitue un handicap, les moyens des opérateurs français stagne entre 2018 et 2022 les dotations de l'État aux entreprises de l'eau du oh visuel public extérieur ont subi des baisses de l'ordre d'un et demi pour sans que les recettes propres des chaînes hein diminution en raison de la crise sanitaire ne puisse les compenser, dans le même temps l'accroissement des tensions internationales, nos partenaires à renforcer les moyens consacrés à l'heure audiovisuel extérieur, c'est ainsi qu'en 2021, la chaîne allemande des doubles vies et la branche internationale de la BBC se sont vus allouer respectivement 396 et 355 millions d'euros, ces chiffres sont à confrontés aux 250 5 millions d'euros tout disposé France Médias Monde cette même année, TV5Monde répondant qui appelle à une logique différente de surcroît le secteur audiovisuel est tenu de s'adapter aux nouveaux usages, ce qu'il fait bien et avec le succès que nous lui connaissons France 24 est le 1er média français sur YouTube, tandis que la plateforme TV5Monde plus lancé en 2020 proposent des contenus visionnés dans plus de 200 pays et territoires et si la promotion de la francophonie de mer, la Pierre angulaire, le plurilinguisme reste un enjeu croissant. RFI a renforcé au Sahel son offre en langues africaines grâce à un financement de l'Agence française de développement, une étude montre que ces programmes sont très suivies au Sahel France Médias Monde a, par ailleurs, dans le contexte à la guerre en Ukraine renforcer son offre en Europe orientale, avec le soutien financier du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, c'est ainsi qu'une offre de RFI, 100 % numérique, un Ukrainien a une a été lancée en octobre 2022, nous appelons à la pérennité et stabilité des financements du ministère des Affaires étrangères et de l'Agence française de développement, ce budget de l'audiovisuel extérieur est plutôt favorable, même si l'inflation en relativise la portée : il nous faudra rester attentif aux évolutions des conditions international particulièrement troublé. Merci. Monsieur le rapporteur pour avis de la commission de la culture, de l'éducation, de la communication. Madame la présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, la presse n'allait déjà pas très bien ces dernières années, elle a ainsi vu ses recettes divisées par 8 depuis 2000 car dépouillé de ses ressources publicitaires par les plateformes et victime collatérale d'une information désormais disponible gratuitement et où chacun est devenu expert en tout, ce constat, nous le partageons nous les payons depuis des années et je sais l'attention que vous apportez, Madame la Ministre à cette question si essentielle à notre démocratie, pourtant les éditeurs, les journalistes ne sont pas restés immobiles, certains titres ont su développer de nouveaux modèles économiques, d'autres ont bien d'avancer dans la transition numérique, j'ai ainsi réalisé ou non de la commission de la culture, un rapport au mois de juillet dernier sur la presse quotidienne régionale, qui souligne les difficultés, mais également les perspectives et les ambitions de cette presse qui va du village au monde crise mais adaptation avec le soutien jamais démenti des pouvoirs publics à travers par exemple le plan filière qui a enregistré des résultats remarquables pour les imprimeries, or les conséquences de l'inflation sont venus percuter de plein fouet, c'était des fils encore trop fragile, avec l'explosion des prix du papier, des titres juste à l'équilibre, plonge dans le rouge, les autres reporte des investissements pourtant nécessaires de cela, Madame la Ministre, vous êtes bien entendu nullement responsable cependant ce qui vous revient, c'est l'accompagnement, or si les crédits de cette année progresse essentiellement pour des raisons liées à la réforme du portage du du postage, presque rien n'est prévu pour compenser au moins partiellement, la hausse des coûts du papier je dis presque, car une disposition introduite dans le projet de loi de finances rectificative prévoit 5 millions d'euros pour la seule près ce que dit Anne nationales et régionales, l'ardoise se monte, on en est pleine à 175 millions d'euros, ce n'est ni sérieux ni adapté, il est important de souligner que la presse n'a touché qu'une infime fraction des 150 millions d'euros du crédit d'impôt pour le premier abonnement dispositif adopté pour soutenir en sortie de crise pandémique et qui a été, je dois le dire, torpillé par des lourdeurs administratives en voie d'être supprimés cette année sans grande considération d'ailleurs pour les quelques éditeurs, en particulier dans la presse en ligne et qui avait commencé je pouvais compléter cette somme par les 500 millions d'euros de l'amende infligée par l'Autorité de la concurrence en novembre dernier à Google pour non respect d'injonction dans le cadre de la rémunération des droits voisins, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la presse rapporte à l'État, mais on voit pas la couleur en cas de besoin donc 650 millions d'euros de disponible 10 % seulement de cette somme serait la hauteur des enjeux du moment il il resterait toujours 585 millions d'euros pour l'État, pour cette raison, Madame la Ministre, et à regret, je dois le dire, la commission a décidé de s'abstenir sur l'adoption des crédits du programme 180 Presse et médias et de s'en remettre, dans ces conditions à la sagesse du Sénat, je vous remercie. Rapporteur pour avis de la commission de la culture l'éducation et de la communication. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, la sinistrose ambiante semble avoir largement contaminées la presse des articles alarmistes, paru en octobre, ont ainsi fait état, je cite, de la panique qui se serait emparés du cinéma de son cri d'alarme, en un mot, les salles seraient aujourd'hui face à un destin funeste, sans grand espoir, il est vrai, comment le nier que les chiffres ne sont pas à la hauteur des espoirs de l'après-crise 50 millions de spectateurs en moins en 2020 et en 2021 par rapport à la seule année 2000 19 et une baisse de fréquentation de 30 % pour 2022 années qui n'aura donc pas permis le le retour à la normale, cependant il sans tomber dans l'angélisme, je crois, importante d'apporter quelques nuances ce constat, les chiffres sont bien meilleurs que la moyenne des années 90 qui s'établissait alors à 135 millions de spectateurs, ensuite, il faut bien mesurer l'impact différé de la crise sur les productions, si la France a maintenu au niveau de production grâce, il faut le reconnaître, au soutien massif des pouvoirs publics, comme je le souligner l'année dernière, telle n'a pas été le cas dans d'autres pays, notamment aux États-Unis où les tournages ont été littéralement stoppée pendant plus d'un an, or le cinéma américain est essentiel au cinéma français les gros films vont venir des spectateurs en salles qui en profitent pour découvrir les Oeuvres nationale mais ces films pas encore terminés ou à la sortie décalée ne sont tout simplement pas revenue en salles, les studios visant plutôt 2023, on doit donc alors se réjouir de l'immense succès de Top Gun Maverick 7 millions d'entrées, mais aussi de la production française ambitieux qui ont retrouvé leur public comme la nuit du 12 de Dominik Moll, il existe donc bien public prêt à aller dans les salles, ce constat est d'autant plus vrai pour le public jeune qui est le plus revenue au cinéma, il faudra certainement un travail spécifique pour les publics plus âgés, je souhaite, Madame la Ministre, que la campagne de commune communication lancée par le CNC porte ses fruits et que vous puissiez trouver en fait un moyen d'échapper aux sollicitations pressantes d'un illustres prédécesseurs au ministre de la culture. Au ministère de la culture, enfin je crois qu'il faut lever plusieurs malentendus qui trop complaisamment répandues finisse par détourner le public des salles non, le prix des billets n'est pas astronomiques, à quelques exceptions près, il est en moyenne de 7 euros et seuls 15 % des spectateurs paient plus de dix euros leur place, non les plateformes ne tue pas les salles, j'ai d'ailleurs pris connaissance à ce propos avec intérêt d'une étude de Médiamétrie qui monte, que les publics les plus jeunes, ceux précisément qui reviennent dans les salles désertes, les plateformes de streaming au profit des vidéos courtes sur Internet quel retournement de situation, vous l'aurez compris, même si les défis sont nombreux et requiert toute notre attention, je suis persuadé que nous devons pas les aborder avec pessimisme, bien au contraire, c'est dans cet état d'esprit que la commission a souhaité me confiait ainsi qu'à ma collègue, Céline Boulay-Espéronnier à ma collègue Sonia de la Provoté, une mission sur la filière cinématographique que nous abordons avec enthousiasme exigence pour proposer au Sénat une vision complète du secteur nous examinerons notamment, le dossier est toujours d'actualité, de la chronologie des médias dans la lignée des travaux de Catherine Morin-Desailly en 2017 ainsi que la sonde du CNC, la commission de la culture, a donc donné un avis favorable à l'adoption des crédits du cinéma pour 2023 je vous remercie pour votre. La parole est à. Jean-Raymond Hugonet. Rapporteur pour avis de la commission, hein, pardon monsieur j'ai oui, excusez-moi, la parole est à Julien Bargeton je je comprenais pas pourquoi vous étiez tranquillement assis à votre. Merci la présidence on se ressemble un peu, c'est pour ça, il y a quelque chose de réjouissant, a constaté que, après une période pandémique qui nous a tous marqués, les industries culturelles connaissent en 2022, une très belle progression et devrait rapidement dépasser leur niveau d'avant-crise, je dis bien réjouissant car, en dépit des problèmes et des difficultés à surmonter que je vais évoquer cela traduit de l'appétit et la curiosité de nos compatriotes pour la culture sous toutes ses formes, j'en veux ainsi pour preuve les chiffres remarquables de l'édition, supérieur de 15 % à 2000 19 et quel signal plus encourageant que le succès du Pass culture qui permet à la jeunesse, de découvrir de nouveaux univers, on a parfois critiqué ce dispositif sous prétexte qu'il ne servirait qu'à acheter des Mangas grand succès connaît un très grand succès, tant mieux, mais je n'ai pas assez relevé que 60 % des jeunes qui achètent un Manga avec le Pass repartent avec un autre livre, vous entrez pour One Peace et vous sortez avec Marcel Proust, tout n'est pourtant pas rose dans le secteur, les relations entre auteurs et éditeurs traverse une phase difficile, la signature d'un accord entre les 2 parties, prévu le 25 octobre dernier a été un peu la surprise générale, rejetée par les auteurs, qui souhaite ouvrir le dossier des rémunérations s'il n'appartient pas aux pouvoirs publics d'intervenir directement, ils doivent s'efforcer de jouer un rôle de médiation, et je crois, Madame la Ministre, que vous avez pris ce problème à bras le corps, que je connais votre attachement aux livres et à ceux qui le font, le Centre national de la musique doit trouver son rythme de croisière après la tempête du Covid quelle mission, quel financement quelle participation des uns et des autres à cette maison commune, patiemment, telle était l'objet de notre table ronde de la commission le 19 octobre le gouvernement m'a confié une mission sur le sujet, la gageure est élevé, je m'appuierai bien entendu sur les travaux déjà menés par le Sénat sur ce sujet du gouvernement, celle dont l'ambition du gouvernement qui a lancé le plan France 2030, au sein duquel un milliard d'euros sera consacré aux industries culturelles et créatives 1 milliard ce n'est pas rien, tous les amoureux de la culture, tous ceux qui ont conscience de son importance en termes économiques, en termes d'influence internationale ne peuvent que se réjouir des moyens supplémentaires qui vont structurer le paysage pour les années à venir, année 2022 oblige, je ne peux pas conclure sans un mot des conséquences du choc inflationniste ainsi pour prendre 2 exemples : la BNF consomme autant d'électricité qu'une ville de 20000 habitants avec son demi- 1000000 de mètres carrés de surface vitrée, c'est plus une montagne qu'un gouffre en la matière, concrètement, le surcoût estimé à 3,6 millions d'euros en 2023 ne doit pas obérer sa capacité à mener des projets il assurer l'entretien courant, autre acteur très concerné les libraires, le secteur dégage de très faibles marges et doit aussi su suivre la hausse des salaires, il ne faudrait pas que le renouveau du livre soit empêchée par la dynamique, les difficultés économiques de nos libraires, il faudra donc en 2023 faire coïncider les fortes ambitions du secteur avec les contraintes du moment sous le bénéfice de ces observations, la commission de la culture, a émis un avis favorable à l'adoption des crédits du programme livre et industries culturelles, je vous remercie. Rapporteur pour avis de la commission de la culture l'éducation et de la communication. Madame la présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, quelle est la situation de l'audiovisuel public le bilan du précédent quinquennat c'est limité pour l'essentiel à un travail d'assainissement budgétaire avec la mise en oeuvre d'une trajectoire budgétaire de moins 190 millions d'euros sur la période 2018, 2020 la perspective de la campagne présidentielle laissait espérer qu'un projet pour l'avenir de l'audiovisuel public pourrait émerger des débats pour redéfinir sa place dans un paysage largement bouleversé par l'arrivée des plateformes or non seulement aucun projet n'a émergé au cours des derniers mois mais rarement la situation du secteur aura paru aussi confuse pour au moins 4 raisons : première raison le gouvernement a indiqué que l'évolution du secteur n'était pas sa priorité, même s'il n'exclut pas totalement de rouvrir le chantier d'une réforme au printemps 2023 2ème raison l'élaboration de nouveaux contrats d'objectifs et de moyens, a été reporté d'une année, il faudra donc se contenter de simples avenants et attendre la fin 2023 pour connaître les objectifs et les moyens que l'actionnaire entend assigner aux entreprises de l'audiovisuel public pour la période 2024 2028 d'ici là, les entreprises concernées sont au choix dans l'attente ou dans la continuité 3ème raison: la suppression de la contribution à l'audiovisuel public, cet été, s'est accompagnée d'une solution de financement provisoire pour par une part de TVA, mais c'est l'inconnu qui domine concernant l'après 2024 ce qui crée un climat d'incertitude préjudiciable dans les entreprises concernées quatrièmes raisons enfin la fusion avortée entre TF1 et M6 fragilise aujourd'hui ces 2 groupes privés mais aussi France Télévision puisque la plateforme Salto apparaît aujourd'hui condamnés, du fait des difficultés des 3 actionnaires à poursuivre leur coopération. Par ailleurs, la fusion aurait eu un effet de rattrapage sur les prix de la publicité qui aurait également profité à France Télévision, le groupe public se trouve donc doublement pénalisés au final 2023 apparaît déjà comme une nouvelle année de transition, c'est pourquoi je souhaite rappeler les 2 propositions principales faites en juin dernier dans un rapport conjoint réalisé à l'initiative de nos commissions de la culture et des Finances consacrée au financement de l'audiovisuel public premièrement, apporter des garanties au financement des entreprises de l'audiovisuel public à travers la création d'une commission indépendante chargée d'évaluer les besoins pluriannuelle de l'audiovisuel public, deuxièmement fusionner les 4 entreprises nationales, France Télévisions, Radio France, l'INA et France Médias Monde pour assurer leur pérennité de et développer leur offre numérique, le projet de loi de finances pour 2023 prévoit une hausse des crédits de 3 pour 100 destinée à compenser l'accroissement des charges fiscales consécutifs à la suppression de la cape et à amortir la hausse de l'inflation la hausse des moyens et donc à relativiser : je souhaite maintenant que la nouvelle ressource soit définie dès 2023 afin de figurer dans les comme 2024 2000 28 et de mettre un terme à l'incertitude sur le financement, compte tenu des nombreuses interrogations qui entourent l'avenir de l'audiovisuel public, la commission de la culture, a décidé de s'abstenir sur l'adoption des crédits relatifs au compte de concours financiers avances à l'audiovisuel public, du projet de loi de finances pour 2023 et s'en remettra dans ces conditions à la sagesse du Sénat j'indique, pour ma part que je voterai ces crédits, merci de votre attention. avant de d'ouvrir la discussion générale, et donner la parole à notre collègue Bernard via l'air, je vous donne un peu de visibilité si chacun d'entre nous et vous et très raisonnable, nous pouvons finir l'examen de ce de cette mission avant la suspension de de la fin de l'après-midi, si vous n'êtes pas raisonnable, nous reviendrons tous a présidé la parole est à monsieur Bernard d'air pour cinq minutes pour le groupe RDSE. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues. La presse, la télévision, la radio, le livre, la musique, le cinéma sont traversés par la même difficulté : la révolution numérique, celle-ci a modifié en profondeur les usages de nos concitoyens et impacté le modèle économique de plusieurs grandes entités si l'on ajoute à cela la crise sanitaire, puis, aujourd'hui, l'inflation, c'est dans un contexte flottant où se mêlent enjeux structurels et conjoncturels que les pouvoirs publics doivent accompagner tous ces secteurs, non sans difficultés, la tâche est immense, l'absence, à court terme de réforme de l'audiovisuel public, comme l'a rappelé, notre rapporteur général en est peut être le symptôme tôt ou tard, il faudra cependant qu'elle intervienne d'autant plus vite que la contribution à l'audiovisuel public, n'existe plus, si nous ne sommes pas nostalgique de cette contribution, mon groupe partage quelques-uns des grands principes préconisés par le Sénat, à travers sa mission sur le financement de l'audiovisuel public, une stratégie de regroupement des entreprises de l'audiovisuel public, d'un côté et une budgétisation des ressources de l'autre. Tout autant que le secteur audiovisuel, la presse écrite, le livre et les industries cru culturel ont besoin d'un soutien public fort, les moyens de la mission, en hausse de 0 6 % en autorisations d'engagement et de quatre quatre pour quatre 4 % en crédits de paiement seront utilement complété par le plan d'investissement France 2030 cette orientation est indispensable, comme j'ai pu le dire pour la culture, lors du débat précédant ces secteurs sont également au coeur du projet républicain. En particulier à travers le soutien à la presse et à sa distribution, il est question de veiller au pluralisme de l'information, un principe indissociable de la démocratie, je partage le constat souvent exprimée, ici d'une réorientation du système des aides à la presse, il mérite au minimum d'être mieux que que l'éré corrélé avec ses objectifs de diffusion de pluralisme et de modernisation, s'agissant de la distribution, l'élu du Rhône que je suis ne va pas se plaindre des Messageries lyonnaises de presse, le brillant second devenu 1er devant France messagerie pour reprendre les mots du rapport de la commission culture je ne parlais pas de l'OL pour pas froisser mes collègues, cependant, il s'agit, sérieusement, de veiller à ce que les 2 opérateurs puisse lui survivre au sein d'un marché structurellement en baisse concernant le versant éditoriale de la presse, je me réjouis de la bonne résistance de l'Agence France-Presse dans un climat concurrentiel tendu avec les grands acteurs de l'Internet, l'AFP délivre une information qualitative qu'conforte garçon grâce à son service remarqué de vérification des faits la stabilité en 2023 de la subvention versée par l'État, conformément au contrat d'objectifs et de moyens 2019, 2023 devrait conforter sa position, même si les défis qui concerne l'agence sont loin d'être épuisé. Je souhaiterais également évoqué la situation du dont le modèle était également fragilisé, je m'inquiète du blocage entre les éditeurs et les auteurs qui ne parviennent pas à signer un accord sur une plus juste rémunération des seconds, faut-il rappeler une évidence au Syndicat national de l'édition sans création, il n'y a pas d'édition. Quant aux librairies le soutien qui leur a été apportée durant la pandémie a été essentiel elles attendent toutefois un geste concernant le seuil minimal pour les frais de port, j'en profite pour évoquer le sort de plus en plus incertain des quelque 150 librairies expatriés qui souffre encore davantage du problème des frais de port, aggravée par celui des délais de livraison pour leurs clients, il faut absolument les aider car elle représente indiscutablement un levier de la francophonie dans le monde, enfin, je terminerai par un mot sur le Scénique Chine cinéma durement éprouvée pendant la pandémie ce secteur inquiète depuis longtemps et, après avoir cité Malraux tout à l'heure, je citerai Mitterrand devant le Parlement européen en 95 qui disait alors que nous célébrons le centenaire du cinéma, l'art le plus populaire du siècle n'a jamais été si menacée dans chacun de nos pays, il n'a d'ailleurs plus besoin d'être menacée dans un certains nombres de ces pays là, car il a déjà disparu depuis cette date, le modèle français résiste, il faut dire que le CNC accompagne plutôt bien les mutations auxquelles le cinéma doit faire face, nous devons cependant toujours rester attentif à l'équilibre à trouver, avec les plateformes de streaming, la principale menace une fois encore travailler au maintien d'une création cinématographique française dynamique, c'est contribuer au rayonnement de notre pays et de notre souveraineté culturelle dans le monde, mes chers collègues, dans ce contexte, le RDSE votera les crédits de la mission. Merci, la parole est à monsieur Max Brisson pour cinq minutes pour le groupe Les Républicains. madame la présidente, madame la Ministre Mesdames, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, à l'heure où nous débattons du budget de la culture pour 2023 comme tout à l'heure, la question qui s'impose et la pertinence du fléchage des crédits ainsi pendant que l'industrie du niveau d'après ce débat contre l'inflation des prix du papier que c'est de la musique fait face aux évolutions comportementales de ses consommateurs et ne bénéficient pas de CNM efficient, celle du cinéma, rencontre une baisse inquiétante de fréquentation alors que s'amoncellent pour les salles, la menace d'une remise en cause de la chronologie des médias, une industrie, quant à elle, ne cessent de tirer habilement son épingle du jeu, c'est celle des jeux vidéo qui enregistre une progression exceptionnelle de son activité de treize que 5 % sur les 2 dernières années, au point de faire de la France, l'un des principaux leaders du marché notamment dans Sud et d'édition, un exemple qui invite à l'optimisme, comme je vous le disais tout à l'heure votre projet de budget prend-il vraiment compte cette diversité des situations dans le fléchage des crédits alloués, la réponse est disons insuffisamment pour autant comme nous croyons comme vous, Madame la Ministre, au retour des jours meilleurs, les sénatrices et les sénateurs LR voteront les crédits accordés à cette mission, néanmoins, nous avons un point de divergence de taille qui a déjà été exprimée le traitement réservé à l'audiovisuel public, non pas sur la suppression de la redevance en tant que telle mais plutôt sur la méthode employée, car une fois encore, comme l'on dit Roger Karoutchi Jean-Raymond Hugonet nous assistons, impuissants, à la mise en oeuvre du d'une décision dont la finalité à Paris aussi floues que la prise de décision aurait été précipitée ni retrouvons-nous pas là tous les ingrédients d'un mode de gouvernance une annonce inattendue qui aboutissent Renault mesures que le gouvernement pris de court, peine à justifier et à financer cette mesure amplifie en fait une réalité un pilotage on un pilotage à vue sans cap, sans stratégie qui ne génère que du malaise, les personnels de l'audiovisuel public, déjà inquiets sont désormais décontenancé par une annonce électorale dont la mise en oeuvre a été imposé à marche forcée sans que ne fut pris le temps de réfléchir aux missions et à l'organisation de l'audiovisuel public dans un paysage bouleversé et qui n'a plus rien à voir avec celui qui, présidé à l'élaboration de la dernière loi d'orientation en 1986 je regrette donc le caractère précipité de cette décision, je regrette qu'elle n'ait pas été pensé dans un cadre général qui aurait permis d'anticiper ses conséquences et de justifier sa plus-Value, surtout, je regrette que nous n'ayons pas eu en débattre pour s'interroger collectivement sur l'avenir de l'audiovisuel public, le format et le modèle que nous souhaitons lui donner autant d'éléments qui aurait pu constituer le corps d'une loi, projet souvent annoncé mi-éternellement repoussées, selon toute vraisemblance, ni 2022 ni certainement 2023 2 succès droit 1986 date de la dernière loi nous prenons acte avec regret de ce nouveau rendez-vous manqué et pourtant que de sujets à traiter sur la place et les missions du service public sur le droit voisin la chronologie des médias, l'indépendance des rédactions, l'éthique des journalistes, les moyens et les missions de la com que de sujets envisagés face un paysage audiovisuel éclatée et où pourtant jamais on a autant parlé de risque de concentration, il n'y aura donc pas de grande loi sur l'audiovisuel seul en fait de près du prince isolé aura fait bouger les choses, nous en reparlerons, Moscou n'rediscuteront des avenants aux contrats d'objectifs et de moyens pour l'instant sans enthousiasme et suivre l'avis de nos 2 excellents rapporteurs Roger Karoutchi et Jean-Raymond Hugonet nous voterons sans enthousiasme les crédits affectés au compte spécial d'audiovisuel public et avec un peu plus d'envie, ceux de la mission Médias livre et industries culturelles et vous voyez madame la présidente, que j'ai tenus la mission que j'ai rock donne du temps. Merci. Prenez exemple sur Monsieur Bresson Madame Vanina Paoli-Gagin c'est à vous pour cinq minutes. Oui, madame la présidente, madame le Ministre, mes chers collègues, lors de la crise sanitaire, le soutien public en faveur des industries culturelles a été massif, il faut le dire, les tendances futures sont excellentes en 2022, les industries culturelles ont vu leur chiffre d'affaires a augmenté de 10 % pour atteindre les 18,2 milliards d'euros, le projet de loi de finances pour 2023 leur consacrent plus de 700 millions d'euros en autorisations d'engagement s'agissant de la Bibliothèque nationale de France, nous nous sommes tous, se réjouit de la réouverture du site Richelieu le 17 décembre dernier après un chantier de 10 ans la BNF et cette année, doté de 70 % des crédits du programme, on parle de plus de 232 millions d'euros en crédits de paiement, il faut rappeler que les 3 quarts du budget de la BNF sont dédiés aux dépenses de fonctionnement pour accueillir le public dans de bonnes conditions et assurer la préservation des ouvrages et documents, ces coûts risquent d'exploser avec la crise énergétique que nous traversons, concernant le livre et la culture, l'année 2021 a été qualifié d'exceptionnel, tant les ventes ont atteint des records, je souligne le succès du Pass culture ça a déjà été rappelé grâce auquel les libraires ont pu bénéficier d'une hausse de leur chiffre d'affaires, c'est une excellente nouvelle, mais il faut prendre ces chiffres avec précaution car il découle d'une situation hors norme aussi pour 2023 le PLF prévoit près de 23 millions d'euros en crédits de paiement reste en suspens la question de la hausse du coût du papier, ainsi que la question des relations entre auteurs et éditeurs et plus particulièrement des rémunérations au sujet de la musique enregistrée, le streaming a désormais pris le lead, je parle en mauvais français avec 10 millions d'abonnés en France et un chiffre d'affaires en hausse de 13 % en 2021, les perspectives sont très enthousiasmante, avec une prévision pour 2032 de près de 35 millions d'abonnés 2023 de près de 35 millions d'abonnés à un service de streaming en France, acteur majeur du secteur, le Centre national de la musique a démontré toute sa pertinence et son efficacité lors de la crise sanitaire, le projet de loi de finances pour 2023 lui destine 27 8 millions d'euros, mais des redéploiements de crédits pourraient être prévu au cours de l'année pour compenser la baisse de ses ressources propres, le cinéma, quant à lui, a bénéficié d'un fort soutien pendant la crise, avec un montant total de 430 millions d'euros, dont la totalité aura été dépensés à la fin de l'année, ces dernières semaines, nous avons été informés du recul préoccupant de la fréquentation des salles. Les premiers résultats dans l'écouter un petit peu, ou du moins la laisser paraître un peu de calme. à défaut de m'entendre les premiers résultats 2022 affiche un recul de 30 % par rapport à ceux de 2019, prends le plan France 2030 réservent 350 millions d'euros à la filière de l'image, le jeu vidéo, cela a été dit est un secteur qui affiche une belle croissance de 1,6 % en 2021, 5,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires, après des résultats déjà exceptionnel en 2020, c'est un secteur d'avenir qui représente un vrai levier d'attractivité et de rayonnement de la France, comme ont pu le souligner plusieurs acteurs majeurs de ce secteur lors de la table ronde organisée au Sénat le 12 octobre dernier il est nécessaire de poursuivre les efforts en sa faveur concernant la presse et les médias, le projet de loi de finances pour 2023 propose 360 et 11 millions d'euros de crédit en crédits de paiement, soit une progression de près de 6 % par rapport à 2022 après la crise sanitaire, la presse reste fortement dépendante au financement public, ce n'est pas une situation tenable sur le temps long, notre groupe est favorable à une évaluation des aides afin d'étudier la pertinence des crédits mobilisés reste à évoquer le compte de concours financiers avances à l'audiovisuel public, la suppression de la contribution à l'audiovisuel public public intervenu cet été ne fait pas débat tant elle nous paraissait injuste inadapté, en revanche, le financement du secteur par le fléchage d'une fraction de TVA ne semble pas être une solution satisfaisante sur le long terme, il faut poursuivre la réflexion pour conclure notre groupe s'inquiète des conséquences de la crise énergétique et de l'inflation pour les établissements et acteurs culturels les plus fragiles, toutefois : nous nous félicitons de la reconnaissance de l'importance des moyens fléché par l'État, vers nos industries culturelles et créatives, grâce à ce soutien conséquent ces industries participant au rayonnement de notre pays et faisant sa force doivent être aidés pour cette raison le groupe les indépendants votera ces crédits jour. Merci Madame la présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, la grande majorité des acteurs concernés par cette émission, mais il y a le livre et industries culturelles se trouvent aujourd'hui en grande fragilité, une fragilité née du bouleversement qu'a représenté pour les secteurs de l'information et de la culture, la généralisation des activités en ligne mais une fragilité qui a aussi été accentuée hier par la crise sanitaire et la fermeture des lieux culturels et qui le sera demain, par la mise sous cloche du pays avec la tenue des Jeux olympiques, plus que les autres secteurs, la culture subit de nos jours, une grande Exposition due au fait du prince, comment mesurer en effet n'aime pas que de la politique culturelle de l'État qui, d'une main, annonce le financement de milliards d'euros de projets culturels sur 5 ans dans le cadre du plan France 2030 et de l'autre menace de déprogrammer ou reporter les festivals en 2024 seuls les secteurs numérisé comme celui du jeu vidéo semblent épargnés et peuvent se projeter sur le long terme l'avenir dira également si la belle santé du secteur du libre-se maintiendra et je dis avec inquiétude que la fréquentation des bibliothèques municipales est toujours inférieur de sa fréquentation en 2019 en même temps la situation du cinéma et plus inquiétante car le système actuel repose pour partie sur la taxation des entrées en salle, l'entrée en vigueur des des Chris Mad qui acte la participation des plateformes de vidéo à la demande au financement de productions françaises ne garantit pas le retour des spectateurs en salle, la montée en puissance de la vidéo à la demande durant le confinement et le développement des formats très courts sur les réseaux sociaux représentent une concurrence peu chères, voire gratuites. Face à cette fragilité, l'État doit adapter l'aide financière qui l'apporte à chacun de ces secteurs il accompagné l'émergence de nouveaux modes de financement pour protéger les forces intellectuelles et créatives de ce pays,

dans le détail, cela représente 250 millions pour le développement d'offre culturelle immersive 350 millions d'euros pour un appel à projets, fabrique de l'image et 400 millions d'euros pour l'accélération des industries culturelles, France 2030 30 ah donc plus vocation à soutenir des initiatives émergentes qu'à préserver l'existant, l'attribution du pouvoir de la co-tutelle du CNC, de la Caisse des dépôts et des consignations nous éclaire également sur la forte logique économique qui sous-entend l'appel à projets, fabrique de l'image échappant du fait au ministère de la culture, nous ne pouvons donc pas nous en satisfaire la situation de la presse écrite, nous inquiète également, malgré le rebond de 2021, la question du système de distribution reste irrésolue aussi des aides à la presse devrait être orientés et conditionné comme nous l'avons évoqué lors de la commission d'enquête sur la concentration des médias, il me semble, Madame la Ministre, que le gouvernement a laissé peu de chances au crédit d'impôt pour le premier abonnement, nous avions d'ailleurs déposé plusieurs à demande demande destinée à l'étendre et à l'adapter, aucun n'a été retenue, l'avenir de l'audiovisuel public nous semble aussi compromis après 49 ans d'existence, la redevance a tiré sa révérence, elle est remplacée par une solution provisoire de financement qui crée comme il a été dit, un climat d'incertitude, le service public a besoin d'un financement stable et pérenne, sans être soumis aux aléas de la conjoncture politique ce financement est injuste car cette ponction de TVA pour pour tous les Français, ils ils participent tous au même niveau, ce qui n'était pas le cas, je vous le rappelle, de la redevance, il est encore possible d'améliorer le financement de l'audiovisuel public en augmentant la progressivité, nous avions proposé un amendement en ce sens là encore rejeté, nous attendons des garanties sur la pérennité de l'audiovisuel public c'est moyens son indépendance, l'importance de protéger ce pluralisme dépasse d'ailleurs notre pays tandis que se mènent des guerres de désinformation à travers le monde vous avez souligné le monsieur le rapporteur, le succès de TV5 Monde à l'étranger en 2022 sur 300 millions de francophones hein 8 millions de visiteurs sont originaires d'Algérie, du Maroc ou de l'Espagne, ce n'est certes pas l'audience la BBC World Service, qui compte 350 millions de spec téléspectateurs mais réserve d'audience reste à conquérir pour toutes ces raisons, nous ne voterons pas les crédits alloués à l'avance, disait public. Puis, moi, j'ai dépassé mon temps. La parole est à monsieur Gattolin pour six minutes non non, vous avez pas dépasser, je vous en empêcher. Madame la présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, impossible Madame la ministre, impossible à l'occasion de cette discussion générale sur les médias et les industries culturelles, de ne pas rendre hommage à Pascal Joseph, un homme de télévision exceptionnel qui nous a brutalement quitté la semaine dernière. Merci. à travers les nombreuses fonctions qu'il a occupé tant au sein des médias publics que dans les chaînes privées ou dans le monde du conseil Pascal Josèphe et nos devenu nonobstant sa retenue naturelle, un des acteurs les plus influents du paysage audiovisuel des 4 dernières décennies encore choqués par la disparition de celui avec qui j'ai très souvent eu le bonheur de travailler au cours de ma vie professionnelle j'avoue que l'avalanche d'éloges dont il a fait l'objet depuis une semaine, mais clair chaque jour encore davantage sur l'étendue impressionnante du respect qu'il suscitait, nous sommes ici nombreux à avoir bénéficié de ces perspicace analyse sur l'état de notre duo visuel et de ses mutations prévisibles, vendredi dernier, Jean-Pierre Leleux, notre ancien collègue me rappelait combien ces avis était inspirant pour les législateurs que nous sommes son expertise était toujours mue par un souci rare de l'intérêt général, sa disparition prématurée est une perte immense et ses écrits publiés sont malheureusement trop peu nombreux, comme on dit en Afrique, ce continent qu'il chérissait tant quant à sage disparaît, c'est une bibliothèque qui brûle pour autant et dans le débat qui nous a gêné Nîmes ici aujourd'hui, il serait bon, je crois, de lire ou de relire les premières pages du projet qui est étayé sa candidature à la présidence de France Télévisions en 2015 Pascal était un fervent défenseur de l'audiovisuel public, c'est la raison pour laquelle afin d'assurer sa survie à l'ère du numérique et de l'explosion des nouveaux acteurs internationaux, il considérait urgent d'entreprendre sa réforme, de grands principes guidaient son ambition à ce sujet d'abord que la vocation première du service public était dope servir, servir qui le servir le public évidemment se servir, servir et non se servir qu'à la tentation est souvent forte pour certains acteurs de l'audiovisuel, comme d'ailleurs dans tout le domaine de la culture d'oublier l'utilité de l'intervention publique cette hiérarchie des devoirs nécessite d'être périodiquement rappeler au risque sinon de voir le ministère se transformer en institution au service des seuls acteurs des industries culturelles à ce propos, nombre d'entre nous ont encore en mémoire la manière dont nous avons dû batailler pour faire aboutir une loi visant à supprimer la publicité dans les émissions destinées aux enfants sur le service public, une mesure pourtant plébiscitée par les Français, les associations de parents d'élèves, les consommateurs et tout le corps de la santé, la levée de boucliers que nous avons essuyé de la part des milieux dits professionnels, y compris de la part des dirigeants de du service public, à l'époque, reste dans les annales de cette maison et que dire au passage du rôle joué à l'époque par le CSA qui, après consultation des acteurs du marché et au sol, a cru bon devoir édicté un décret d'application restreignant le Champ d'application déjà étroit de cette loi sans même auditionné le Sénat qui en était à l'origine et qui a adopté en seconde lecture à l'unanimité, ce texte, la seconde ambition de Pascal Josèphe en prolongement de la précédente, c'était que la télévision publique devait porter et être porté par un véritable projet, un projet de société autant qu'un projet d'entreprise un projet visant à rassembler pour résister à la fragmentation toujours accrue du corps social, faire société pour retrouver et surtout incarner les valeurs fondamentales de notre République et de l'état de droit pour Joseph, la mère des batailles à l'heure du numérique de la délinéarisée et de la démultiplication des canaux de diffusion était celle des contenus, autrement dit la bataille du sens et lorsqu'on parle de contenu porteur de sens, on pense naturellement mais de manière trop exclusif à l'information, sa qualité, son indépendance et son pluralisme, on oublie trop souvent l'impact considérable de la fiction du patrimonial et même du divertissement sur les constructions mentales et dans la diffusion des idées, la fameuse série L'Instit que Pascal Josèphe porta sur les fonds baptismaux alors qu'il était directeur des programmes de France 2 en est une des plus belles illustrations, encore aujourd'hui, là encore, au moment où nous semblons redécouvrir l'importance des grands narratif et du rôle majeur qu'ils occupent dans la consolidation de nos identités collectives, la vision de la télévision, selon Pascal Josèphe, témoigne une fois de plus de son extrême pertinence et de sa nature anticipatrice et ce qui vaut pour notre audiovisuel national vous au moins tout autant pour notre audiovisuel extérieur aujourd'hui frontalement attaqué, notamment en Afrique par des narratif autoritaire développées par la Russie, la Chine ou encore la Turquie, les paroles du président de la République à ce propos, à Toulon, le 9 novembre dernier lors de la présentation de notre revue nationale stratégique nous oblige alors Madame la Ministre, au-delà du vote de ce budget de grands chantiers nous attendent, vous attendent si nous voulons redonner à notre de visuel sa pleine utilité sociale dans un monde en profonde transformation, je vous remercie. Madame la présidente, madame la Ministre, messieurs, mesdames les rapporteurs le budget que vous nous proposez et ton tremplin il semble aller dans le bon sens, avec une hausse affichée pour cette mission, mais c'est de l'affichage, car non seulement, cette augmentation est 2 fois moins importante que l'inflation, c'est donc une baisse, mais en ce qui concerne l'audiovisuel public il ne corrige pas la gigantesque baisse depuis 5 ans, qui l'a réduit à l'os, au moment où il est plus que nécessaire, au contraire de lui donner de l'oxygène pour remplir ses missions essentielles, d'information et de programmes culturels de qualité face à la concurrence des grands groupes privés et plateformes étrangères prédatrice à la désinformation organisée et à l'uniformisation des contenus, en effet, l'audiovisuel public connaît une situation très difficile, vous avez baissé son budget significativement pendant 5 ans, tout en vous privant de moyens pour son financement avec la désindexation de la Cap sur l'inflation, à partir de 2019 puis la fin de l'affectation de la TOCE l'audiovisuel public et maintenant la fin de la redevance, dans le même temps, vous avez réduit son périmètre avec la fin de France oh et heureusement que France 4 que vous aviez décidé de supprimer, a été sauvée in-extremis grâce en particulier à une très forte mobilisation de nombreuses sénatrices et sénateurs de la gauche et d'autrement dans cet hémicycle oui, malgré les discours convenus sur sa nécessité après l'avoir dénoncé, au grand bonheur de tous ceux qui veulent fin, honte de la République avait dit le président de la République, le service public de l'audiovisuel a connu des heures sombres sous le précédent quinquennat le plan dit d'économie affectant toutes les sociétés de l'audiovisuel public décidée en 2018 pour 4 ans, a constitué une perte de 688 millions pour lui dans son ensemble, cela s'est traduit aussi par le sacrifice des salariés avec 900 emplois supprimés à France Télévisions après des nombreux plans de départs depuis 10 ans et 4200 emplois à Radio France tous équivalents temps plein, et vous venez de parachever ce travail de sape en décidant cet été de supprimer purement et simplement la contribution à l'audiovisuel public pour financer l'audiovisuel en lui substituant une part de la TVA système ne garantissant ni son indépendance ni sa pérennité ni la justice sociale, puisque c'est l'impôt le plus injuste que tout le monde paye de la même façon qu'il soit riche ou pauvre, et même les personnes qui étaient exemptés jusque-là de la contribution du fait de leur situation de grande précarité.

et qui n'est plus exclusif aujourd'hui le poste de télévision à l'heure où l'on regarde sur une multitude d'écrans les programmes, mais elle avait le mérite de garantir l'indépendance ainsi qu'une pérennité depuis sa création, il fallait donc la réformer pour qu'elle soit non seulement juste mais moderne, vous n'avez fait ni l'un ni l'autre, nous avons fait une proposition alternative à travers un amendement que vous n'avez pas soutenu, qui crée une contribution progressive cette alternative et entraînerait une économie sur le coût de la redevance pour 85 % des foyers fiscaux français, c'est une solution plus juste socialement plus moderne car ne s'appuie en plus au seul téléviseur et surtout qu'ils sanctuarisent un financement pérenne indépendant et Direct, nous avons déposé une nous avons déposé une l'avenir de l'audiovisuel n'est plus garanti car son mode de financement et temporaire, en effet, à partir du 1er janvier 2025, il ne sera plus effectif et vous avez fait savoir que le financement du secteur se ferait alors via le budget de l'État, un schéma qui avait pourtant été retoqué cet été par le Conseil d'État, je disais que votre proposition d'augmentation de budget était en trompe l'oeil, en effet, elle n'est même pas à la hauteur des prévisions d'inflation pour 2023, par exemple, quid de l'augmentation de 50 % de la facture d'électricité de Radio France et de l'augmentation de 22 % des coups de serveurs informatiques, j'ai proposé avec mon groupe, un amendement en première partie du budget pour pallier aussi à ce manquement mais vous ne l'avait pas soutenue non plus cette augmentation se traduira donc par une nouvelle baisse effective pour notre audiovisuel public pourtant il mérite d'être soutenu et pas qu'avec des belles phrases, alors que les médias télé et radio sont en baisse constante depuis 10 ans, Radio France et France Télévisions ont connu des records d'audience, Radio France réunit 15 millions de Français quotidiennement sur ses antennes, avec une progression de 2 millions d'auditeurs en 4 ans, France Télévisions quand elle touche 80 % de la population française chaque semaine tout écran confondus, représentant plus de 50 millions de citoyens ce succès sur le linéaire mais également sur le numérique est due à leurs investissements massifs sur fonds propres, sur les 3 dernières années, ils ont investi, Radio France 31,4 millions France Télévisions 511 millions pour innover sur la même période, avec une progression de 34 % en 2 ans, ils ont également réalisé un travail remarquable et remarquée lors des confinements de même le service public de l'audiovisuel est essentiel pour le financement de toute la création audiovisuelle et cinématographique française sans leur investissement importants les risques pour tout le secteur sont réels et pour être entraîner la fragilisation de toute la chaîne des acteurs jusqu'à la production, ce travail important réalisé par l'audiovisuel public, c'est aussi celui d'Arte et de France Médias Monde à côté et avec Radio France, France Télévisions Lina et TV5 Monde face à la concurrence internationale, avec notamment les Gafam, l'audiovisuel public doit continuer d'innover, et pour cela il lui faut un investissement à la hauteur de nos ambitions, c'est pour toutes ces raisons que nous voterons contre, sur le compte spécial avances à l'audiovisuel pour la presse, l'effort est insuffisant face à la crise à l'inflation au prix du papier à la crise du secteur et puis toujours pas ce que nous avons demandé à travers différents travaux une refonte des aides à la presse, j'ai pu parlé précédemment de création cinématographique et de l'impact du Covid sur l'audiovisuel public, le cinéma était également fortement impactés par cette crise sanitaire avec 96 millions d'entrées en 2021, la fréquentation Reggie certes une hausse de 47 % par rapport à 2020, mais représente une baisse de 55 % par rapport à 2019 2ème meilleure année en terme de fréquentation depuis 1966 cette situation est inquiétante pour le financement de la création et ce n'est pas la mise en application de la 10 ratisse Mad qui me permettra de combler ce manque de recettes, d'autant que la hausse des moyens du CNC pour 2023 ce sera seulement de 3 donc inférieure à l'inflation attendue pour ce qui est du livrent le budget de l'action est positif mais les inquiétudes du groupe socialiste, écologiste et républicain pour le secteur sont autre entre une concentration dans ce secteur, toujours plus importante, l'incertitude sur l'avenir d'Editis, numéro 2 français et l'impact que cela peut avoir sur la diversité, l'autre sujet inquiétant et la flambée des matières premières, si le chiffre d'affaires des éditeurs a connu une progression de 12,4 % le secteur connaît un vrai bouleversement des petites maisons d'édition connaissent de très fortes difficultés face aux plus grandes maisons d'édition avec des marges trop faibles avec les temps difficiles marquées par la pandémie, les éditeurs indépendants ont retrouvé les Lecteurs, mais la crise du papier et des manoeuvres financières dans le secteur sont inquiétants, il faut aider ce secteur plus plus massivement enfin l'industrie musicale n'est également pas en reste avec une situation compliquée que connaît l'ensemble du spectacle vivant, si le chiffre d'affaires de la musique enregistrée, connaît une progression la recette des billetteries de concerts, baisse de 10

pour finir, ce n'est pas parce que nous vivons une crise énergétique et inflationniste forte que la culture doit être minoré, c'est au contraire parce qu'il y a cette prise énergétique, sociales, économiques, climatiques et démocratique que plus que jamais la culture doit être. Doit être au coeur des politiques publiques pour faire autour des valeurs qu'elle incarne République ensemble. La parole est à madame Céline Brulin pour le groupe républicain, communistes, écologistes. Madame la présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, les crédits de cette mission sont marqués par une insuffisante prise en compte de l'inflation galopante et de la crise énergétique que nous traversons, par l'insuffisance de moyens dont la puissance publique devrait pourtant se doter pour faire face aux plateformes géants du web et autres grands groupes qui concentre de plus en plus de médias dans les mains de quelques-uns et même par des choix qui risque d'affaiblir considérablement la puissance publique à l'image de la suppression de la contribution à l'audiovisuel public qui n'est en rien un coup de pouce au pouvoir d'achat des Français, celle-ci n'est en effet que provisoirement, compensée par une fraction de TVA, l'impôt le plus injuste qui soit, et dont personne n'est exonéré, à la différence de la redevance et vous n'avez pas anticipé le fait que cette décision aurait pour conséquence de rendre les entreprises de l'audiovisuel public redevables de la taxe sur les salaires, ce qui nuance sérieusement l'engagement d'une intégrale compensation et qu'adviendra-t-il après 2025, nous souhaitons que vous répondiez à cette question lors de nos débats, Madame la Ministre, pour ce qui concerne la presse qui avec l'audiovisuel public, un pilier de notre démocratie, l'explosion du prix du papier, avec une augmentation bien supérieure à l'évolution d'autres produits menace de nombreux titres et du même coup le pluralisme 150 millions d'euros devaient être con consacrée au crédit d'impôt sur le premier abonnement décidé lors de la crise sanitaire, le dispositif n'ayant pas fonctionné, pourquoi ne pas affecter ces crédits à un soutien d'une autre forme, permettant de faire face à ces surcoûts, sans parler de l'amende de 500 millions d'euros du par Google et fort justement par notre rapporteur Michel Laugier, l'article 40 de la Constitution ne nous empêche, nous parlementaires de le décider, mais le gouvernement peut le faire et il serait souhaitable que ces d'privilégie les titres indépendants et favorise le pluralisme, cela pourrait même préfigurer une réforme des aides à la presse, comme l'a notamment demandé notre groupe en proposant le doublement de l'aide aux quotidiens à faibles ressources publicitaires dans le cadre de la commission d'enquête sur la concentration des médias concernant le livre, il convient de revaloriser le niveau minimum des frais de port, comme le demandent les libraires indépendants, puisque celui-ci est fixé dans dorénavant à trois euros alors que les frais de port leur revienne à un peu plus de 7 euros si effectivement ce seuil a le mérite de présenter une première étape, nous devons aller plus loin pour conforter le prix unique du livre, et rétablir les conditions d'une concurrence équitable entre les libraires et les plateformes en ligne, je souhaite insister, Madame la Ministre, sur les conséquences de l'augmentation du prix de l'énergie, cette augmentation considérable va affecter les salles de cinéma, et là encore nous pensons aux salles indépendantes, d'autant que les problèmes de pouvoir d'achat rencontrées par nos concitoyens peuvent affecter la fréquentation qui n'a pas encore retrouvé son niveau d'avant-Covid elle pèse aussi très lourd sur la Bibliothèque nationale de France, laquelle fait face à un surcoût estimé à 3 6 millions d'euros en 2000 22 et près de 15 millions d'euros en 2023, celle-ci a déjà connu la suppression de 300 postes en disant, alors même qu'elle voit ses missions augmenter avec la réouverture du site Richelieu la poursuite de la numérisation des documents ou encore le dépôt légal de numérique, il est temps d'engager un vrai débat sur le financement du Centre national de la musique, les trois ressources dont dispose le CNM ne permettent pas à l'établissement d'assurer les missions qui lui incombent d'accompagnement de la filière musicale en effet avec la baisse de 20 à 25 % de la fréquentation dans le secteur du spectacle vivant et en l'absence d'un projet de loi de finances suffisamment ambitieux l'année 2023 risque d'être compliqué, demi pour 100 sur le chiffre d'affaires générés par le streaming contribuerez à financer le CNM, avec l'Avantage d'aller chercher l'argent là où il y en a, cette taxe constituerait un modèle de redistribution qui pourrait rapporter plus de 20 millions d'euros chaque année enfin, concernant le secteur des jeux vidéos, nous regrettons le manque d'évaluation du crédit d'impôt dans le secteur bénéficie celui-ci pourrait d'ailleurs être conditionnée à l'amélioration des conditions de travail dans un secteur où la précarité et l'usage abusif des heures supplémentaires, restent très élevés, par conséquent, en raison d'un budget bien trop fragile, à nos yeux pour des secteurs essentiels à la vie démocratique, nous ne voterons pas ces crédits, je vous remercie.

Madame la Ministre, mes chers collègues. J'associe à mon propos, mon collègue du groupe Union centriste Jean gris qui s'exprimera pour la partie médias et audiovisuels, je débuterais mon propos par l'inquiétude qui pèse sur le secteur du cinéma, les Français ne sont jamais ceci peut aller au cinéma depuis 909 d'après les chiffres du CNC, le soutien au secteur des salles de cinéma et donc urgent si l'arrivée de nouveaux acteurs comme Netflix Disney, plus c'est Amazon Prime profitent financièrement à la filière, c'est à quel prix artistiques pour quel coût pour l'exception culturelle française et pour quelle évolution du public qui risque de s'éloigner encore plus des salles, ce budget, soulignant le affiche un soutien fort et bienvenue au CNC et à la cinémathèque française, de même les dispositifs fiscaux incitatifs pour le cinéma maintenu et développé participent largement à ce soutien concernant le Live, les nouvelles sont bien meilleurs après une année 2021 exceptionnel en librairie le livre continue de bien se porter, plus de 10 % en volume et en valeur par rapport à 2019 l'actualité du secteur est notamment marquée par la mise en oeuvre de la loi proposée par notre collègue Laure Darcos, ce qui amène reconnaissance et oxygène à la filière est un 1er pas pour les frais de port pour autant les coûts du papier, de l'énergie sont des menaces nouvelles sérieux à prendre en compte et à suivre notamment pour les petits éditeurs du côté de l'industrie phonographique, la dynamique est aussi positive, avec une 5ème année de croissance d'affilée et une protection, si ton dans les nouvelles mesures budgétaires le lancement du portail national de l'édition accessible qui va permettre, d'ici 2025 de se mettre en conformité avec les exigences européennes en matière d'accessibilité, simplifier les démarches des personnes handicapées pour se procurer repéré des livres est un atout supplémentaire pour la filière est une mesure des d'inclusion essentiel, le Centre national du livre, quant à lui, a les moyens pour accomplir ses missions doté d'un nouveau contrat d'objectifs et de performance pour la période 2022 2026 arrêts qui la rage bienvenue de ces missions s'annonce, il était très présent sur le soutien économique à la filière et ça joue déjà désormais dans ses objectifs, celui du développement, le développement de soutien à la lecture pour une politique culturelle et d'émancipation majeur pour nous tous et nous toute autre sujet, la situation d'avis, Bibliothèque nationale de France, est à surveiller, car l'établissement doit faire face à des nouvelles missions à plafond d'emplois constants, notamment, la réouverture du site Richelieu le musée ou le développement du dépôt légal numérique l'impasse budgétaire liée à l'inflation risque de conduire la BNF à ralentir et repousser des investissements importants, la création du Centre de conservation Damien la sécurisation de l'esplanade du site de Tolbiac et le renouvellement de son système à venons-en au Centre national de la musique, son financement Contini de soulever de vives interrogations l'accompagnement de la filière musicale par cette institution, impose une réflexion approfondie quant à ses missions et au financement supplémentaire pour que le CNM plus l'influence du streaming et du mur mérite du numérique prouve que les plateformes ah conçurent ont un rôle à jouer dans son budget le CNM a soutenu efficacement la filière durant la crise sanitaire, mais les ressources qui lui sont alloués sont inférieurs à ce qui avait été envisagé au moment de sa création, nous attendons le résultat de la mission de notre collègue Julien Bargeton pour donner enfin un cadre optimal à son financement je terminerai par le secteur du jeu vidéo fleuron national et secteurs économiques ultra dynamique, le fonds d'aide aux Jeux aux joue un rôle en soutien à l'écriture, la pré-production et la production des entreprises de création, nous soulignons cet effort pour un secteur très pourvoyeur d'emplois et qui valorise la France au plan international pour conclure madame ma Ministre nous retenons les efforts faits par le ministère dans ce budget, pour soutenir les secteurs des du livre et des et des industries culturelles, elles vont devoir faire l'objet d'un suivi très attentif, il participe ce secteur largement à notre économie et font pour les citoyens, bien plus simple. je vous remercie. Madame la Ministre, mes chers collègues, comme vous le savez, cette mission rassemble les crédits que le ministère de la Culture consacre au développement et au pluralisme des médias, il a sa politique en faveur du de la lecture publique et des industries culturelles, elle comporte de programme, le programme 180 Presse et médias et le programme 334 Livre et industries culturelles. Il n'a échappé à aucun d'entre vous, que la presse dans son ensemble a particulièrement souffert des années Covid et a dû faire face à une érosion important de son audition de son audience, qu'elle n'est pas parvenu à combler à ce jour, la désaffection du lectorat ce cumul malheureusement à des difficultés d'ordre structurel déjà anciennes, en particulier l'érosion de la diffusion papier et la transition numérique inachevée, certes, les pouvoirs publics ont mis en place des mesures d'urgence afin de garantir la continuité de la distribution de la presse et d'aider les acteurs les plus impactés par la crise sanitaire, mais dans ces aides, Madame la Ministre, n'oubliez surtout pas la presse de la connaissance et du savoir, ces mesures, ce sont d'ailleurs cumuler avec les aides transversales, dont l'ensemble des acteurs économiques a pu bénéficier en 2023 les dotations du programme 180 évolue de près de 10 % afin notamment de soutenir la mise en oeuvre de la réforme du transport de la presse, mais cette évolution positive ne tient pas compte malheureusement de la très forte augmentation du coût de papier en fin de compte, le saupoudrage des dépenses, notamment fiscales et sociales ne contribue pas, de mon point de vue à traiter à la racine les maux qui affectent l'ensemble des titres de la presse, s'agissant des radios associatives, acteurs de proximité important : le projet de loi de finances 2023 leur apporte une aide renforcée à travers le fonds de soutien à l'expression radiophonique locale abondé à hauteur de 1 virgule 7 millions d'euros, c'est une nécessité de cohésion sociale et je l'approuve, j'en viens à présent au programme 334 Livre et industries culturelles pour évoquer les crédits dédiés aux livres et à la lecture dans le contexte économique que nous connaissons, je voudrais mettre une crainte, celle de voir tout un pan de l'économie du livre s'effondrer comme vous le savez, les librairies sont le commerce de détail le moins rentables avec des marges extrêmement faible et des charges fixes élevés, salaires et loyers, elles sont donc particulièrement exposés aux conséquences de l'inflation et j'appelle le gouvernement à la vigilance sur ce sujet, permettez-moi également d'exprimer un regret, celui de la réforme mitigée des frais d'envoi des livres achetés sur les plateformes de vente à distance, pourtant voté à l'unanimité en 2021, dans le cadre de ma proposition de loi sur le livre, le montant de 3 euros minimum et la quasi-gratuité à partir de trente-cinq euros d'achat ne donne pas à mon avis aux libraires, les moyens de lutter, hein, mais à armes égales contre les géants Amazon et de s'installer sérieusement sur le créneau de la vente à distance, et j'espère surtout que Bruxelles dans sa notification n'y mettra pas carrément un coup d'arrêt, s'agissant du Centre national du livre, ces crédits sont abondés de 1 virgule 1 millions d'euros afin de lui Rom permettent de renforcer son action de soutien à la diffusion des Oeuvres et à la présence des auteurs sur l'ensemble des territoires ces crédits supplémentaires ont également pour objectif d'accompagner les éditeurs dans la mise en oeuvre de nouvelles obligations d'accessibilité aux personnes en situation de handicap, je ne peux que m'en réjouir, de même je salue l'intérêt que l'État porte à la Bibliothèque nationale de France, qui bénéficiera d'un abandon abondement conséquent de ses crédits d'investissement de fonctionnement lui permettant de mener à bien son ambitieux programme de modernisation du site François Mitterrand pour autant sera-t-elle en mesure de faire face aux conséquences de la crise énergétique, je n'en suis pas convaincu. Concernant la musique enregistrée, se pose en 2023 la question cruciale des moyens dont devra disposer le Centre national de la musique pour assurer la plénitude émission que la loi lui confie si Madame la Ministre de la Culture a rappelé que le budget 2023 du CNM était suffisamment solide, ce modèle de financement a néanmoins aviver les tensions parmi les professionnels de la musique, dans ce contexte, la mission parlementaire confiée à notre collègue Julien Bargeton est la bienvenue et elle permettra, n'en doutons pas de dégager des pistes pour un cadre financier cohérent avec toutes les précautions d'usage, je voulais souligner que la piste d'un financement moyen de la taxe sur la diffusion en visio vidéo physique et en ligne des contenus audiovisuels, dite taxe YouTube peut sembler pertinente plutôt que celle d'une éventuelle taxe streaming permettant de mettre à contribution les acteurs de la musique enregistrée payante, je ne voudrais pas conclure cette intervention sans évoquer la situation du cinéma, quelques couleurs de que quelques couleurs depuis la fin de la crise sanitaire, même s'il convient de rester prudent au regard de la baisse de la fréquentation de 30 % observée entre 2000 19 et 2022, la situation du Centre national du cinéma s'est quant à elle, stabilisées mais restent fragile à moins de vue financier. En dépit de l'augmentation de 1,9 % des taxes affectées en 2023 toutefois, dans son avis budgétaire notre collègue Jérémy Bacti n'a pas manqué de souligner le contexte économique particulier dans lequel évolue le cinéma peu favorable à la prise de risque, ainsi que les enjeux de la sobriété énergétique et du remboursement des prêts garantis par l'État, je vous remercie. Merci, la parole est à monsieur Jean, un vrai pour le groupe Union centriste.

madame la présidente, dames, la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je voudrais tout d'abord excuser notre collègue Catherine Morin-Desailly, spécialiste de lieu de visuel qui a été retenu par d'autres engagements je voudrais l'associer naturellement à mon intervention comme l'a dit notre rapporteur, jamais la situation de l'audiovisuel public n'aura paru aussi confuse incertaine que ça, c'est en fin d'année 2022 de rentrer dans une nouvelle étape après le vote de la loi audiovisuelle portée par Franck Riester nous voilà aujourd'hui au point mort puisque Roselyne Bachelot l'enterré en 2020, cette loi aura été cette loi aurait pourtant permis entre autres de clarifier le modèle économique et le modèle de financement pourtant promise par Emmanuel Macron en 2017, elle semblait indispensable, cerise sur le gâteau, cet été, au détour du PLFR on supprime la contribution de l'audiovisuel public, sans avoir pris soin d'en évaluer les conséquences et réfléchi, un mode de financement alternatives pérennes à l'occasion d'un véritable débat dans nos commissions, vous le savez madame la Ministre, notre groupe Union centriste au-t-il à l'accroissement de la dette publique souhaitait le report d'une année de suppression le temps précisément d'une étude sérieuse et d'un débat éclairé aujourd'hui nous achetons le fait que l'existence du compte de concours financiers à l'audiovisuel public est maintenu, alimenté par une France une fraction du produit de la TVA correspondant au niveau de dépenses prévues par la trajectoire financière des entreprises maintenant l'incertitude demeure sur le mécanisme qui sera retenu à compter de 2025 pour financer l'audiovisuel public de manière pérenne à cet égard, nous regrettons que les préconisations ne nos rapporteur de création d'une instance indépendante chargée de proposer une élévation pur annuelle des besoins de l'audiovisuel public, idée défendue par notre collègue Catherine Morin-Desailly dans des rapports antérieurs n'ait pas été retenues par le gouvernement, par ailleurs, les crédits inscrits sont certes en hausse mais cela doit être relativisée car nous avons découvert les effets fiscaux de la suppression de la caps donner non communiqué lors du PLFR à cela, s'ajoute pour France Médias et Arte, la perte du droit de déduire la TVA ayant pour conséquence d'augmenter leur charge en 2000 22 et 2023 reste l'inflation et les coûts de l'énergie qu'auront des conséquences non négligeables sur le budget, en dépit des économies réalisées à la hausse affichée des crédits ne se fera ne suffira donc pas pour compenser tous ces difficultés, nous craignons aussi que ces moyens ne suffisent pas à financer les nouvelles priorités de ces entreprises français les divisions doit être structurellement et financièrement capable d'affronter la concurrence et continuer à financer la création quant à l'audiovisuel extérieur, amené à jouer un rôle essentiel dans le monde troublé et menaçant que nous vivons l'actualité est là pour nous le rappeler tous les jours, nous sommes inquiets d'un niveau de ressources le financement de France Médias Monde et d'Arte n'est en effet plus suffisamment indépendant une dotation d'État s'étant substitué à une dotation publique voilà pourquoi en l'absence, à ce stade de mécanismes de financement appropriés et inscrit dans une loi organique, ce que ce que préconise ni plus ni moins que le rapport demandé à Lydia que nous ne pouvons que suivre l'avis du rapporteur, elle nous abstenir sur ces crédits, le groupe centriste, madame la ministre attaché aux missions de l'audiovisuel public restera particulièrement vigilants, exigeants dans les semaines à venir pour que l'émission dont il est doté, ne soit pas pas plus longtemps fragilisé et les personnels rassurer rassurés sur leur avenir, je vous remercie. Madame la présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, alors que les différents secteurs sont touchés par une crise multiforme, la hausse des crédits affectés ne suffit pas à masquer de véritables difficultés sur l'efficacité et la pertinence des dispositifs actuels, nous devons déplorer l'absence de véritables réformes pour une meilleure adaptation aux nouveaux enjeux, les usagers et les usages change les publics non plus les mêmes goûts et les acteurs de l'industrie culturelle propose de nouvelles démarches, le numérique est désormais une donnée incontournable dans tous les médias pour l'audiovisuel public, il faut aussi, il faut ainsi reconnaître l'absence d'une véritable réforme d'Apple d'ampleur attendue, la suppression de la redevance audiovisuelle est resté avant tout que la traduction d'une promesse électorale, une décision adoptée sans vision d'ensemble et sans solution concrète pour notre audiovisuel public, rien n'a été engagée sur son organisation, qui reste nécessaire, il y a quelques mois, mes collègues, Roger Karoutchi, Jean-Raymond Hugonet proposer la création d'un média public puissants et innovants pour répondre notamment au défi du numérique en raison de la concurrence des plateformes, il en est malheureusement rien, nous sommes loin de nos voisins allemands ou britanniques qui ont su mettre en place un réseau attractif et reconnu la hausse des crédits ne doit pas faire illusion : elle vise surtout à neutraliser les conséquences fiscales de la suppression de la redevance, le problème du financement des médias publics et prégnant, si le niveau des recettes et maintenu, rien n'a été fait pour évaluer les besoins de l'audiovisuel public et l'horizon 2025 nous inquiète quant à la presse, rien n'a été fait sur la réforme des aides, sauf pour les aides à la distribution, ce qui reste insuffisant, pas de redéfinition des rapports entre le système actuel des aides et le contexte numérique, nous avions émis le voeu avec le récent rapport de notre collègue Michel Laugier, que la presse régionale soit mieux aider pour la digitalisation en raison de nouveaux usages constatés chez les Lecteurs ce secteur doit être accompagnée pour qu'ils puissent se réinventer pour qu'ils puissent trouver lui-même les solutions, or nous ne les percevons pas. Pour rester dans le domaine de la culture, on doit saluer l'attachement des Français au livre, avec des ventes de livres, en hausse a été évoqué, mais ce qui est gagné d'un côté, grâce au goût des Français pour la lecture peut être hélas perdue par la hausse des prix du papier, rendant le prix des ouvrages inabordable. Concernant les frais de port pour les livres, ma collègue Laure Darcos savez déploré un alignement sur le modèle Amazon le niveau minimum pour des frais de port pour les livres est trop faible, ce n'est pas un message sérieux pour nos libraires et pour l'édition, l'application de la loi sur l'économie du livre est décevante, les éditeurs, les libraires et au-delà les Lecteurs sont en attente de fortes décision quant à la musique, il faut noter la poussée continue du streaming, c'est une consommation nouvelles destinées à être pérenne et qui pourrait être une base pour d'éventuelles ressources le financement du CMN du CNM reste posée, il a, il est insuffisant et une solution pour ces recettes s'impose : quelles seront les nouvelles ressources adaptées au streaming, faudra-t-il une taxe sur cette forme de consommation pour financer le CNM, là aussi, nous manquons de perspectives claires, parlons du 7ème art et laisse lui aussi éprouvé par la crise, le cinéma a symbolisé la vulnérabilité de la culture face à la crise sanitaire, nous sommes sortis des polémiques sur l'ouverture des salles mais la fréquentation a chuté d'un tiers par rapport à 2019, comme si les contraintes des gestes barrières était resté dans les esprits une véritable jauge mentale qui substitue aux anciennes parce qu'il manie l'image, le cinéma subit la forte concurrence d'Internet et des plateformes numériques, il y a donc urgence à réviser les soutiens à ce secteur comme le CNC s'y était engagé en janvier 2020 nous sommes en attente de décision forte comment redonner tout simplement aux Français le goût des salles de cinéma, voilà un test pour la politique du gouvernement, enfin la place du jeu vidéo se consolide

soutenons la création si nous voulons que notre pays garde sa place et comment prendre en compte la nécessité de préserver les jeunes publics, donc nous déplorons l'absence de réformes vitales et nécessaire dans cette mission, alors que des perspectives positives existent donc avec beaucoup de réserve, nous voterons les crédits de cette mission. Merci. Et Madame la Ministre, c'est à vous.

Madame la présidente, monsieur le président de la commission, messieurs et Madame, les rapporteurs spéciaux mesdames et messieurs les sénateurs. Je suis très heureuse de poursuivre cet examen de la seconde partie du budget du ministère de la culture à travers les crédits de la mission Médias livre et industries culturelles et le compte d'affectation spéciale avances à l'audiovisuel public les enjeux couverts par le livrer les médias et par notre diesel publics sont fondamentaux pour l'avenir de notre démocratie, surtout à un moment où notre pays est confronté, comme la plupart des sociétés démocratiques à une crise de l'information, nous sommes dans cette aire de l'immédiateté qui avait si bien analysé, Pascal Josèphe à qui vous avez magnifiquement rendu hommage cher André Gattolin, merci de cet hommage effectivement, recul de la confiance des citoyens dans les médias, transformation des usages perte de repère face à la profusion d'informations diffusées en ligne fragilisation du modèle économique de la presse, les défis sont nombreux pour consolider les acteurs des médias du livre des industries culturelles et créatives et permettre à la France de rester une puissance de rêve pour reprendre des mots de Malraux, ce budget 2023 se veut ambitieux, je dirais même, je pense qu'il est historique, ce sont 704 millions d'euros de crédits budgétaires 4,3 pour 100 de plus que l'année passée pour cette mission Médias livre et industries culturelles. Le compte d'affectation spéciale avances à l'audiovisuel public s'élève de son côté à 3 8 milliards d'euros, soit une hausse de un peu plus de 3 % par rapport à l'an dernier. Je m'y étais engagé cet engagement est tenu non seulement la compensation de la redevance c'est fait à l'euro près mais ce budget prévoit une hausse des dotations aux sociétés de l'audiovisuel public pour prendre en compte les effets fiscaux du changement du mode de financement et compenser les effets de l'inflation. La mission Médias livre industries culturelles pour 2023 et orientées autour de plusieurs grandes priorités, je veux d'abord évoqué le développement de la lecture qui m'est très cher sur tout le territoire dans la suite de cette dynamique, très forte, qui avait permis la lecture, grande cause nationale, s'il ne faisait aucun doute que les Français étaient attachés au aller à la lecture, vous l'avez tous dit la crise sanitaire a été l'occasion de le rappeler et de mettre en lumière notre première industries culturelles. Les librairies et les maisons d'édition ont été touchés par la pandémie, mais le soutien public, a été au rendez-vous avec de nombreux dispositifs sectorielles, sans compter, sans oublier le plan de relance pour les 2 dernières années. Le soutien au secteur du livre doit se poursuivre, ce budget est l'illustration de cette ambition 10 millions d'euros supplémentaires sont consacrés pour le développement de la lecture sur tout le territoire soutenir nos bibliothèques, le réseau des librairies, les maisons d'édition en région renforcé aussi des manifestations littéraires nous lançons également en lien avec le ministère des solidarités de l'autonomie et des personnes handicapées, le projet d'une nouvelle plateforme accessible à toutes les personnes en situation de handicap qui va référencer les livres adaptés à chaque handicap, ce sont 5 millions d'euros qui sont prévues jusqu'à 2025, des Budgets spécifiques seront aussi versés au Centre national du livre, pour inciter les éditeurs à adapter davantage de livres pour les personnes en situation de handicap des aides vont également être mises en place pour financer renforcer le transport des livres, ce sont plus 1 1000000 d'euros dans le budget, via la centrale de l'édition, pour faire face aux difficultés d'acheminement dont vous avez conscience vers notamment les territoires d'outre-mer et à l'international vers les librairies francophones, un enjeu qui me tient très à coeur. Notre mission est également de garantir le pluralisme des médias et l'accès à une information fiable, libre vérifier indépendante, c'est un enjeu majeur, je l'ai dit, pour l'avenir de notre démocratie dans les mois à venir vont se tenir les états généraux du droit à l'information auquel l'ensemble des acteurs concernés vont être associés ainsi que bien sûr tous les parlementaires qui le souhaitent pour le secteur de la presse, l'année 2023 marque la fin du plan de filière presse qui était l'un des plans majeur du plan de relance, mais je veux quand même rappeler l'ampleur qu'a été ce plan inédit avec 377 millions d'euros qui ont permis de financer les transition écologique numérique du secteur et vraiment réaffirmer l'attachement de l'État à cette presse qui là encore est un enjeu vital pour notre démocratie, le ministère de la Culture va continuer à soutenir le secteur la priorité que nous avions définie avec la filière, c'était la réforme de la distribution sur lesquels nous avons travaillé déjà depuis plusieurs mois, c'est pour ça que le budget est en hausse de 17,3 millions d'euros pour les aides à la diffusion, la compensation au transport postal. Mais vous avez raison, la hausse des coûts, notamment du prix du papier est une préoccupation forte, une préoccupation légitime des professionnels, je sais que vous y a tous attentifs et nous allons avoir l'occasion d'en parler lors de l'examen des amendements de millions d'euros sont également consacrées aux études préalables et au lancement des travaux d'un projet qui est très important à mes yeux la future Maison du dessin de presse futur lieu d'Exposition de création et de médiation, je veux également vous assurer de ma volonté de mener un état des lieux assez complet. Des aides à la presse pour travailler à cette réforme, que vous appelez de vos voeux, je ne suis ministre depuis 6 mois, j'ai déjà négocié un bon budget, mais maintenant, je vous l'accorde, nous devons travailler sur cette réforme des aides à la presse. Qui n'est pas une mince affaire pour le secteur des médias. Nous continuerons de soutenir les radios de proximité pour la 3ème année consiste utile en augmentant les crédits du fonds de soutien à l'expression radiophonique locale pour accompagner la croissance du nombre de radios associatives éligibles à ce fonds, puisque nous sommes passés de 690 en 2017 à 744 en 2022. Comme pour la mission culture. J'insiste aussi sur le fait que ce budget permet de répondre aux besoins immédiats du contexte énergétique. Mais aussi de préparer l'avenir en mettant la transition écologique de nos établissements de nos opérateurs au coeur de l'ensemble de nos politiques publiques 8 millions supplémentaires permettront d'accompagner les établissements publics de la mission Médias livre et industries créatives, face à l'inflation, ça c'est en en fonctionnement pour le Centre national de la musique 900000 euros sont prévus pour accompagner la transition écologique du secteur de la musique en 2023 c'est une amorce évidemment il y a les années suivantes, je sais, vous l'avez tous mentionnés, l'enjeu du financement du Centre national de la musique est au coeur de vos préoccupations. Le sénateur Julien Bargeton vient de commencer sa mission sur le financement de la filière musicale dans son ensemble, mais je voulais tout de même vous rassurer : n'a l'air très clair sur l'étape 2023, le budget 2023 je vous avez indiqué que le Centre national de la musique avait des des reliquats du plan de relance, je les ai revérifié il y a autour de 20 millions d'euros de reliquat qui vont s'ajouter au budget 2023 du Centre national de la musique, donc, n'ayez crainte, en 2023 le secteur sera bien accompagné et nous aurons les conclusions de la mission pour rediscuter ensemble de l'avenir, à plus long terme. Le secteur du cinéma, vous l'avez tous mentionnés, merci de votre engagement pour nos cinémas. Ce secteur a fait l'objet d'un soutien sans précédent sans faille du gouvernement pendant la crise sanitaire, il va continuer à être soutenu le montant des taxes affectées au CNC va au CNC va atteindre 711 millions d'euros, une légère hausse par rapport à 2022. L'enjeu principal des semaines passées, les mois à venir, évidemment celui de la fréquentation de nos salles de cinéma, vous l'avez tous dit une baisse de fréquentation attendue à la fin de cette année, de l'ordre de 25 % peut être 30 % de baisse, j'espère que 25 % de baisse mais je reste optimiste, je suis optimiste, pourquoi, parce que je puisse être optimiste, déjà dans l'histoire, au début des années 90 on nous avait prédit la mort du cinéma parce que la télévision à les tuer le cinéma nous avions chuté à une fréquentation annuelle de 110 millions de spectateurs en 1992 et pourtant les salles se sont réinventées les films ont été au rendez-vous et, petit à petit la pente a été remonté et nous sommes arrivés en 2019 avant le Covid à 213 millions de spectateurs sur l'année, donc c'est possible, c'est possible, le cinéma n'était pas mort par la télévision, le cinéma ne sera pas tué par les plateformes par ailleurs cet optimiste je le puisse, dans la comparaison avec nos voisins européens, quand je vois que 60 % de baisse de fréquentation en Italie 40 pour % en Allemagne ou en Espagne ou en dehors de l'Europe moins cinquante pour cent, en Corée du Sud, je me dis que tout de même, le secteur du cinéma en France a mieux résisté que les Français restent un peuple de cinéphile et que nous avons un vrai appétit pour les films français en salle l'émotion en salle sur grand écran, comme ont pu le montrer, le succès de films comme Revoir Paris la nuit du 12 en ce moment l'innocent Simone le voyage du siècle ou encore novembre l'État accompagne fortement cette reprise à travers le passe culture aussi nous l'avons évoqué tout à l'heure, puisque pour vous prendre un exemple uniquement entre janvier et août 2022, ce sont 2 5 millions de séances de cinéma qui ont été réservées via le passe culture, c'est un vrai appui à la fréquentation des jeunes et donc le public de demain également, je veux préciser quelque chose par rapport au plan France 2030, que vous avez été plusieurs à mentionner ce que les l'État accompagne le secteur du cinéma aussi via ce plan qui est massif, qui est très ambitieux Madame de Marco, je voulais juste vous dire que le ministère de la culture est pleinement impliquée dans dans ce plan puisque le CNCC, le ministère de la culture, c'est une administration centrale du ministère de la culture même, nous sommes pleinement mobilisés sur cet appel à projets grande fabrique de l'image qui vient d'être clôturé 175 dossiers émanant de 13 régions, vous voyez la diversité ont été déposées, on a la trois objectif : soutenir des infrastructures de tournage soutenir des studios de jeux vidéos d'animation d'effets visuels de post-production et soutenir des formations parce que là on a un enjeu aussi de développer les compétences et les talents, tout ça, c'est le plan France 2030 et le notamment l'appel à projets grande fabrique de l'image qui est très territoriale et qui brosse vraiment l'ensemble des secteurs des industries créatives, j'en viens maintenant au compte d'affectation spéciale avances à l'audiovisuel public qui augmente de 114,4 millions d'euros pour atteint 3,8 milliards d'euros. Nous avons eu de nombreux débats cet été, je ne vais pas y revenir, surtout qu'il ne me reste plus que 4 minutes 30, nous avons pleinement tenu nos engagements, je l'ai dit, je le redis, le PLF 2023 apporte une compensation à l'euro, près de la redevance et des effets fiscaux liés au changement de financement, bien sûr, nous avons aussi tenu compte en partie de la hausse des coûts de l'énergie, et bien sûr de l'inflation, je ne reviens pas sur tous les chiffres que j'ai explicité en commission mais je veux rappeler que toutes ces hausses, entreprise par entreprise, ont été déterminés par l'État sur la base de projections qui ont été produites par ces entreprises et discuter bien sûr avec elle. Nous avons eu l'occasion à plusieurs reprises d'échanger sur le calendrier, la trajectoire financière pluriannuelle de l'public va être fixé en 2 temps dans un 1er temps un avenant au contrat d'objectifs et de moyens actuels 2000 22022, ce qui va être signé là d'ici la fin de l'année 2022, qui va fixer les cibles à atteindre et la dotation publique de 2023, dans un second temps à Lucy de travaux qui vont évidemment associer le Parlement dans le cadre d'un dialogue nourri avec les entreprises de l'audiovisuel public de nouveaux contrats d'objectifs et de moyens vont être au au cours de l'année 2023 et vont être adossé à une trajectoire de dotation pluriannuelle, je l'ai dit je souhaite que ces nouveaux contrats d'objectifs et de moyens et une durée de 5 ans. Pour se donner la plus grande visibilité possible et j'ai déjà indiqué quelques grands axes grandes priorités qui à mes yeux doivent guider ces nouveaux contrats d'objectifs et de moyens, nous avons parlé de l'information, sa fiabilité, son pluralisme, nous avons parlé de la jeunesse, n'oublions pas les derniers chiffres Royaume-Uni les jeunes regardent cette fois moins la télévision que leurs aînés des chiffres dont nous ne sommes plus très loin, nous avons parlé de la création, nous savons l'importance du financement de la création par le diésel, public, nous avons évoqué la proximité nous avons évoqué je vous remercie aujourd'hui de le rappeler l'importance de l'audiovisuel extérieur, surtout à un moment de grande manipulation de l'information et d'ingérence étrangère. Voilà, Mesdames et messieurs les sénateurs, les quelques priorités que je voulais réaffirmer pour cette mission Médias livre et industries culturelles les ambitions que je peux porter pour l'audiovisuel public, je voulais saluer votre engagement sur ces enjeux et je me réjouis de pouvoir poursuivre avec vous l'échange nourri que nous avons entamé ces derniers mois et je libère 2 minutes de temps pour la suite. Je vois que vous préféreriez qu'on finisse cette après-midi je veux merci, je vous rappelle que pour la cette mission de la conférence des présidents a fixé la durée maximale de la discussion à 2 heures 15, ce qui devrait nous amener à 20 ça, comment ça tourne donc si vous ne avez pas fini, vous savez que c'est reporté après nous commençons avec les amendements portant sur l'écrit, de la mission Médias livre et industries culturelles avec un amendement de monsieur dessus de 526.

cette année, enfin l'année prochaine mais il reste quand même des inquiétudes, et notamment des inquiétudes, porté par les petits acteurs culturels et donc même si nous saluons la mission qui a été confiée à un autre collègue Bargeton sur les ressources du CNM, elle devrait rendre ses conclusions qu'en courant 2023 et donc en traduction PLF ça veut dire plutôt au 24. Et donc pour nous proposons pour soutenir les filières musicales d'instaurer un fonds doté de 20 millions d'euros pour l'année 2023 pour que le CNM puisse tourner tourner un bol d'air financier qui devrait lui permettre de passer l'année difficile avant de disposer de ressources pérennes. Quel est l'avis de la commission sur cet amendement. Retrait ou avis défavorable, comme l'a dit le gouvernement, et comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons reçu les responsables du CNM, qui n'ont pas de soucis financiers pour l'année 2023 qui en ont pour 2024 donc la mission de Julien Bargeton décidément très cité doit nous donner dans quelques mois, et à partir de là, on demandera évidemment à ce que le budget soit réaménagé. votre amendement est déjà pris en compte, puisque j'ai indiqué un reliquat d'environ 20 millions d'euros que j'ai obtenu un report sur 2023, donc il y aura bien un plus de 20 millions d'euros dans le budget 2023 du Centre national de la musique en attendant de préparer l'avenir. Monsieur Bargeton. Merci ma présidente rapidement pour pas rallonger les débats puisque la mission qui m'a été confié, a été cité s'agit en effet de faire le point sur les dispositifs notamment du Centre national de la musique et leur bilan donc de revenir sur l'historique et puis d'en tirer des conclusions d'analyser le marché, ses besoins d'objectiver et de documenter la réalité des besoins et notamment des feuilles de marché qui justifie l'intervention publique de d'élaborer des scénarios de voir qu'elles sont toutes les pistes possibles avec leurs avantages et leurs inconvénients et puis enfin de faire un certain nombre de position proposition d'ailleurs sur le Centre national de la musique, mais pas simplement de manière générale sur la la gouvernance, l'organisation et la stratégie en matière de filière musicale en France, donc pour toutes ces raisons, et par cohérence vis-à-vis du rapport que je dois rendre évidemment je je ne pourrai pas voter, c'est cet amendement mais, mais, en tout cas évidemment la défense de votre amendement et il croyait bien que que je je m'appuierai aussi sur les travaux du Sénat et sur les remarques nombreuses des de de mes collègues sur le sujet de du financement de la filière musicale en France merci beaucoup. Nous soutenons en tous points l'état d'esprit et la volonté exprimée par cet amendement, on a pensé aussi à faire quelque chose allant dans ce sens mais symboliquement tout de même dans ce débat, le fait de devoir gagé sur des crédits pris à la presse et très problématique parce que le le secteur de la presse aujourd'hui n'est pas celui sur lequel on peut aller chercher à grappiller des sous pour alimenter le reste donc nous allons nous abstenir.

Cet amendement vise à soutenir le modèle des éditeurs privés de services de télévision et de radio à vocation locale opérant dans les territoires d'outre-mer, ces acteurs jouent un rôle essentiel à plusieurs titres, ils mettent en avant des identités des cultures et des traditions locales par une offre de proximité plurielle et diverse, il resserre les Liens entre nos territoires éloignés et la métropole, une mission qui s'est révélé crucial pendant la peu et ils assurent le rayonnement de la France sur les bassins Pacifique indien et Caraïbes, ces opérateurs permet également un accès gratuit aux meilleurs programmes des chaînes privées hexagonale pour les populations locales, je n'oublie pas leur audience et leur poids économique, il rassemble près d'un 1000000 de personnes chaque jour sur 3 zones et emploie plus de 500 salariés d'hiver et et environ 700 intermittents qui travaillent au sein de groupes audiovisuels intégré dans les territoires, hélas, malgré tous ses atouts, leur modèle économique est aujourd'hui gravement menacée en raison des charges anormal de transport et de diffusion liées à leur éloignement du territoire national et aux spécificités de leur zone géographique de diffusion dont craignant que ces éditeurs de télévision et de radio ne subisse le même sort que celui de la presse régionale quotidienne régionale, notamment les Didi les liquidations qu'ont vécu le GIR et France Antilles cet amendement d'appel vise à sensibiliser le gouvernement sur la nécessité d'accompagner leur modèle et de garantir leur pérennité. Merci madame Jasmin pour le 564. à vocation locale opérant dans les différents territoires d'outre-mer et à garantir leur pérennité afin que, à l'instar de ce qui se fait dans l'Hexagone et dont bénéficie évidemment nos concitoyens les populations des outre-mer continue de bénéficier de manière effective de la gratuité d'accès à de nombreux programmes de la diversité des offres audiovisuelles du pluralisme des expressions, ainsi que de la mise en valeur des identités et cultures locales, il s'agit également de préserver des emplois Directs et indirects environ entre 500 et 700 en fonction des périodes mais l'objectif in fine et et que le gouvernement accepte de créer une aide directe et pérenne, allant en ce sens dès 2020 23 pour rappel, le rapport de la délégation des outre-mer de 2 entre 2018, 2019 avec comme rapporteur Jocelyne Guidez et Maurice Antiste prévoyait déjà qu'il y ait une prise en compte réelle, la situation des outre-mer à l'époque il s'agissait de fermer France oh, nous avons été opposé plus ou moins, mais le gouvernement a fait un choix, et aujourd'hui nous voyons que nous avions raison, compte tenu des conséquences que nous voyons, par rapport à la situation des différents médias dans nos territoires, donc je souhaite vraiment que ce sera pris en compte et que nos outre-mer sera doté de moyens suffisants pour permettre à ces médias de poursuivent leur activité merci. Monsieur rapporteur, quel est l'avis de la commission sur le 679 et le un système très spécifique, avec quand même une petite réserve sur les deux amendements c'est qui sont engagés sur le livre et la lecture, ce qui quand même, c'est un peu peu un peu difficiles, chacun le comprend bon même si je sais les obligations de la LOLF mais que ce soit, cet élément là où le reste mais vie du gouvernement. Madame la ministre, le rapporteur sollicite votre avis. Merci madame la présidente, monsieur le rapporteur oui c'est gagé sur le livre et justement je venais d'expliquer l'augmentation dans le budget pour la distribution des livres notamment en outre-mer, là vous parlez j'ai pas très bien compris si vous parlez globalement de tous les médias en outre-mer ou spécifiquement des éditeurs privés de services de télévision, de radio à vocation locale il y a eu effectivement une aide exceptionnelle pendant la crise sanitaire, certes, à l'issue de la crise sanitaire, on voit bien qu'il y a des fragilités économiques plus structurelle, je je je considère un peu votre amendement plutôt comme un amendement d'appel qui va nous inviter dans ce cette réforme des aides à la presse et aux médias, radios et télé réforme des aides aux médias et au pluralisme au sens large, je pense à regarder de plus près, mais là j'ai pas l'évaluation très précise, et je voudrais pas réduire l'aide que nous avons pour le livre, notamment pour l'outre-mer donc demande de retrait. Pour les deux. OK, monsieur le rapporteur, vous suivez la Ministre bien donc je mets Madame Robert. Oui merci ma mère représente très brièvement pour dire que, effectivement, ce sont 2 amendements mais vous avez que le gage, on passe de 1 1000000 à 10 millions c'est quand même pas rien, la différence, l'évaluation qui a été faite par notre collègue Victoire Jasmin avec les acteurs et bien de un 1000000, et bien sûr le gaz sur les livres à la lecture n'est pas, nous ne le souhaitons pas donc nous demandons à la ministre de lever le gage d'un million. Bien je madame la ministre ayant donné un avis défavorable, j'imagine que vous ne l'avez pas gages, donc je vais mettre aux voix, d'abord, l'amendement 79 double avis défavorable qui est pour. Oui, donc, qui est contre. Qui s'abstient, il n'est pas adopté le 564 maintenant, qui est pour. qui est contre.

qui est contre. n'est pas adopté le 721 madame de. Merci madame la présidente, cet amendement vise à créer une aide exceptionnelle de 5 millions d'euros à destination des éditeurs de presse d'information politique et générale dites IPG il vient orienter plus spécifiquement cette d'aide ponctuelle vers les éditeurs de presse qui touchent aujourd'hui moins de 350000 euros par an, or aide spécifique aux postage et au portage soutenir les petits éditeurs de presse IPG c'est venir en aide à ceux qui sont les moins aisés des et qui souffrent le plus d'augmentation significative du coût du papier qui a plus que doublé depuis janvier 2021 en effet, les aides à la presse en général sont déjà capté pour leur grande majorité, pas la presse papier plus particulièrement pour les grands groupes de la presse papier, rappelons que le groupe aujourd'hui en France, Les Échos-le Parisien, propriété de Bernard Arnault et le 1er bénéficiaire des aides de la presse en France avec plus de 15 7 millions d'euros en 2021 au seul titre des aides individuelles, j'espère qu'au vu combien trier mes chers collègues, que cette aide ponctuelle doit donc être fléché vers ceux qui en ont le plus besoin des titres de presse fragilisé par l'augmentation continue du coût les papiers et qui nous incombe de soutenir, au nom de la pluralité des opinions de la diversité des médias dans nos territoires et de la Défense, une presse libre, merci. Retrait ou défavorables, c'est franchement pas les éditeurs de presse IPG qui sont ni les plus mal servis, ni les plus menacés donc dans dans tout ce que nous avons demandé au gouvernement sur la réforme des aides à la presse, franchement, je pense qu'il faut attendre un peu, cette réforme sur la diversité sur l'ensemble des aides mais c'est pas les IPG qui sont et de loin les plus menacés, qui plus est vous gagez là encore sur Presse et médias, c'est quand même un petit peu compliqué, je le reconnais, madame la Ministre. Merci madame la présidente, madame la sénatrice demain. Cause c'est cet enjeu du du soutien au secteur de la presse face à la hausse du prix du papier, nous l'avons identifié depuis plusieurs mois, le Sénat d'ailleurs également mis en lumière ses difficultés à travers le travail du sénateur Michel Laugier, que je remercie, qui a remis un rapport à la fin du mois de juin dernier. Dans le cadre du projet de loi de finances rectificative pour 2000 dans 22 vous avez voté il y a quelques jours, un dispositif exceptionnel et ponctuel, proposée par le député Denis Masseglia à hauteur de 5 millions d'euros, ils y sont. Plus largement, en ce moment, nous travaillons à un dispositif qui va être exceptionnels et conjoncturels de soutien pour les éditeurs les plus en difficulté. Pas uniquement éditeurs de presse IPG je précise, qui voient leurs coûts de production augmenter de manière très très très significative, donc je je peux pas encore vous annoncer ce montant, il ne sera pas, il sera pris sur des crédits existants redéploiement peut être du plan de relance ou en tout cas en gestion, je, je suis en train d'y travailler, j'espère pouvoir vous confirmer ce montant dès que possible, plusieurs pistes sont à l'étude, mais en tout cas, il y aura bientôt une enveloppe supplémentaire pour soutenir les éditeurs de presse face à cette hausse du coût du papier, donc c'est une demande de retrait. Encore une fois, je, je, je pense que l'intention est tout à fait louable de cet amendement, mais je mets en garde sur le danger de créer un autre programme alors que l'enjeu est de faire que dans ce programme, un autre programme financé ponctionné sur le programme existant alors que l'enjeu est de procéder à une redistribution plus équitable à l'intérieur et je suis complètement d'accord avec le fait qu'aujourd'hui on doit inverser la façon dont les aides à la presse ou constitué les grands groupes qui sont adossés à des grands groupes très solide financièrement, souvent d'ailleurs étranger au monde de la presse aujourd'hui reçoivent l'essentiel de l'aide publique, ce qui est antinomique avec l'aide publique publique c'est pas pour aider ceux qui sont solides et qui ont d'autres moyens privés de tenir et

il faut remettre les choses à l'endroit et y compris avoir une augmentation de ce programme, mais faire un programme à côté, en ponctionnant ce programme, je pense que c'est laisser au gouvernement le choix de choisir sur sur quoi il ponctionnera et d'ailleurs il peut fonctionner sur déjà la petite ligne qu'il y a dans le programme pour aider la la presse indépendante et les nouveaux entrants, donc ça serait quand même, c'est une possibilité, nous on s'abstiendra sur l'amendement mais sur le fond, on est complètement d'accord avec l'intention. Je mais aux voit cet amendement double avis défavorable. Qui est pour, qui compte. Il s'est abstenu, n'est pas adopté le 680 madame brûle, Merci madame la présidente. Ce cet amendement propose une aide d'urgence de 3 millions six en direction de la Bibliothèque nationale de France 3 millions six qui correspondent au surcoût de l'énergie pour l'année 2022, monsieur le rapporteur, vous avez dit qu'il fallait beaucoup plus pour la Bibliothèque nationale de France, je ne saurais mieux dire mais vous avez évoqué aussi le gouffre qu'il fallait combler et nous proposons de commencer à le combler avec cette aide d'urgence, je ne reviens pas sur la situation que connaît globalement la Bibliothèque nationale de France, mais pour faire face au surcoût énergétique, il nous semble que ce serait indispensable, et nous demandons au gouvernement de lever le gage en ce sens, merci. Retrait ou défavorables, j'ai dit tout à l'heure par non pas par plaisanterie mais par provocation que si on fait les changer toutes les fenêtre s'étaient des dizaines de millions sur le surcoût de l'énergie, les responsables, admettent que dans le redéploiement en interne, ils y parviennent, pour 2023 je vous cache pas, Madame la Ministre, que pour 2024 si évidemment il y a encore des travaux et des charges supplémentaires, la BNF devra trouver des ressources supplémentaires, mais le le budget de la BNF a augmenté de 10 % en 4 ans, il est à 233 millions d'euros, qui plus est vous gagé sur Presse et médias bon à un moment, ça, ça devient un peu compliqué, donc je je préférerais franchement qu'on en reste là, merci Merci madame la présidente, alors pour la BNF, en fait, nous faisons une augmentation assez nette au PLF 2023 de sa subvention de 8 7 millions d'euros tout de même. Dont 5 millions sont fléchés. Pour accompagner la hausse des coûts parce que on a évalué dans cette enveloppe, ce que j'ai présenté tout à l'heure de 56 millions quels étaient les établissements qui étaient de véritables passoires thermiques je ne reviens pas sur l'exemple des 10000 fenêtre s', c'est vrai que la BNF est une passoire thermique, donc nous venons en aide à ces établissements les plus en difficulté, demande de retrait puisque vraiment c'est pris en compte, plus 8 7 millions, dont 5 millions pour l'inflation. Donc je mes voix cet amendement double avis défavorable qui est pour, qui est contre, qui savent ce n'est pas adopté le 523 Monsieur de. Merci madame la présidente, on revient sur les aides à la presse avec un amendement qui puisse énormément d'appels ah les aides à la presse, on trouve beaucoup dédié à la presse nationale, la presse régionale, quotidienne et hebdomadaire, mais il y a quasiment rien pour la presse régionale mensuelle, bimensuelle bimestriel ou trimestriel que c'est quasiment rien, c'est pas une image sur les 197 millions d'euros au total d'aides à la presse les publications régionales périodiques non quotidienne ou hebdomadaire bénéficie uniquement des crédits alloués à la 3ème, section soit 50000 euros, sa copine lorsque l'on regarde dans le détail, on s'aperçoit que le montant est si faible que seulement 6 Ty Tryon eu accès en 2022, ce chiffre est surprenant car alors se consulte la liste des publications d'information politique et générale régionale autre que quotidienne et hebdomadaire publié par la CPP AP on, on s'aperçoit que celle-ci contient 138 publications sur le territoire : 6 titres sur 138 il y a un ras-le-bol qui commence à s'installer chez certaines publications un sentiment que les aides sont focalisés sur les titres proches des lieux de pouvoir sur ceux qui maîtrisent le système il y a surtout le sentiment qu'il faut revoir d'urgence les procédures d'attribution des aides du ministère pour être éligible aux aides au pluralisme, il faut remplir 4 critères que ces 138 remplissent toutes tous un taux si faible attribution n'a donc pas compréhensible, ces journaux n'ont pas les moyens et les ressources humaines nécessaires pour disposer d'effectifs, spécialisé dans les relations avec votre ministère, donc il est temps de leur simplifier la vie, c'est l'objet de notre amendement qui doublent le montant alloué à l'aide à la pluralité pour ces publications afin de d'éveiller les consciences au sein du gouvernement et l'inciter à revoir d'urgence ses procédures d'attribution. Qu'est l'avis de la commission. Retrait ou défavorables, notre collègue dit lui-même : 138 titres 50000 euros ça fait donc 500 euros par titre même pas donc c'est c'est très symbolique, moi je préfère franchement qu'on aboutisse, comme on l'a souhaité à une vraie réforme à une vraie remise à plat des aides à la diversité, de manière à ce que le gouvernement prenne un certain nombre d'engagements, mais reconnaissez, chers collègues, que 50000 euros pour 100 38 titres sur la diversité en région, c'est, c'est c'est oui, oui, mais ça c'est symbolique, je l'entends bien c'est un amendement d'appel mais je j'attends plus du gouvernement une remise à plat des aides. Madame la Ministre même avis

Qui est contre. Ils sont adoptés, nous allons procéder l'examen des amendements sur les crédits du compte spécial avances au deux le public

lors du précédent quinquennat le financement de l'audiovisuel public a perdu 200 millions d'euros et lors du PLFR 2022 il a été bouleversé par une réforme menée à la hussarde cette année en plein contexte inflationniste, le budget de France TV n'augmente que de 1 % alors que la société voici charge augmenté de 95 millions d'euros ses concours financiers n'augmente que de que 50 7 millions d'euros, il est donc impératif pour conserver un service public de qualité, de lui assurer des ressources suffisantes et pérennes et lui donner de la visibilité pluriannuelle des ressources Gaudy visuel. Vous pouvez défendent les deux en même temps, s'il vous plaît. Tout à fait, cet amendement est un amendement d'appel pour alerter sur le que représente la réforme du financement de l'audiovisuel public pour les sociétés de l'audiovisuel public 22 millions d'euros supplémentaires pour France TV un coût supplémentaire non amorti par l'État, ce fut une réforme menée à la hussarde lors du PLFR 2022 à tel point que l'on constate après coup que les nouveaux crédits n'étaient pas assujettis à la TVA des sociétés se retrouve assujetti à la taxe sur salaire 22 millions donc on passait par l'État, nous demandons que l'État compense cette perte mais surtout cet épisode doit nous alerter et surtout alerter le gouvernement sur les conséquences de réformes menées un peu trop vite. Madame la présidente, chers collègues, je commencerai par le deuxième parce qu'en réalité il est satisfait : vous demandez 22 millions d'euros destinée à compenser l'assujettissement à la taxe sur les salaires, il est satisfait, puisque le projet de loi de finances prévoit, comme pour tous les autres sociétés de l'audiovisuel public une compensation intégrale de la taxe sur les salaires versés par France Télévisions à hauteur de 22 4 millions d'euros, donc votre amendement est pleinement satisfait par le PLF sur le premier amendement le 506 bon vous demandait 45 millions d'euros de plus sur France Télévisions que vous sur France Médias Monde c'est-à-dire quand même que vous prenez 20 % des crédits complet de de France Médias Monde pour France Télévisions, comment vous dire, vu les difficultés de France Médias Monde je compense sérieusement pas qu'on puisse baisser les crédits de France Médias Monde, aussi important soit-il sur sur cet ensemble et dans ces conditions, un avis défavorable de la ministre. Merci madame la présidente, madame la sénatrice je je rejoins l'avis du rapporteur pour ce qui est de la compensation des effets fiscaux des effets de l'inflation du changement de de du mode de financement, j'ai répondu l'engagement a été tenu, là j'ai le sentiment que vous voulez, en quelque sorte rattrapé les années de baisse du précédent quinquennat sauf que ces économies qui ont été faites, finalement, elles ont pu être faites avec une ambition maintenu pour l'information pour la qualité des documentaires, des enquêtes pour la qualité de l'audience numérique et d'ailleurs, des synergies nouvelles ont eu lieu aussi entre Radio France et France Télévisions, on a pu voir France Info par exemple naître France 3 France Bleu, aujourd'hui, donc on voit bien que ces économies non pas impacté ni les audiences ni l'ambition de l'eau Dusep public et ce sont ses ambitions qu'il nous faut regarder aujourd'hui pour l'avenir par rapport aux défis de l'avenir dont j'ai parlé rapidement dans mon propos liminaire et et Lyon d'abord cette discussion sur les objectifs avant d'avoir la discussion sur les moyens pour la trajectoire pluriannuelle que j'ai souhaité pour 5 ans dans les nouveaux contrats d'objectifs et de moyens, demande de retrait sinon défavorable. Très bien, monsieur Assouline. Oui, non, on ne peut pas nous dire en fait que toutes ces baisses gigantesque depuis 4 ans, c'était finalement bien puisqu'elles ont l'audiovisuel public a rempli sa mission de façon extraordinaire, parce qu'en réalité, ils l'ont rempli à la sueur du front, on les a mis à l'os, mais maintenant on sait très bien que si on ne rattrape pas un certain nombre de retard, les investissements nécessaires pour être compétitif, puisque c'est un domaine qui coûte très cher : la révolution numérique, ça coûte cher pour être à au niveau des plateformes et pour être dans une situation de concurrence donc considérer que finalement tout ça est amorti et que maintenant tout va bien, non, ça va mal, et y compris le service public ne va plus pouvoir continuer, même ceux qui faisaient avant, par exemple sur le sport quand Amazon arrive, vous allez voir si on peut être à la hauteur pour Roland Garros par rapport aux offres qui mettent sur la table et cetera, et cetera, donc il faut une augmentation, ceci dit, nous avons nous proposé 2 amendements dans la première partie du budget sur les recettes pour permettre d'augmenter à cette hauteur, effectivement et ce rattrapage que vous réclamez pour France Télévisions, c'était un amendement qui allait chercher un supplément de recettes un amendement structurelle qui, proposer une alternative au fonctionnement par la TVA, avec une contribution progressive mais en aucun cas, nous pensons qu'aujourd'hui cette nécessité de de rattrapage du manque pour l'audiovisuel public ne peut se faire au détriment et à budget constant sur l'audiovisuel extérieur, aujourd'hui plus que jamais dans l'audiovisuel, il faut renforcer l'audiovisuel extérieur, qui est aussi alors, et dans la situation de guerre en Ukraine de crise internationale, c'est certainement pas là qu'il faut baisser la gare l'information, c'est d'abord dans ce domaine. Je vais donc mettre aux voix cet amendement 506 qui a reçu un double avis défavorable qui est pour. Je retire les deux amendements et les deux oui, OK, très bien, merci, je suis saisi d'une demande de scrutin public par le groupe, les républicains sur les crédits du compte spécial avances à l'audiovisuel public. Je vous rappelle que l'avis de la commission est favorable. Le scrutin est ouvert.

On laisse tomber, plus personne ne demande à voter, le scrutin est clos.

Nombre de votants 344 Nombre de suffrages exprimés 273 pour l'adoption 182 contre 91, le Sénat a donc adopté, je vais suspendre la séance, elle sera reprise à 21 heures 45 pour l'examen de la mission recherche et enseignement supérieur, la séance est suspendue.

Merci